Séance. Est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Il y en a-t-il en séance. Je n'en vois point. Le compte rendu analytique donc. Est adoptée. Sous les réserves d'usage. Madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, je voudrais simplement rappeler que le Sénat hier a rendu un hommage à nos policiers. Tués dans un terrible accident hier et manifesté sa solidarité. Et aussi c'est penser à l'infirmière du CHU de Reims. Assassiné. je dois dire que ça doit être l'occasion de de nous rassembler au sourde un certain nombre. De valeurs, je voulais le le rappeler. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance et retransmise en Direct sur Public Sénat et sur notre site d'Internet chacun sera. Attentif au cours de nos échanges, au respect des valeurs essentielles de notre assemblée le respect. Le respect des uns et des autres et et le respect du temps. La parole est au président Jean-Claude Requier. Pour le groupe du Rassemblement démocratique social. Européen. Monsieur le président. Merci monsieur le président, madame, la Première ministre. Je souhaite vous interroger sur votre responsabilité en matière de planification écologique et énergétique. L'urgence climatique n'est plus à démontrer. Nous déplorons s'vos territoires territoire en particulier en Occitanie voire sécheresse et ses salles désormais sans répit. Je souligne aussi que l'on engagement européen nous impose d'accélérer la réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030. En France, disons seulement baissé de 25% depuis 2990 rwandais 55% attendus. Vous avez annoncé lundi dernier un plan d'action avec des objectifs chiffrés. Mon groupe est très attentif à ces cibles. Nous souhaitons avant tout que l'effort soit équitable, juste comme vous l'avez d'ailleurs rappelé

celui de la conversion des outils de production agricole, industrielle ou encore celui de la lutte contre le gaspillage de l'eau, y compris des eaux grises et usé dans les normes d'usage devront être rapidement réviser pour compenser le déficit croissant en au clair. Tout cela va nécessiter un accompagnement conséquent. Je pense en particulier aux collectivités locales qui devront être soutenus pour furent faire face à leurs besoins et de nombreux. En matière de rénovation énergétique des terrains publics les questions des déchets ou de mobilité. Celle-ci bénéficie déjà du Fonds Vert puisqu'il est question de planifier l'écologie le Fonds Vert sera-t-il pérennisé à long terme avec quel montant au-delà des 2 milliards d'euros déjà prévus et quel bilan d'étape. Pouvez-vous en faire. Pour vous répondre à la parole est à madame la Première ministre. je veux tout d'abord à mon tour exprimer toute ma solidarité aux collègues et aux proches des agents décédé tragiquement ces derniers jours et exprimer tout ne tout mon soutien tout le soutien de mon gouvernement aux agents qui s'engagent chaque jour pour nous protéger nous soigner. Assurer l'éducation de nos enfants et parfois malheureusement au péril de leur vie. Alors Monsieur le Président Ruquier en effet hein. Chaque jour, les conséquences du dérèglement climatique deviennent plus visibles et préoccupante. Je pense notamment aux sécheresses de ces derniers mois ou encore aux feux de forêt. Nous avons besoin d'une action forte pour limiter le dérèglement climatique pour nous adapter à ses conséquences inéluctables et pour restaurer notre biodiversité. Nous prenons des mesures sans attendre. C'est le sens du plan eau qui a été présenté par le président de la République ou encore des du renforcement des moyens pour la sécurité civile et je voudrais souligner le Sénat y contribue pleinement avec la proposition de loi pour mieux prévenir les feux de forêt sur laquelle une commission mixte paritaire se réunira prochainement. pour réussir la transition écologique. Nous devons planifier des actions de long terme pour notre biodiversité pour la gestion de nos ressources naturelles et pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, vous le savez, nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux au niveau européen. Nous sommes en avance sur nos objectifs 2019 2023 et nous avons pratiquement rattrapé le retard accumulé sur la période 2015 2018. Mais il nous faut encore accélérer et doubler le rythme de de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Depuis le mois de septembre avec les ministres et l'ensemble des acteurs. Nous avons identifié, secteur par secteur les leviers à actionner pour baisser nos émissions et pour être acceptable, vous l'avez souligné, l'effort doit être justes et équitablement répartis. La moitié reviendra aux entreprises, notamment les grandes entreprises. Un quart sera réalisé par l'État et les collectivités et un quart par les ménages et pour être réussi la transition écologique doit aussi se faire avec nos concitoyens, nous devons les accompagner dans les changements à venir et formés aux métiers de la transition écologique. J'ai réuni lundi un conseil national de la transition écologique pour partager nos objectifs, secteur par secteur et dans le courant du mois de juin, nous serons en mesure de présenter une planification écologique complète. Mesdames, et messieurs les sénateurs, hein. Réussir la transition écologique, c'est aussi nous adapter et anticiper tous les cas de figure, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a annoncé le week-end dernier le lancement de travaux pour préparer la France en cas de hausse des températures de 4 degrés. Que ce soit pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour nous adapter aux effets inéluctable du dérèglement climatique ou pour restaurer la biodiversité. Nous avons besoin des collectivités de nombreux projets concrets se mettent en place, notamment grâce au soutien du Fonds Vert se font, ce sont 2 milliards d'euros dès cette année et je vous confirme comme je l'avais annoncé que ce fonds sera pérennisé. Je vous remercie.

Merci la parole est à notre collègue Jacques verdict pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Merci monsieur le président, monsieur le ministre des Transports Clément Beaune. Justement, si on veut gagner tous ensemble. Est-ce vraiment le moment de saper le fret ferroviaire publique comment, Monsieur le Ministre. Peut-on fixer les trajectoires du plan climat. Comment peut-on viser le report de la route vers le rail et acceptée en même temps que fret SNCF. L'acteur public majeur de cette transition indispensable soit dépecé démantelé. La Commission européenne par sa procédure contre la France pour aide d'État soi-disant illégale ah fret SNCF mettent en péril la survie même de cet acteur essentiel à la mutation des transports, Monsieur le Ministre, ce n'est pas par des procédures technocratique par l'application aveugle d'une doxa libérale que l'Europe réussira mais par sa capacité à concrétiser son Green Deal à atteindre un objectif européen 2030 du fret ferroviaire à 30% de part modale la France on est encore loin. Ça commence à bouger. Ne laissons pas briser cet élan entre la cause du climat et celle de la concurrence, le choix est est une évidence, Monsieur le Ministre, plutôt que de tenir cette ligne résolu vous préférez en prendre votre parti et consentir à en finir avec fret SNCF telle qu'il existe aujourd'hui le liquider pour lui substituer avec 2 entités une structure assez différentes pour que la DG Concurrence admettent la discontinuité économique comme ils disent et donc renonce à exiger le remboursement des aides abandon des trains complets de 500 emplois. Garanties sociales et salariales en danger sérieux. Ouverture du capital cessions d'une part des locomotives aux concurrents renoncement aux appels d'offres pour des années pour le trafic dédié. Monsieur le Ministre, comment ce scénario de mise à la découpe pourrait-il ne pas briser le rebond ferroviaires nécessaires, serez-vous le ministre des transports qui a liquidé fret SNCF. La parole est au ministre délégué en charge des Transports monsieur Beaune. Merci, merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur faire Nick comme vous je crois très fermement à l'avenir du fret ferroviaire et c'est une part essentielle de notre stratégie de planification écologique et d'ailleurs avec le plan fret qui est déployée depuis maintenant 2 ans, nous avons inversé une tendance historique qui était celle du recul de la part du fret ferroviaire dans le transport de marchandises en France pour la première fois depuis 2015, cette part est en train de réaugmenter et nous ne lâcherons pas cette ambition que nous partageons je crois tous ici. Pour cela, il faut en effet à l'opérateur public de référence du fret ferroviaire et je suis bien déterminé à le maintenir. Quelle est la situation, Monsieur le Sénateur par il faut dire la vérité sans facilité et sans démagogie pour préparer l'avenir. C'est que il y a en effet une procédure qui a été ouverte publiquement le 18 janvier dernier par la Commission européenne. Après plusieurs échanges avec la France. Je me suis occupé de ses dossiers. Dès mon arrivée au ministère des transports, il y a un peu moins d'un an, j'ai tout fait, nous avons tout fait, du côté des autorités françaises pour empêcher l'ouverture cette procédure pour contester comme vous venez de le faire. Les aides réputé illégal sur la Commission européenne versé pendant 15 ans par les gouvernements successifs ah fret SNCF. La procédure a été engagée et donc nous avons aujourd'hui un choix qui est simple et claire et que nous devons partager soit nous disons que nous allons en effet jusqu'au bout de cette procédure, c'est une possibilité mais disons-le aussi, très franchement, le risque est simple et c'est une quasi-certitude c'est la mort totale et cette fois la liquidation de fret SNCF 4800 salariés et des milliers de kilomètres aujourd'hui de rails et de fret ferroviaire en France. Je ne veux pas de cette solution et donc oui j'assume que en responsabilité pour le pas mettre en danger les femmes et les hommes du fret ferroviaire pour garder un groupe public de fret ferroviaire qui a un avenir et que nous soutiendrons. Nous devons trouver le plus rapidement possible un accord pour mettre fin à l'incertitude et éviter la mort de cet opérateur. Nous aurons l'opérateur public. Nous aurons un opérateur qui ne sera pas privatisée qui gardera l'immense majorité de ses activités sans aucun licenciement évidemment et sans aucun report modal car j'y suis engagé, nous réinvestissons en même temps dans le fret ferroviaire de manière totalement inédite. Nous amplifions encore le plan déployés depuis 2021 pour renforcer cette ambition. Monsieur Véronique. Oui, Monsieur le Ministre, vous vous disait ne pas vouloir mettre en danger. Vous avez parlé de jouer à la roulette russe. L'avenir du fret ferroviaire. Mais dans quel jeu risqué langage et vous en croyant qu'avec une telle désorganisation les chargeurs, les acteurs économiques ne retourneront pas à la route ne resteront pas dans les camions. La parole est à notre collègue Dany Wattebled pour le groupe les indépendants République et le territoire. Monsieur le président, monsieur le ministre de l'Intérieur. Mes chers collègues. Notre pays traverse une semaine noire. Hier matin, nous apprenions au décès d'une infirmière sauvagement agressé. Dimanche matin. Paul Manon Steven ont succombé à un accident du lance-inouïe. Dans l'exercice de leurs fonctions dans le nord. Ces 3 policiers de moins de 25 ans était au début de leur carrière et avait toute la vie devant. L'un d'entre eux étaient pas de familles d'un enfant de 11 mois, tandis qu'un autre allait devenir père. Monsieur le Ministre. Vous êtes venu rencontrer leurs collègues lundi et les Nordistes vous en remercie. Le groupe les indépendants veulent veulent rendre un vif hommage. Et mais Power leurs pensées vont à l'ensemble de ces familles meurtries et à l'âge de l'encens l'adolescente qui avait le secourir. Après la douleur. Et la colère, viendra le temps des questions. On sait désormais que les 2 occupants du véhicule ayant percuté ces fonctionnaires. Sont connus pour usage de stupéfiants et d'alcool. On apprend ensuite que le chauffard conduisait sous l'emprise de ces substances. Les policiers, gendarmes et pompiers ces héros du quotidien sont de plus en plus confronté à des violences insupportables. Et intolérables. Lors de leur intervention. Comme de, de nombreux événements récents nous le rappelle à chaque drame. L'émotion est plus forte. Ce climat d'hostilité nourrie par le silence assourdissant de certains soucieux. D'entretenir une atmosphère de défiance envers les forces de l'ordre. Ces femmes et ces hommes le garant, sont les garants de l'Ordre Républicain. Il mérite une protection et un soutien encore plus fort et surtout intangible. Mais il faut que la justice suive. Monsieur le Ministre, je veux dire c'est de questions, quelles mesures entendez-vous prendre afin de soutenir et de campagne et les familles des victimes dans cette période. Pouvez-vous nous dire comment le gouvernement entend poursuivre son action pour soutenir nos forces de sécurité intérieure contre les multiples menaces auxquelles elles sont confrontées. Secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. Vous avez la parole. Madame le ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Houat Bali. Effectivement, vous l'avez dit, le métier, les métiers de policiers et de gendarmes, sont des métiers de plus en plus difficile. Eu égard aux exigences légitimes de nos concitoyens et aux risques et aux menaces qui pèsent sur eux. Ils ont besoin de tout notre souci soutien pardon et à ce titre je me joins aux hommages qui ont été rendus à l'Assemblée nationale et ici même et par la Première ministre aux 3 policiers qui sont décédés. La semaine dernière dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis le 1er janvier dernier, ce sont 2380 gendarmes et policiers qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Et on peut souligner la ce policier blessé lors de la manifestation du 1er mai. Par un cocktail Molotov et tous ceux qui ont été blessés dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines. Le Parlement a voté la Lopmi et et il m'appartient de de vous remercier qui a doté la police et la gendarmerie de moyens exceptionnels des moyens humains et budgétaires d'abord avec 15 milliards d'euros supplémentaires et des moyens statutaires qui permettent de valoriser et de mieux prendre en compte la carrière de nos, de nos militaires, de nos gendarmes et de de nos policiers, nous entendons bien bien évidemment et c'est l'objet de votre question poursuivre nos efforts pour mieux protéger les policiers, les gendarmes. C'est déjà en cours de déploiement, puisque ce sont des caméras piétons qui sont développés qui sont déployés pardon dans tous les commissariats, c'est une protection fonctionnelle, qui est facilité c'est une cellule d'assistance

Nous avons également et grâce au soutien du Parlement crée le délit spécifique. De de violences volontaires sur argent sur agent pardon, chargé de la sécurité intérieure et de protection des agents en bord de route. La Lopmi a également créé 20 postes de psychologues qui permet d'Akon. Pardon d'accompagner au mieux les policiers et les gendarmes, le ministre de l'Intérieur est très attentif à la protection des forces de sécurité intérieure avec l'aide du Parlement. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Christine Lavarde. Pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Ministre, 2023 mois de mars avec la plus faible natalité depuis 1994 2022 années avec la plus faible fécondité depuis 1946. Pourquoi les Français ont-ils moins d'enfants. On pourrait penser à l'éco-anxiété. On pourrait surtout penser au problème du logement. Cela fait des mois que les élus locaux vous alerte sur la crise du logement et pourtant le Conseil national de la refondation consacrée à ce sujet a été reporté sine die. Il devait se tenir le 9 mai. On pourrait penser au manque de moyens financiers sous François Hollande le quotient familial, les allocations familiales ont diminué sous Emmanuel Macron, les allocations familiales ont été faiblement revalorisé la CMG a diminué alors que les 1000 premiers jours. Alors qu'il existe des excédents. La branche famille hein. Virgil 9 milliards d'excédent en 2022 à près de 9 milliards en 2021 5, 8 milliards d'erreurs comptables. Le constat est sévère la sentence sans appel, la Cour des comptes a refusé de valider les comptes de la branche famille pour 2022 mais aussi difficultés à faire garder les enfants de moins de 3 ans alors que les 1000 premiers jours avait été érigé comme une priorité. Aucune des préconisations du rapport Cyrulnik n'a trouvé une traduction législative ou réglementaire. La conférence des familles de 2022 annoncent un droit opposable à la garde pour 2027, un rapport de l'IGAS du 11 avril dernier dénonce la baisse de la qualité d'accueil la restitution du CNR, petite enfance, prévu au mois de mars reportée, elle aussi. La Coges la future coches est toujours en cours de discussion. Elle sera donc connue des acteurs avec au moins plus de 3 mois de retard. Le constat est sombre. Alors Monsieur le Ministre qu'allez-vous proposer au président de la République qui semble enfin s'inquiéter des chiffres alarmants de la natalité. Pour vous répondre. La parole est au ministre des solidarités. De l'autonomie, personnes handicapées. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice l'Avare vous aborder plusieurs questions dans votre question, je voudrais revenir d'abord sur la question de la non-certification des comptes par la Cour des comptes, des comptes 2022 de la branche famille de la Sécurité sociale qui nous interroge à la fois sur les difficultés qui ont pu conduire à cette non certification qui remet pas en question. D'ailleurs la bonne tenue des comptes de la branche mais. Qui dénonce un certain nombre de problématiques, en matière de contrôle interne de la branche auquel nous veillerons à remédier à la fois en travaillant sur la sécurisation du système. Avec le projet de solidarité à la source pour veiller à une meilleure, des prestations sociales à une simplification en luttant contre le non-recours en une du temps contre la fraude et en luttant contre les indus dans la branche et vous abordez une 2ème question qui est celle de la question de la natalité. Dans notre pays. Alors vous le savez, le taux de natalité aujourd'hui il est proche de 1,8 enfants par femme. C'est un taux de natalité qui est en forte baisse et qui ne permet pas le renouvellement des générations dans notre pays qui doit tous nous inquiéter parce qu'il pose un certain nombre de problèmes, notamment il fait peser sur notre système de protection sociale des tensions qui sont extrêmement forte et donc mon rôle en tant que ministre des familles et de la petite enfance, c'est aussi bien de répondre aujourd'hui à l'envi des familles de pouvoir avoir des enfants dans notre pays puisqu'on sait que le désir d'enfant est d'environ 2, 4 enfants ce que nous, nous pensons, c'est que avant de penser augmenter les prestations ou les allocations familiales pour pouvoir favoriser. Ce voilà ce cette réponse à ce désir d'enfant, c'est d'abord d'améliorer les services aux familles et comme vous l'avez dit, l'une des premières préoccupations aujourd'hui des familles dans notre pays, c'est de savoir comment elles vont pouvoir faire garder. Leur enfant, on le sait il manquerait environ 200.000 places d'accueil. Du jeune enfant. Le président de la République s'est engagé à mettre en place ce service public de la petite enfance. La Première ministre fera des annonces dans les jours qui viennent pour vous dire comment nous répondrons à cette question. Alors vous ne m'avez absolument rien proposé pour autant des idées. Nous, nous en avons par exemple prendre en compte la taille des logements familiaux dans la comptabilisation SRU. Supprimé la modulation des allocations familiales. Supprimer la tarification horaire de la su qui est complexe et qui engendrent nombre de fourre-tout donner un véritable pouvoir de sanction au PMI. Monsieur le Ministre à chaque enfant qui naît le monde recommence une politique familiale ambitieuse et la meilleure réforme des retraites. Vous disposez de 6 milliards pour financer cette politique. La parole est à notre collègue Stéphane Demilly pour le groupe. Si de l'Union centriste. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, je souhaite vous parler d'un sujet de fond très grave. Mais permettez-moi de le faire par le biais d'une rhétorique un peu inhabituelle, celle d'une charade une charade intitulé je fais ce que je veux quand je veux comme je veux et où je veux. Mon 1er est une manifestation dite musical interdite par deux arrêtés préfectoraux. Mon 2ème a réuni, malgré l'état de droit dans lequel nous vivons. Plus de 30.000 personnes dans un petit village de l'Indre, qui a subitement vu sa population multipliée par 273. Pour devenir l'espace d'un long week-, la capitale de la rave Party. Mon 3ème. Malgré la mobilisation de 320 gendarmes s'est soldée par plus de 500 prise en charge par les services de secours dont 30 évacué en urgence absolue. Mon 4ème a généré 15 tonnes de déchets dans le terrain privé d'un propriétaire qui a vu converger en quelques heures, sans en être averti une marée humaine de teufeurs et mon tout, Monsieur le Ministre, apporte de l'eau au moulin de ceux qui s'inquiètent du délitement de l'autorité de l'État. Monsieur le Ministre, cet épisode du Teknival est loin d'être isolé. D'autres départements, y compris le mien ayant dû subir cette dictature de l'urgence et de la masse. Je sais bien, comme le rappelait Machiavel que le choix est rarement entre le bien et le mal mais entre le pire et le moindre mal, mais j'ai néanmoins de questions à vous poser à propos de cet épisode affligeant. La première et peut être naïve, mais comment se fait-il que tout le monde était au courant de ce rassemblement, sauf ceux qui devait l'être. Ma 2ème question Eduardo pragmatique pour dissuader ce genre d'événements illégaux et dangereux. Sans parler de l'alcool et de la drogue. Ne faut-il pas durcir les sanctions contre les organisateurs qui aujourd'hui individuellement ne risque rien, si ce n'est 1500 euros d'amende. Monsieur le Ministre ces images de tant de désinvolture ont une résonance terribles dans l'opinion publique, mais je pense que vous le savez. Pour vous répondre. La parole est à la secrétaire d'État. En charge de la citoyenneté. Madame Backès. vous nous interrogez sur le rassemblement festif musical du 17 mai dernier. Baptisée Teknival French Tech 2023 et comme vous l'avez dit, il a été non déclarés aucune demande d'autorisation n'a été fait. Les renseignements territoriaux puisque c'est votre première question avait bien identifié l'organisation en cours d'une manifestation de ce type dans le centre de la France mais et vous le savez aussi le lieu exact a été défini quelques heures avant le rassemblement et ce sont en quelques heures, jusqu'à 25.000 personnes qui se sont réunis sur le site et dans l'urgence ont été organe a été organisé cet cet événement pardon alors que et vous l'avez dit, les conditions ne s'y prêtait absolument pas ni d'un point de vue sanitaire, ni d'un point de vue de la sécurité. Sous l'autorité du préfet et en urgence et je veux remercier les services de l'État qui se sont rendus disponibles est rendue extrêmement efficace pour accompagner cette manifestation, les moyens de la préfecture des services de l'État ont été mis en place les services du du département avec notamment la mobilisation des sapeurs-pompiers et des associations de sécurité civile. Le préfet a coordonné un dispositif opérationnel pour garantir l'ordre public avec succès et pour garantir d'éviter la circulation de festivaliers qui sortait sous l'emprise de l'alcool. Nous avons renforcé les moyens de manière significative. Vous avez parlé de 320 gendarmes, ce sont 434 gendarmes qui ont été mobilisés sur l'opération pour empêcher tout droit tout trouble majeur à l'ordre public et nous pouvons, je crois, tous ensemble, souligné le bilan de l'opération avec 30.200 personnes et traite 13.300 voitures qui ont été contrôlés, 155 verbalisations pour conduite en état d'ébriété 32 verbalisations pour stupéfiants la saisie de 300, 300 grammes de cannabis d'un kilo d'herbe de cannabis de 40 grammes de cocaïne et cetera et cetera. Nous avons également saisi les groupes électrogènes et les organisateurs pour la plupart ont été identifiés. Les procédures sont en cours et ils seront bien évidemment sanctionnés. Je vous remercie. La parole est notre collègue Michelle Gréaume pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'économie. Voilà plus de 60 jours que des salariés de Vert Baudet dans le Nord sont en grève. Pour rappel, cette usine est composé majoritairement de femmes. L'entreprise Vert boudé l'une des 59 entité détenue par le fonds d'investissement et Keystone un fond de dimension européenne. L'examen du bilan financier de l'entreprise est édifiant. Entre 2018 et 2021. La marge nette est passé de moins 0,7% à plus de 3,6% la valeur ajoutée de 49. 7 millions à 56,6 millions d'euros et sur la même période, la part des salaires par rapport au chiffre d'affaires est passé de 15 jours à 12. A % l'unique revendication de ses salariés est une augmentation de salaire de 150 euros. Tous les chiffres montrent que cette revendication est légitime. Actuellement l'inflation les les rattraper les fins de mois sont difficiles depuis deux mois, pas de dialogue avec la direction des propos sexistes à leur Intervention des forces de police intimidation à la menace de licenciement, tout y passe. Les salariés sont déterminés, leur lutte devient emblématique. Les salaires dans l'entreprise varie entre 1300 et 1500 euros mensuels. Malgré leur ancienneté quand le dirigeant perçoit une rémunération de 60.000 euros par mois. Cette grève met en lumière une question centrale, comment faire ses choix de vie sans un salaire digne. Comment être véritablement libre sans indépendance économique. La solidarité, le soutien de tout le monde du travail s'exprime, y compris financièrement et quelque part cette lutte est devenue celle de tous les salariés du pays par procuration. Mais les 2 ministres vous prétendez appeler au partage de la valeur. Il n'y a-t-il pas avec eux vers bouder une belle occasion de sa mise en oeuvre. Merci. Pour vous répondre. La parole est ministre du travail. Merci monsieur le président. Merci mesdames et messieurs les sénateurs Madame la sénatrice. Vous évoquez le le conflit social en cours au sein de l'entreprise Vert Baudet et plus particulièrement dans l'établissement situé dans votre département. ce conflit social est bien connu des services de mon ministère et mon cabinet. Il a été ouvert autour du 20 mars et. Un accord a été signé d'accord majoritaire sur lequel vous pouvez avoir une appréciation signé par 2 organisations syndicales Force ouvrière et la CFE-CGC en soulignant que ces 2 organisations représentent lors des dernières consultations 63% des suffrages exprimés dans l'entreprise, la CGT n'a pas souhaité signer cet accord et a laissé le mouvement se poursuivre et encourager sa poursuite dès le 9 avril. Les services de la direction départementale de l'économie de l'emploi, du travail et de la solidarité ont initié de médiation cette médiation s'est traduite par une première décision de l'entreprise, en l'occurrence 30. Embauches 30 recrutement de personnel en intérim dont le la mission d'intérim a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er mai dernier l'accord qui a été conclu fin mars prévoit une augmentation de la rémunération, mais il est vrai pas par une voie salariale par la mise en oeuvre de de primes et d'autres modalités de rémunération. depuis il y a un certain nombre de contacts qui ont été initiés et mon cabinet a notamment permis un échange et un rapprochement entre le cabinet de la secrétaire générale de la CGT, madame Binet et la direction générale de l'entreprise. Une réunion s'est à nouveau tenu lundi dernier il y a 3 jours avec des propositions nouvelles de la direction que la CGT a à nouveau refusé à l'heure où nous parlons, il y a environ 70 salariés sur les 340 que compte le site, qui sont toujours en grève. d'autres réunions sont prévues, je souhaite évidemment que le dialogue social permette cet aboutissement dans le respect des prérogatives de fac chacun dans le respect aussi de l'accord majoritaire qui a été signé il y a maintenant quelques semaines je termine d'un mot, monsieur le président pour dire que madame la sénatrice a évoqué l'intervention de la police pour. Enlever et faire ôter les les points de de grève les piquets de grève. Cette intervention de la police à la demande du préfet de région a été faite en application une ordonnance rendue par le tribunal saisi par l'entreprise, il y a plusieurs semaines. Merci la parole est à notre collègue Michel Dagbert pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Merci monsieur le président, ma question s'adresse au ministre chargé des Transports Clément Beaune et porte sur le fret ferroviaire, comme quoi dans cet hémicycle on peut poser deux fois la même question, mais sous un prisme différent subissant la forte concurrence de la route. La part du rail dans le transport de marchandises n'a cessé de diminuer durant ces dernières décennies. Elle est ainsi divisé par 2 entre 2006 et 2019 pour passer de 20 à 10%. C'est un fait, c'est une réalité. Les avantages du fret ferroviaire sont pourtant indéniables faisant de celui-ci, un formidable outil de la décarbonation des activités économiques. Un train de marchandises équivaut à 40 camions il réalise près de 10 fois moins d'émissions de CO2 et consomment 6 fois moins d'énergie à la tonne transportée que le mode routier, ça aussi c'est un fait. Le conseil d'orientation des infrastructures dans ses différents rapports a d'ailleurs souligné l'importance qu'il y avait à le développer aussi le gouvernement a affiché à plusieurs reprises sa volonté et vous l'avez rappelé. Monsieur le Ministre, de soutenir le transport de marchandises par le rail, l'objectif d'un doublement de la part modale du fret d'ici 2030 a été inscrit dans la loi climat et résilience du 22 août 2021. De plus, une stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire comportant 72 mesure a été présenté et 170 millions d'aide supplémentaires par an ont été alloués. Ce soutien additionnel sera prolongé jusqu'en 2027. Dans ce contexte, les difficultés rencontrées par la filiale de fret de la SNCF. En effet inquiète puisque la Commission européenne et ça été rappelé à démarrer une procédure en janvier aussi je sais l'investissement qui est le vôtre, Monsieur le Ministre, pouvez-vous annoncer. Les mesures que vous avez annoncé hier et nous dire le calendrier de la mise en oeuvre de ce dispositif visant à à faire. Perdurer le fret SNCF et à rassurer ses salariés. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Dacbert. Je le redis, nous vivons une situation difficile au regard de cette procédure engagée par la Commission européenne et je le réaffirme parce que le sujet d'une grande gravité. Je ne ferai pas le choix de la facilité qui consisterait simplement à passer le dossier au suivant et à verser dans quelques mois ou quelques années des larmes de crocodile sur l'entreprise qu'on aurait laissé mourir par démagogie et donc je veux régler cette situation aujourd'hui. D'ici la fin de l'année pour répondre très précisément à votre question par un accord. Oui un accord exigeant avec des lignes rouges très précises évidemment la préservation intégrale de l'emploi, aucun licenciement et la préservation dans un opérateur public ferroviaire dont l'avenir est viable de plus de 90% des effectifs actuels. Je crois que c'est une mesure très importante sans aucune privatisation. Il est évident qu'il doit y avoir un capital public au sein d'un groupe ferroviaire qui est celui de la SNCF et sans aucun report modal car vous avez rappelé les avantages du fret ferroviaire. Nous en sommes convaincus, et un train de fret, c'est l'équivalent de 40 camions, c'est 10 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes le gouvernement qui a enfin redressé la part du fret ferroviaire en France. Nous continuerons cela et ce que je propose, ça n'est pas une solution du moindre mal, ça n'est pas un avenir au rabais, c'est un avenir sérieux et positif pour le fret ferroviaire publique et privée en France car nous aurons besoin de beaucoup d'opérateurs pour développer ce mode de transport et c'est pour cela que nous avons annoncé, sous l'autorité de la Première ministre un plan amplifié et accéléré pour le fret, 200 millions d'euros seront alloués dès la fin de l'année prochaine pour l'aide au wagon isolé pour les aides à l'exploitation pour les opérateurs de fret notamment l'opérateur de fret ferroviaire publique c'est une visibilité donnée jusqu'à 2030 pour garantir les investissements et le redressement de la part du fret ferroviaire en France dans les contrats de plan État-Région, ce seront 2 milliards d'euros qui seront mobilisés en investissement 4 fois supérieur à celui que nous avons vécu sur la période précédente de contrat de plan État-Région pour investir dans le Gare de triage pour investir nos lignes de fret, c'est un effort qui n'a jamais été fait dans notre pays et nous prolongerons de 2 milliards d'euros supplémentaires jusqu'au début de la décennie C'est donc un effort dans la durée, un effort sérieux. Je ne veux pas qu'on vive dans l'incertitude. Je veux qu'on prépare l'avenir avec les salariés du fret ferroviaire public français. Merci la parole est à notre collègue Martine Filleul pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, monsieur le Président, je souhaitais à mon tour, rendre hommage aux trois policiers de Roubaix, décédé dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai une pensée pour la famille et à laquelle je sais s'associe l'ensemble de cet hémicycle. Monsieur le Ministre, depuis 2 mois les 72 salariées de Vert Baudet demandent à pouvoir vivre dignement du fruit de leur travail pour beaucoup des femmes en grève pour la première fois de leur vie. Face au refus catégorique de la direction d'augmenter les salaires. Un compromis dans la douleur a été trouvé. 0% d'augmentation salariale, mais des primes des socialiser le délégué CFDT le dis très clairement. C'était cela ou rien. Le 0%, on l'a très mal vécu alors grévistes ou non, personne ne peut trouver normal qu'après 20 ans de boîte. Les salaires plafonne au SMIC au moment où tout augmente, je partage l'inquiétude de ces femmes salariées grandes perdantes de la réforme des retraites, de ne pas voir abonder leur pension avec ses primes. Face à un blocage de cette nature. La réponse ne peut être celle de l'intimidation et de la violence mais vers Baudet n'est qu'un exemple parmi d'autres. Durant la période du Covid. Vous nous expliquiez la main sur le coeur qu'il n'y a qu'il y aurait un avant et un après pour les travailleurs de première ligne, alors allez-vous continuer à adresser des voeux pieux au patronat à coups de demande ou bien allez-vous enfin endosser le rôle d'un État qui met réellement pratique le partage juste de la valeur on se plaçant aux côtés des travailleurs. Pour vous répondre à la parole était ministre du Travail, du fait de l'emploi de l'insertion, monsieur Dussopt. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Sophie elle. Je je je complète les propos que j'ai tenu il y a quelques instants. Réponse, madame la sénatrice. Mais peut être pour évoquer de points. 1er point, vous avez parlé d'intimidation et de violence et je suppose que vous faites référence. À l'agression qui a subi un des délégués CGT de de l'entreprise en question. Le délégué CGT en question été reçue par les représentants de la préfecture et il lui a été vivement conseillé vous l'imaginez, de décider de déposer plainte à l'heure où je m'exprime devant vous, et à ma connaissance, cela n'a pas été fait et il les responsables de la préfecture se sont même heurté à un refus de dépôt de plainte. Vous évoquiez, madame la sénatrice. L'accord intervenu à la fin du mois de mars. Je vous confirme, mais vous en connaissez la teneur que cet accord prévoit une prime à hauteur de de 650 euros de mémoire ainsi qu'un certain nombre de dispositions relatives à la rémunération, sans qu'il y ait d'évolution salariale particulière. Vous dites l'État doit jouer son rôle. Nous le faisons dans le respect du prérogatives des prérogatives. Des acteurs du dialogue social à la fois par une médiation locale par une intervention toujours sous forme de médiation et de prise de contact intervention qui s'est traduite par la réunion que j'ai évoqué il y a un instant, qui s'est tenue avant-hier qui n'a pas débouché sur un accord. Je l'ai dit à Madame, la sénatrice agréable à l'heure où nous parlons, 72 des presque 350 salariés de Vert Baudet sont en grève et maintiennent leur mouvement de grève. Une réunion doit se tenir en toute fin de semaine je pense qu'à un nombre de propositions seront faites et et j'espère, seront de nature à avancer dans la résolution de ce conflit, mais nous sommes face à une situation particulière et je sais que vous entendrez je crois en tout cas cet argument vous nous demandez d'intervenir finalement pour décider à la place de celles et ceux qui sont chargés du dialogue social la l'employeur et les organisations syndicales, il y a eu une décision, vous pouvez porter une appréciation négative sur l'accord intervenu à la fin du mois de mars. Mais cet accord, vous le savez et que, et considéré et à juste titre comme majoritaire puisque signé par des organisations syndicales représentant 63% des salariés concernés. Madame Filleul. Monsieur le Ministre de de votre réponse qui ne me satisfait que partiellement. Car au-delà de l'exemple de Vert Baudet et des volontés de négociation, hé bien il y a il y a une situation nationale qui se pose celle. De la politique salariale Les Français veulent veulent pouvoir vivre dignement de leur travail et aujourd'hui, je regrette que votre gouvernement ne soit pas au rendez-vous de cette attente des Français. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Henri Leroy pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, madame, la Première ministre en 2022, près de 500.000 migrants légaux sont entrés en France établissant un record absolu. être il faut ajouter les immigrés illégaux. Plus de 300.000 selon les estimations de Frontex, l'échec du gouvernement à contrôler l'immigration et pas tant le coût économique de cette immigration est un sujet que le nom peut plus éluder l'aide médicale d'État continue de progresser de plus de 12% cette année pour atteindre un point culminant à 1,2 milliards d'euros et l'accueil des immigrés pèse de plus en plus sur nos finances publiques, le coût social de l'immigration et de moins en moins acceptable. La loi n'est pas respecté les OQTF ne sont pas exécutées. Sans oublier le communautarisme et la violence qui gangrène l'autre société touchant bien souvent les Français les plus modestes. Des solutions existent. Pour reprendre le contrôle de l'immigration, certains pays comme le Danemark, nous démontre qu'il n'y a pas de fatalité, mais encore faut-il en avoir la volonté, l'excellent rapport du sénateur buffet nous manque d'ailleurs la voix en le domaine. Des propositions concrètes ont été faites par les républicains et de propositions de loi dont une constitutionnel offrent de nouvelles perspectives. Madame, la Première ministre, la France va mal, ils vont regarder ailleurs vous préféré temporiser en adoptant une approche du en même temps, cher au président de la République, madame, la Première ministre ma question est simple, quand allez-vous ouvrir les yeux sur le drame qui se joue sous vos yeux et vous emparer sérieusement de ce sujet. Pour vous répondre, la parole. Au ministre de l'Intérieur, les Outre-mer monsieur Gérald Darmanin. comme vous. Nous sommes évidemment préoccupés par les questions migratoires comme partout en Europe, 60% de demandeurs d'asile par exemple se sont présentés à nos frontières et tous les pays, vous l'avez constaté, quelles que soient les régimes politiques quels que soit d'ailleurs le choix qu'ils ont fait en matière migratoire ont les mêmes difficultés. Je vous ferais remarquer quand même c'était pas entre question que depuis le début de l'année, il y a moins de demandes d'asile aujourd'hui qui en a eu depuis les 3 dernières années, contrairement à ce qui se passe chez nos voisins européens puisqu'on est à 110.000 demandes d'asile en moyenne si on annonce de le mois d'avril, et deuxièmement nous avons augmenté l'exécution des OQTF et c'est passé que ce con consulaire de plus de 20% depuis le 1er janvier. Alors vous évoquez des propositions, nous sommes évidemment heureux de les entendre. Nous n'avons pas encore vu les 2 textes proposés par les l'air nous avons compris qu'il ne faisait pas totalement consensus avec les centristes du Sénat qui vont déposer le même je crois des textes, monsieur, le monsieur le sénateur, pour discuter avec l'ensemble de l'échiquier politique et singulièrement avec la majorité sénatoriale, puisque nous avons déposé un texte et vous avez déjà commencé à l'étudier en commission dans les propositions DLR que nous avons lu ce week-end il y a des choses tout à fait concordantes. La fin de la fin de la double peine, par exemple pour les étrangers délinquants l'intégration obligatoire par l'apprentissage du français, la simplification du droit, c'est-à-dire le rapport buffet. Nous avons évidemment beaucoup. De convergences, il y a aussi des différences. Monsieur le sénateur, et notamment des, des, des divergences de principe sur lequel, sans doute, il faut que nous débattions vous proposez pour certaines dispositions de sortir de la Convention de Genève de 1951 de sortir des traités de l'Union européenne de sortir du Conseil de l'Europe de sortir de la CEDH et si c'est tout à fait vrai, c'est une question importante que se ferait Frexit migratoire. Il faut évidemment que nous puissions échanger sur les propositions constitutionnelles mais avouez que c'est si nous faisons un projet de loi ordinaire. Je veux redire que, à la demande de la Première ministre j'ai entrepris des négociations, les discussions avec le groupe LR du Sénat avec les centristes avec tous les autres groupes qui le souhaite bien évidemment pour j'espère à l'automne, discuter de ce texte. D'en parler et de commencer d'être concret, comme vous l'a proposé le gouvernement. Oui, monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous savons que vous êtes un homme d'écoute et que vous nous entendrez mais ma question s'adressait à madame, la Première ministre. 7 Français sur 10 dénonce le trop plein d'immigrés en France. Ils ont ces français des difficultés pour se soigner, pour s'alimenter pour vivre décemment dans un climat d'insécurité ou la violence devient quotidienne, alors madame, la Première ministre et donnez-leur un peu d'espoir. Réagissez merci. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce seront les divers responsables de la ruine de la terre qui organiseront le sauvetage de du peu qu'il en restera et qui après l'abondance gérerons la pénurie et la survie. Voilà ce que prophétisé le penseur Bernard Charbonneau. Il y a 40 ans. Plus 4 degrés Celsius et quand même la catastrophe annoncée sans aucune adaptation possible tout le littoral français sous l'eau, des vagues de chaleur bien au-delà des 40 degrés auquel tout le monde ne pourra pas survivre des sécheresses sévères des pénuries d'eau, des pertes de récoltes. Notre modèle est en cause le perpétuer alors qu'il se heurte à ses limites, relève d'un déni impardonnable notre lutte contre la crise climatique doit s'intensifier car elle va générer des dommages colossaux qui n'en est pas conscient votre mantra pas d'impôt, pas de taxes nous mène dans l'impasse. Nous devons faire en disant ce que nous n'avons pas fait en 30, dit le rapport de Jean Pisani-Ferry qui n'est pourtant pas un dangereux Ekotto éco-terroristes et qui propose entre autres solutions de lever un impôt sur les 10% les plus aisés pour financer la transition écologique. À vrai dire il n'y aura rien d'extravagant à imaginer qu'ils contribuent à cet effort à la hauteur de leurs moyens en effet changer sa chaudière et acquérir une voiture électrique n'est pas à la portée de tous les Français et pourtant la réduction conséquente en gaz à effet de serre et donc l'habitabilité de la planète profiteront à tous une répartition équitable et non seulement la moindre des choses mais relève d'une justice sociale absolument indispensable pour l'emporte pour emporter l'adhésion et l'acceptabilité de tous. Nous n'avons cessé depuis 2017 de vous proposer des mesures fortes comme justement l'instauration d'un ISF climatique en pure perte. Comment envisagez-vous les financements nécessaires au changement radical qui s'impose à nous. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Preville. Le rapport Pisani-Ferry commandé par le gouvernement. Il traite de beaucoup de choses sur les 156 pages. Je note que vous vous concentrez sur les trois qui concerne la fiscalité, vous auriez pu souligner. Qu'il insiste sur la cohérence de la stratégie de planification pour. Portée par la Première ministre. Et en citant très exactement cette phrase du rapport. Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, disant qu'il nous faut faire en disant ce que nous n'avons pas fait en 30 ans, c'est en fait une citation d'Élisabeth Borne qui date d'octobre dernier au moment du lancement du CNR sur le climat et la biodiversité.

D'insister sur la hauteur de la marche sur le chemin qui nous reste à parcourir, plutôt que de donner le sentiment que certains avaient la solution parce que la vérité c'est que depuis qu'il n'y a plus d'écologistes au gouvernement. Le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre a doublé. Et. Une partie de ceux qui par le passé. Étaient les plus activistes et les plus radicaux et qui nous inciter à sortir du nucléaire. À l'époque serait aujourd'hui responsable si les gouvernements successifs les avait écoutés d'une hausse des émissions qui nous aurait considérablement éloignée de là où nous en sommes aujourd'hui, en termes d'empreinte. Alors dans ce domaine il y a à la fois un plan une stratégie double l'atténuation présenté lundi. L'adaptation qui est nécessaire et qui pour le coup n'ait dit un déni, ni un renoncement, mais juste une manière de regarder ensemble le fait que la trajectoire n'est pas la bonne maille. La question du financement. Elle ne peut pas être tabou mais dans la manière dont elle est traitée par Monsieur Pisani-Ferry, elle évoque plusieurs pistes d'abord faire en sorte de réorienter les dépenses. Nous sommes dans les champions du monde en termes de prélèvements obligatoires. L'écologie ne doit pas être le prétexte pour augmenter les impôts il faut réorienter des dépenses et réorienter de la fiscalité mais en aucun cas ne se servir de ce prétexte pour aller ajouter à une forme d'écologie qui écartera une partie de nos concitoyens. Alors qu'on a besoin de tout le monde pour réussir compte tenu de l'ampleur du défi. Madame Préville. Oui, merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. Mais on ne peut pas se satisfaire de la situation, quel que soit ce qui a été engagé. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été engagés mais nous avons des inquiétudes notamment sur les condamnations récurrentes. Pour inaction climatique pour non respect de la qualité de l'air sur des paroles sur la pause environnementale par exemple et sur très concrètement dans les différentes lois des régression environnementale. Je crois qu'effectivement. Je suis d'accord avec vous mais sur sur ce que vous avez dit, sauf sur le fait que c'est une des parties de la solution dont on ne peut pas se passer le, le fait de, d'avoir un petit peu plus de justice sociale et notamment sur l'acceptabilité. La parole est à notre collègue Nadine Bénureau pour le groupe Les Républicains. La commune de Villegongis dans l'Indre, 120 habitants, a dû accueillir 30.000 teufeurs à l'occasion du 30ème Teknival il est compréhensible que les jeunes se retrouvent pour écouter de la musique mais il est inacceptable. Que ce soit en violation du droit de la propriété inacceptable que ce soit en contradiction avec un arrêté préfectoral en l'absence d'organisateurs non identifiables et non d'identifier en l'absence tout simplement d'organisation. C'est donc la collectivité dans son ensemble qui a organisé la sécurité physique et sanitaire des festivaliers de la population. Je veux saluer et remercier les sapeurs pompiers de l'Indre, les associations de la protection civile, les gendarmes les équipes du SAMU, le personnel de santé, les services de l'État, les collectivités pour leur mobilisation 24h sur 24 durant 5 jours. Tout cela a un coût et c'est le contribuable qui paiera, même si et on peut le saluer des confiscations ont eu lieu et 7h. Mais au-delà du financier, il est urgent. Monsieur le Ministre, de réinstaurer un cadre juridique ferme qui permet d'anticiper et de responsabiliser les festivaliers comme cela était le cas avant 2016 l'illégalité entretient la clandestinité et les festivals continueront il existe depuis 30 ans. Alors Monsieur le Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin à l'impuissance de l'État devant ces situations. Merci. Pour vous retenir de la parole est au ministre de la. Ailleurs et des Outre-mer monsieur Gérald Darmanin. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Bénureau merci d'abord des, des propos vous êtes tenu pour les services publics, qu'ils soient départementaux et locaux et bien sûr qui concerne les les gendarmes et singulièrement le préfet je sais qui étaient mobilisés. Je ai eu de très nombreuses fois votre téléphone et ses équipes préfectorale, puisque vous avez parfaitement raison, il y a eu violation du droit de propriété par plus de 30.000 personnes dans votre département. Un rassemblement qui n'était pas. Dès que nous avons eu quelques heures avant l'information qui se rejoindrait sur le site que vous avez évoquées dans cette commune dont je voudrais évidemment salué les élus municipaux et l'engagement qu'ils ont pu avoir malgré. Les difficultés que vous avez dit et les nuisances extrêmement forte. Un arrêté a été pris par monsieur le préfet, mais quand il y a 30.000 personnes et notamment des très jeunes gens

Malheureusement les nuisances inacceptable que l'on a constaté. Nous avons en revanche décidé de contrôler l'intégralité des personnes et vous savez qu'il y a eu plus de 30.000 contrôles, vous l'avez dit vous-mais vous-. Même madame. La sénatrice je voudrais ici dire que 13.363 13.363 véhicules ont été entièrement contrôlée, faisant naître un millier de verbalisation ou d'interpellations pour consommation de stupéfiants et ou consommation d'alcool que de très nombreux. De sortes de drogue ont été saisies. Oui je veux évidemment aussi souligné que le préfet a fait des articles 40 pour que bien sûr et puis s'y avoir poursuite après constitution de qui est responsable de cette situation et qui est l'organisateur de ces fêtes dont on pense Madame la sénatrice, vous et moi qu'il y a beaucoup d'argent derrière tout ça également. C'est sûr que le droit actuel ne nous permet pas dans les circonstances que vous évoquez de pouvoir, poursuivent les organisateurs qui ne se déclare pas il faut que nous travaillons sans doute avec le Sénat, comme nous le faisons sur d'autres sujets, je pense évidemment. Aux personnes qui s'installent illégalement sur les aires d'accueil où les noms hein d'accueil et il y a des propositions de la part du sénat le gouvernement la regardera avec intérêt en lien que le ministre des collectivités locales, Christophe Béchu. Merci monsieur le président, monsieur Ministre vous dites prêts au dialogue pour pouvoir travailler sur cette question, je le redis. En effet, il faut prévoir à l'avance des terrains adaptés à ces rassemblements, car gouverner c'est prévoir et il faut absolument que l'on puisse ne puisse être de nouveau confrontés à une situation comme celle-ci, c'est-à-dire devant le fait accompli. La parole est notre collègue Nadia Sollogoub. Pour le groupe de l'Union centriste. la Cour des comptes a rendu lundi un rapport sur l'avenir de l'élevage bovin qui a causé sur tous les bancs de vives réactions et j'associe à la mienne mes collègues Nathalie Goulet Anne-Catherine Loisier et tous ceux qui sont élus dans des Terres d'élevage bovin, c'est-à-dire beaucoup. Laurent Duplomb vous a interpellé hier sur ce sujet et vous lui avez répondu que vous feriez fermement le choix de la souveraineté nationale en la matière. Mais le rapport en question préconise clairement ceci manger moins de viande, produire moins de viande et être ainsi à l'équilibre et de cette manière, en fait on assume la souveraineté. Alors, pouvez-vous me confirmer, monsieur le Ministre que c'est plus ce que vous voulez pour l'élevage bovin que cette filière d'excellence reste également exportatrice conserve des capacités de production supérieurs à notre auto-suffisance. Je vous remercie.

Qui fait écho à plusieurs questions qui m'ont été posées et qui font écho au rapport de la Cour des comptes. Alors d'abord je voudrais nous inviter collectivement à lire la totalité du rapport de la Cour des comptes et pas se limiter à la page 9 Ehud heureux que seule recommandation qui sont faites, ce serait justice que de regard que Laurent, je vais en dire un mot, le travail qui a été fait par la Cour des comptes 2ème élément. Là où on peut avoir et c'est normal qu'on puisse avoir un débat, y compris avec la Cour des comptes sur l'équilibrage et le le le. Ce qui est proposé par la Cour des comptes, au fond, c'est une simple décroissance une décapitalisation qu'il faudrait forcer pour répondre à des objectifs que par ailleurs nous avons nécessité tenir qui sont des objectifs carbone alors loin de moi l'idée d'abord de dire que l'élevage ne doit pas prendre sa part des efforts qu'il faut faire en terme de décarbonation d'ailleurs ils se sont mis sur ce chemin il y a des travaux de recherche et d'innovation qui qui portent par exemple sur l'alimentation qui permettent de tenir cette trajectoire loin de moi l'idée de dire que la consommation et que les évolutions de consommation ne sont pas à tenir compte depuis 20 ou 30 ans, on sait que structurellement il y a une baisse de la consommation et que parfois on se, on va vers la viande de l'art, viande rouge vers la viande blanche donc tout ça c'est des choses qu'il faut regarder en lucidité. Mais en revanche il y a quelque chose qui est choquant, c'est de proposer comme seule perspective à un éleveur, c'est, ça fait partie des deux recommandations c'est finalement de ne plus être éleveur. Et et ça c'est quelque chose qui me semble-t-il, n'est pas acceptable. D'abord parce qu'humainement, ça n'est pas acceptable et qu'est-ce que deuxièmement sur ces territoires-là en particulier les bovins allaitant. Il y a pas d'autre solution que faire de l'élevage ou rien et 3ème élément et d'ailleurs la Cour des comptes le dit et ça j'invite à le regarder quand même, c'est comment on tient mieux compte des autres services. Que rend l'élevage que celui d'abord de nous alimenter. Qui est quand même un service important et on a besoin je pense de réfléchir à ce que sont les équilibres. De viande et quel et les matières de viande qu'on a besoin de produire en France pour répondre aux besoins de consommation mais deuxièmement quelles sont les aménité comme on dit, qu'apporte l'élevage en particulier l'. Le Le maintien des paysages ouverts la lutte contre les incendies de forêt, le maintien des prairies la préservation de la biodiversité tout ça ça a de la valeur et donc tout ça il faut, il faut en rendre compte. Il faut aussi en rendre compte dans les soutiens financiers qui sont apportées. L'élevage et donc ne caricaturons pas les uns les autres, on a besoin d'avoir une trajectoire carbone au niveau national, mais on a besoin aussi de respecter les éleveurs dans leur travail et dans les différentes différentes utilité et aménité qu'ils apportent à la société française toute entière. Avaient pu aller se mettent dans une prairie il peut mesurer d'un côté le méthane, émis et puis ce qui est capté mais vous qui vous y connaissez, vous savez qu'une vache qui pète au Brésil ou au Canada a exactement le même effet sur la planète que si elle le fait en France Blague à part, Monsieur le Ministre. Mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Dans les, si les politiques publiques maintenant et les experts de la Cour des comptes doivent tenir compte du bilan carbone dans les évaluations des politiques publiques. Alors il va falloir cesser de soutenir le pouvoir d'achat des ménagères qui mettent dans leur coin caddie des bananes ou du café qui ont ce sont des produits qui, un bilan carbone déplorable. La parole est notre collègue Pascal Alizart. Pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mangez des pommes. Un slogan bien connu et sympathique. Il se trouve que l'on peut aussi en en en boire et vous l'avez compris, je souhaiterais vous parler de l'avenir du cidre français. L'activité cidricole génère de nombreux emplois représentent une filière économique importante dans certains territoires ruraux. C'est notamment le cas en Normandie en Normandie mais aussi dans d'autres régions françaises ses cidre français correspondent à des productions de qualité dont certains sous Label fabriqué sur la base de 100 pour de jus de pomme ou de moûts concentrés de pommes fraîches par contre d'autres États européens produit c'est une boisson également appelé cidre à partir d'un pourcentage de jus de pomme bien plus faible, 5, 10 ou 25%. Il s'ajoute ensuite de l'eau et du sucre en quantité, voir même des ex-Oster de goût. Face à ces disparités, la Commission européenne souhaite semble-t-il harmoniser la définition des cidres commercialisé et les professionnels s'inquiètent d'une harmonisation par le bas qui serait préjudiciable à cette filière. Par conséquent, Monsieur le Ministre où en sont réellement les travaux sur ce sujet et comment le gouvernement entend-il préserver le cidre français et nos spécificités au niveau européen. Pour vous répondre. La parole est au ministre de l'Agriculture et de souveraineté alimentaire, monsieur Marc Fesneau. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la question de la filière cidre et nous sommes nombreux, y compris la Première ministre être sensible à la question du cidre. En bon normand que certains d'entre vous sont il y a plusieurs sujets de. Mais le sujet principal que vous posez c'est la question de l'harmonisation du droit. Et de l'étiquetage au fond du cidre. La vérité c'est que la situation aujourd'hui. Il n'y a pas de règles. Et que chacun peut dénommé cidre Sider d'ailleurs dans certains pays des produits qui ne sont pas avec les mêmes degré d'exigence. Le premier degré d'exigence. Vous l'avez dit. Avec une formule, c'est que quand vous buvez du cidre en France il est à 100 pour % le produit. De pommes et il n'est pas mélangées à autre chose La position qui est défendue par la France au niveau européen dans cette caisse ce contexte d'harmonisation. C'est bien une harmonisation qui tire tout le monde vers le haut. Et qui fasse en sorte qu'on essaie de sortir de la situation dans laquelle on est est que nous sommes à frontières ouvertes où des gens peuvent se réclamer de l'appellation. Pas de l'appellation de la dénomination cibles sans en être vraiment et qui permettent de mieux valoriser la qualité du cidre français en particulier de la région que vous connaissez bien et donc c'est là-dessus qu'on essaie de travail avec la commission là le sujet européen c'est toujours le même à la vérité, c'est pas le sujet n'est pas d'avoir raison défendu une position de trouver le sujet c'est de trouver une majorité. Et d'arriver à vaincre les collègues et donc c'est le travail qu'on fait actuellement au niveau européen pour faire en sorte qu'on reconnaisse bien la qualité du site en ce qu'il est le composé à 100% de pommes et que pour le reste, on peut appeler ça comme on veut mais qu'on ne peut pas l'appeler cidre si on est dans le registre d'une harmonisation européenne. Tels sont les éléments que je peux vous dire aujourd'hui, n'est pas acceptable que ce soit quelque chose qui viendrait dégrader. La qualité du cidre français parce que elle est reconnue au travers par les Français et les gros que nous là des frontières et donc on a besoin de le mieux la faire reconnaître et donc l'étiquetage est un élément important. Merci monsieur le ministre, effectivement, la Commission européenne précise que ce rapport je cite ne conduira pas forcément à une proposition législative, or nous savons bien que en fait la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Donc la méfiance et la vigilance doivent être de de mise car on connaît le zèle de certains Nord mateurs. Et on connaît aussi leur capacité à prendre le bon sens à contre-pied vous l'avez compris, Monsieur le Ministre, on compte sur vous.

merci Monsieur le le président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, le 1er mars dernier, à l'initiative de notre groupe, nous organisions dans cet hémicycle un débat sur la mixité sociale à l'école. Le constat implacable étaient partagés sur l'ensemble de nos bancs. Alors qu'en moyenne la proportion d'élèves issus des milieux défavorisés et de 42,6% dans le public allait seulement de 18% dans le privé. Ces écarts ne cesse de se creuser depuis 20 ans. Nous allons vers un système scolaire à 2 vitesses, une école privée réservée aux enfants privilégiés et une école publique pour tous les autres, voilà le véritable séparatisme à l'oeuvre dans notre pays à l'occasion de ce débat du 1er mars. Le ministre de l'Éducation nationale. Disait, je cite parce que l'argent public finance l'enseignement privé sous contrat à hauteur de 73%, je le rappelle, il est normal d'exiger de ce dernier qu'il favorise aussi la mixité des élèves. Il parlait alors de moyens de pression sur les établissements privés sous contrat, notamment en modulant leurs subventions sous forme de bonus malus, mais aussi en jouant sur les allocations de poste, il avait même aborder la question de la sectorisation dont vous estimiez qu'elle avait donné des résultats probants. Nous attendions donc avec impatience des annonces fortes de la part du gouvernement pour mettre fin à cette ségrégation scolaire qui mine notre pacte social et fait de notre pays, un des plus inégalitaire de l'OCDE. Le protocole d'accord que vous avez dévoilé le 17 mai après 2 reports a fait pschitt. Il ne comporte ni exigences contraignantes ni modulation des subventions des allocations de poste ni bonus malus et encore moins de sectorisation nous comprenons donc que ce gouvernement qui défend toujours les plus privilégiés n'agira pas pour plus de mixité scolaire. Quand prendrez-vous la mesure du problème en agissant fortement pour des mesures contraignantes pour mettre la mixité scolaire dans les écoles de France. Pour vous répondre. La parole est à la ministre déléguée chargée de l'enseignement. Et la formation. Je dirais, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Yan Chantrel. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye qui retenu sur le prix, non au harcèlement. Vous le savez, notre ambition est d'avoir une action résolument concrètes de réduction. De la ségrégation sociale de nos établissements scolaires. Nous ne pouvons nous satisfaire en effet de la situation actuelle. L'écart de composition sociale entre élèves des établissements du public mais aussi entre établissements du public et du privé se creuse depuis les années 2000 et vous l'avez rappelé. Pour y remédier, le ministre de l'éducation nationale a d'abord voulu agir sur les établissements publics qui je le rappelle. Rassemble 90% des élèves. C'est pourquoi il a demandé à l'ensemble directeur de s'emparer de différents leviers avec pour objectif de faire progresser de 20%. La mixité sociale dans les établissements publics d'ici à 2027. En ce qui concerne l'enseignement privé. Le ministre a toujours souhaité privilégier la concertation à la contrainte sur ce sujet. D'autant que la préoccupation de la mixité, ce que ce que le social et scolaire et plus que partagés par l'enseignement catholique et qu'ils ont très vite montré leur volonté de s'engager sur ce sujet et c'est bien grâce à cette concertation. Fruit d'un travail de plusieurs mois que nous avons pu signer mercredi dernier un ah protocole d'engagement commun avec le secrétaire général de l'enseignement catholique. Ça n'avait pas été fait depuis plus de 30 ans et je crois qu'il faut le souligner. Ce protocole, il prévoit notamment de suivre avec des indicateurs précis précis les effets de ces actions à travers l'évolution de la mixité sociale et scolaire au sein des établissements privés sous contrat. Je crois que c'est une avancée importante qu'il faut pouvoir souligné. Vous le voyez, pour que cette politique en faveur de l'égalité des chances pour que tous les élèves réussissent. Nous pensons qu'il faut convaincre et non contraindre. Merci la parole est à d'autres collègues Pierre Charon pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, c'est toujours désagréable de s'adresser à un absent en 2022 pour faire face à la hausse continue des atteintes à la laïcité. Vous avez élaboré un plan. Depuis la publication de ce plan, que constate-t-on. Au mois d'octobre dernier, le nom de signalements avait atteint 720. Une hausse de 130% par rapport au mois précédent au mois de mars, il avait encore été dépassé les 500 cas. Monsieur le Ministre, comme vous l'avez déclaré la hausse du mois d'octobre est liée à la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty, mais 500 cas du mois de mars correspond à une remontée chaque année au moment du ramadan dites-vous vos explications très catégorique n'd'ailleurs réussi qu'une seule chose soulevé une polémique et notamment par la Grande mosquée de Paris. Quant au mois d'avril. Dans l'académie de Paris. Les données qui ont été communiqués par vos services ne sont pas bonnes. Je vous laisse le soin de les annoncer, ce sont des chiffres les plus élevés depuis la rentrée de septembre. Il faut aussi ajouter les signalements d'actes d'antisémitisme qui eux ne relève pas d'atteinte à la laïcité mais les procédures pénales. Vos statistiques sont-ils fiables et surtout, sont-elles utiles. La réponse est non. Vos chiffres sont manifestement sous-estimé. Pour le principal syndicat des personnels de direction des collèges et lycées les tenues litigieuse et contestation d'enseignement ou même les difficultés en sortie scolaire ne font pas l'objet de signalements de manière systématique. Vos statistiques sont-elles utiles. La réponse est encore non. Ces chiffres ne traduisent en aucune réponse aux attaques contre la laïcité, les chefs d'établissement se sentent bien seuls, ils attendent des réponses concrètes, ils vous demandent des outils réglementaires pour mieux gérer ces situations. Votre absence de fermeté sur tous les sujets maintient la porte ouverte à toutes les revendications communautaires. Ma question est simple, allez-vous. Monsieur le Ministre vous contenter, mois après mois de recenser les atteintes à la laïcité et de les commenter, vous allez vous enfin donner aux responsables d'établissements des directives claires merci. On vous répond de là. Par l'État, la ministre déléguée chargée de l'enseignement. Madame Grandjean. Afin de de répondre à votre question, je souhaite rappeler plusieurs actions engagées par Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui je le rappelle, est absent pour. Cause de remise de prix sur le l'enjeu de à la lutte contre le harcèlement. Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse a demandé une publication des chiffres mensuels des atteintes à la laïcité que vous avez rappelé ces chiffres sont désormais. Visibles disponible sur le site du ministère de l'Éducation nationale pour plus de transparence, plus de suivi et organisé cette mobilisation pour la lutte contre les atteintes à la laïcité, le ministre de l'Éducation nationale a souhaité la les c'est nécessaire renforcer. Des équipes valeurs de la République et a élargi la formation de tous les personnels de l'Éducation nationale, je voudrais le rappeler, le plan que le ministre a annoncé en novembre 2022, a déjà permis à 300.000 personnels d'éducation, dont 5000 chefs d'établissement et adjoint Je crois que cette formation est absolument concrète, elle permet aux uns et aux autres d'être mieux accompagnés, mieux avec des outils qui leur permettent de lutter efficacement contre ces atteintes à la laïcité, le ministre de l'Éducation nationale a également renforcé les mesures du CF disciplinaires en cas d'atteinte au principe de laïcité en diffusant une circulaire très clair. Au chef d'établissement qui jusqu'à présent resté dans le flou quant aux procédures à mettre en oeuvre. Le ministre de l'Éducation nationale a également institutionnalisé le conseil des sages et de la laïcité en nommant enfin ses membres. 5 ans après la création de cette entité. Les membres historiques ont d'ailleurs tous été confirmé dans ses fonctions. Je voudrais, Monsieur le Sénateur, que nous puissions partager la l'engagement du gouvernement et du ministre de l'Éducation nationale sans faille pour lutter contre ces atteintes à la laïcité. Je crois que, au-delà des mots, les actions sont les plus fortes, l'accompagnement des personnels, l'engagement bien sûr de cela mais aussi l'organisation des mesures disciplinaires, qui sont donc passés par voie réglementaire, récemment encore, merci. Monsieur le président. Monsieur le 1er Ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mes chers collègues. Dimanche matin au commissariat de Roubaix, une équipe de policiers assurent la relève de nuit. Appel de détresse d'une jeune fille. Cette mission est confiée à une jeune patrouille de policiers recueillir 7 mineurs présumés violée pour la protéger et la conduire à l'hôpital. Cette précipitation au service de l'autre sera la dernière. Pour Paul Steven et Manon. Ce matin-là, ils sont partis de chez eux heureux. Il ne savait pas qu'il ne reverrait jamais leurs proches à Roubaix il y a une vraie solidarité entre la police nationale municipale les pompiers. C'est une ville méritante. À l'École nationale de police de Roubaix, la directrice, la commissaire qui Ishchenko. Apprend aux nouvelles recrues. Les difficultés de la profession. Il faudra beaucoup de professionnalisme et de rigueur pour exercer ce métier. Manon stagiaire était prête à entrer dans cette grande famille. Kader Haroun. Le commissaire principal de Roubaix dirige le commissariat avec bienveillance et fermeté. Il leur a dit combien la police c'était un vrai ascenseur social pour tous ceux qui ont à coeur de défendre les valeurs de la République, Monsieur le Ministre, vous êtes fier de vos hommes, vous avez bien raison de les défendre. La mort de ces trois jeunes policiers de Roubaix prouve encore une fois les risques de ce métier. Ils ont été tués par un chauffard ivre, sous l'emprise de stupéfiants roulant à grande vitesse à contresens récidiviste et connu des services de police. Leur décès est un choc immense pour tous leurs collègues, leurs proches. Le nord et plus largement pour notre pays tout entier. Ce qui s'est produit est inacceptable au nom de tous mes collègues, j'adresse mes sincères condoléances aux familles et aux proches des jeunes. Aujourd'hui on se recueille, Monsieur le Ministre, que pouvons-nous faire dès demain pour stopper ce fléau. Je me dois de vous demander, Monsieur le Ministre, si le gouvernement entend prendre des mesures pour intensifier la lutte contre les conducteurs dangereux sous emprise de drogue ou d'alcool et s'il envisage de durcir les peines encourues par l'ordinateur. Ou autre. Pour vous répondre. La parole est au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer monsieur Darmanin. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Brigitte Lherbier merci. Des mots très touchants, que vous avez eu pour ces trois jeunes policiers du commissariat de Roubaix. Parmi les plus difficiles de France qui compte énormément de moyens à la hauteur sans doute. Du dur métier que font les policiers et les parce illustratif. De de de ce site qui vous le savez, vous avez cité le commissaire Haroun fait l'honneur de la police nationale. Moi je veux d'abord dire aux familles de ces policiers demain le président de la République le rendra officiellement hommage à l'École nationale de police de Roubaix. Qu'ils font l'honneur à 24 à 25 à 26 ans de la France du service public et nous pensons tous à leur famille. À ce petit enfant d'un an qu'il aurait eu un an dans les jours qui viennent et à cette jeune femme qui est enceinte d'un de ces jeunes policiers et cet assassin. Celui qui était dans la voiture. Verse parce qu'il faut utiliser les mots qui compte a tué non seulement 3 destins mais baissé l'intégralité de la police nationale. Alors après l'hommage il y a évidemment réfléchir madame. La sénatrice et avec d'autres faits divers parce que ce n'est pas le seul. Trop de chauffard trop d'assassins tuent sur les routes sous l'emprise de stupéfiants. Delecole. Nous travaillons avec le garde des Sceaux. Pour. Évidemment, pouvoir réussir à limiter hein ces drames. Nous avons proposé le retrait des 12 points pour ce qui concerne ce stupéfiant, c'est une mesure réglementaire, le garde des Sceaux a proposé de renommer. Cet homicide comme un homicide routier c'est attendu, il y a beaucoup de propositions d'ailleurs de votre assemblée, elle est sur tous les bancs. Je peux vous assurer que sous l'autorité de la Premier Ministre avec monsieur le garde des Sceaux et en espérant que d'autres drames sont invités par le travail que font les policiers, les gendarmes tous les jours sur les routes pour éviter que ses chauffeurs de continue à tuer. Nous sommes à disposition du Parlement et du Sénat et de vous même, pour pouvoir travailler en ce sens en la mémoire de ces trois jeunes policiers je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. Nous avons terminé avec les questions au gouvernement. Je vous rappelle que les prochaines questions lieu le mercredi 31 mai à 15h. Je vais suspendre la séance elle sera reprise à 16h 30 pour l'examen de 4 conventions internationales puis du projet de loi visant à donner à la douane, les moyens de faire face aux nouvelles menaces. La séance est suspendue.

La parole est donnée à Monsieur Michel Canevet pour une mise au point, au sujet d'un vote. Pour l'école. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, je souhaite opérer une rectification de vote Merci de cette rectification. Merci, cher collègue, acte et donner de votre mise au point, elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concernés. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue. Albert Vecten qui fut sénateur de la Marne de 1983 à 2001. En application du 5ème alinéa de l'article 13 de la Constitution ainsi que de la loi organique et de la loi ordinaire prises pour son application. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis lors de sa réunion de ce jour un avis favorable. 34 voix pour aucune voix contre à la nomination de Monsieur Olivier Thibault aux fonctions de directeur général de l'Office français de la. Biodiversité. En application de l'article 16 bis alinéa 2 du règlement, monsieur le président des. Sénat. Propose la constitution d'une commission spéciale en vue de l'examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Nous pourrions inscrire à l'ordre du jour du 1er juin à 10h 30 l'examen de cette proposition du président du Sénat puis le cas échéant la nomination des membres de cette commission spéciale des candidatures devront être transmises avant le mercredi 31 mai à 15h. Il n'y a pas d'opposition. Il en est ainsi décidé j'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants ont été publiés ces candidatures seront ratifiées c'est la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle l'examen de 4 projets de loi tendant t'a autorisé la ratification ou l'approbation de conventions internationales pour ces 4 projets de loi. La conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifiée. Je vais donc les maîtres successivement aux voix. Je mets aux voix. Le texte adopté par la commission sur le projet. Sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle aux personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État. Dans l'autre signé à Paris le 7 septembre 2021 et de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka relatif à l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle salariée par les membres de la famille des agents des missions officielles de chaque État. Dans l'autre signé à Paris le 23 février 2022. La commission des Affaires étrangères est favorable. À l'adoption de ce texte qui est. Pour. Qui est contre qui s'abstient. Le projet de loi est adopté. Je mets aux voix. Le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole du 30 avril 2010 à la convention internationale 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuse. La commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption de ce texte qui est pour. Qu'ils contrent qui s'abstient. Le projet de loi est adopté. Je mets aux voix. Le texte adopté par la commission sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale. Après engagement de la procédure accélérée autorisant la promesse. De la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal et de la convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal. La commission des Affaires étrangères et favor favorable à l'adoption. Ce texte qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Le projet de loi est adopté définitivement, je mets aux voix le texte. Adopté par la commission sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la principauté d'Andorre concernant l'amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales. Liés aux risques naturels entre Prades et la frontière franco-andorrane. La commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption de ce texte. Qui est pour. est contre qui s'abstient. Le projet de loi est adopté définitivement. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi visant à donner à la douane, les moyens de faire face aux nouvelles menaces. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte et dans la discussion générale. La parole est à monsieur Gabriel Attal Ministre délégué chargé des Comptes publics. Monsieur le Ministre.

Madame la présidente. Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur de la commission des finances. Monsieur le rapporteur pour avis de la commission des lois, mesdames et messieurs les sénateurs. Au moment de vous présenter le 1er projet de loi dédié aux douanes depuis plus de 60 ans. Permettez-moi de partager avec vous la très grande fierté qui est la mienne d'être comme ministre en charge des comptes publics, le ministre en charge des douanes. Une administration dont l'histoire se confond avec celle de la construction puis de l'affermissement de l'État comme avec celle de la construction puis de l'affermissement de l'Union européenne. Une administration qui assure depuis des siècles. Hé bien avant d'ailleurs l'avènement de la République. Des missions régaliennes par excellence, celle d'assurer l'intégrité de notre territoire de consolider la puissance économique et commerciale de la France et de maîtriser les frontières. Le douaniers ont vécu et accompagner les grandes transformations de notre histoire récente. Ils ont accompagné l'accélération de la mondialisation, l'internationalisation des échanges et la diversification du commerce extérieur. Ils ont été la figure de proue de la construction européenne avec la construction de l'union douanière en 1968 et en 93, la disparition des frontières intérieures de l'Union européenne. Ils en ont accompagné tous les soubresauts très récemment encore avec le Brexit et le rétablissement de la frontière de la Manche et ils étaient encore au 1er rang il y a quelques mois pour mettre en oeuvre les sanctions à l'encontre de la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Oui, nous sommes fiers de cette administration ancré au ministère des finances qui dans la paix, comme dans la guerre n'a jamais manqué à ses devoirs envers la nation tout en démontrant une exceptionnelle capacité d'adaptation, une formidable capacité à affronter des enjeux nouveaux avec pour seule boussole. L'intérêt du pays. Oui, nos douaniers ont su constamment s'adapter au bouleversement du monde. Mais le cadre juridique dans lequel ils agissent n'a pas fait preuve de la même plasticité. doutes dédié à la douane a été votée depuis 60 ans. Voilà bien un sujet sur lequel les gouvernements successifs n'ont pas été pris de frénésie normative. Cela n'a pas empêché nos douaniers d'agir efficacement. Mais vous en conviendrez. Il est grand temps de moderniser le cadre de leur action. Et c'est pourquoi le gouvernement propose dans ce texte à la fois des évolutions immédiatement utile et le lancement d'une recodification à droit constant du code des douanes. La mission qui est la nôtre aujourd'hui et c'est l'objet de ce projet de loi, c'est tout simplement de permettre à nos douaniers d'agir le plus efficacement possible. Continuer à agir pour continuer à assurer notre protection, pas seulement celle de nos frontières, mais aussi celle de nos compatriotes et de nos entreprises car c'est bien de ça dont il est question aujourd'hui. Protéger les Français. Protéger notre économie protéger notre souveraineté. Oui, c'est bien cette mission essentielle qu'hier comme aujourd'hui, les agents de la douane assurent jour après jour, ces femmes et ces hommes agissent dans un environnement où les menaces se multiplier et se métamorphose, notamment sous l'effet de la révolution numérique. Ces femmes et ces hommes livrent jour après jour, avec sang-froid. Courage et détermination des combats que nous n'avons tout simplement pas le droit de perdre. Non, nous n'avons pas le droit de perdre la guerre qu'il faut mener contre la drogue. Un fléau qui détruit tant de vies. J'étais il y a quelques mois en déplacement aux États-Unis où j'ai rencontré Léo, responsable de la douane américaine. Ils m'ont parlé des ravages. C'est par les nouvelles drogues en 2021 70.000 américains sont morts d'une overdose de fentanyl cet opioïde de 7 opioïdes de synthèse qui se diffuse à grande vitesse aux États-Unis. Nous ne voulons pas de ça en France et c'est ici et maintenant que ce combat se joue. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Pas le droit d'échouer contre la fraude et les trafics. Pas le droit d'échouer contre la contrebande qui n'est pas seulement une fraude mais un danger insidieux pour la santé publique pour le consommateur français. Pas le droit de perdre la bataille que nous livrons contre la criminalité organisée contre ces organisations tentaculaires qui mobilise des moyens parfois considérables pour déstabiliser notre toute société et qui sont prêtes à tout par seul appât du gain. Mesdames, et messieurs les sénateurs, les agents que j'ai l'honneur de diriger appartiennent à l'administration de la marchandise et de la frontière, celle qui facilite les échanges économiques et gardent nos frontières. Ils appartiennent à une administration qui luttent sans relâche pour protéger nos compatriotes de danger dont ils ne mesurent pas toujours l'ampleur. Ils consacrent leur vie et là risquent parfois pour tenir nos frontières terrestres, maritimes, aériennes et nous y reviendrons frontière numérique aussi car l'espace virtuel est encore trop souvent une zone de non-droit qui charrie des menaces aux effets bien réels. Ils obtiennent des résultats exceptionnels à nos frontières, comme à l'intérieur du territoire national. Près de 105 tonnes de stupéfiants saisis. L'année dernière nos douaniers saisissent 70% des stupéfiants qui sont saisis dans notre pays. 11 5 millions d'articles contrefaits retirés du marché grâce à nos douaniers près de 650 tonnes de tabac de contrebande ou de contrefaçon saisis grâce à nos douaniers pour eux pour nous tous, nous devons être à la hauteur. Être à la hauteur. C'est d'abord donner à la douane, les moyens d'exercer ses missions. C'est l'objet du contrat d'objectifs et de moyens dont nous avons doté la douane. Sur la période 2022 2025. Ce contrat prévoit que la douane bénéficiera de plus de 148 millions d'euros supplémentaires et d'une garantie de stabilité de ses effectifs. Nos priorités d'investissement sont claires, le E-commerce la professionnalisation du métier de gardes frontières et la lutte contre la criminalité organisée. Six mois après mon arrivée, j'ai souhaité affirmer une autre priorité face à la croissance fulgurante des trafics. La contrebande et la contrefaçon des tabacs. Je le dis, c'est un fléau pour la santé publique. C'est un fléau pour la sécurité publique car ces trafics de tabac alimentent des réseaux criminels et mafieux responsable de traite humaine responsable de trafic de stupéfiants responsables parfois de terrorisme ou de radicalisation. C'est un fléau aussi pour nos territoires car ces trafics déstabilise le réseau des buralistes dont nous avons besoin ces commerces d'utilité locale qui sont aujourd'hui. Qui assume aujourd'hui des missions quasiment de service public en permettant le paiement d'amendes de facture du quotidien en assumant des fonctions de relire, de relais pour les colis postaux en étant des interlocuteurs du quotidien et des promoteurs du lien social sur nos territoires. Nous devons aussi. À notre réseau des buralistes une lutte intraitable contre les trafics de tabac dans notre pays et nos douaniers sont au 1er rang de ce combat. Pour ce combat, nous devons changer d'état d'échelle de méthode et de moyens. J'ai annoncé dans le cadre du plan ta que j'ai présenté à la fin de l'année dernière la densification du réseau des Lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation les Lapie qui reviendront dans nos débats ce soir ou la généralisation du déploiement de scanners qui seront des adjuvants essentiel dans la lutte contre la drogue et contre les trafics de tabac 14 nouveaux scanners seront déployés d'ici 2025 et j'ai fixé un objectif qu'en 2025, nous soyons en mesure de scanner 100 pour des colis postaux qui arrivent sur notre sol dans les centres de tri postal, c'est absolument essentiel puisqu'on le sait aujourd'hui, une partie importante du trafic et réalisé via l'envoi de colis, parfois en petite qu'en au sein du colis mais en quantité massive de colis d'ici 2027. Je souhaite que nous investissions 45 millions d'euros supplémentaires dans ces équipements. Être à la hauteur du courage et de l'engagement de nos douaniers c'est aussi sécuriser leur action sur le plan juridique, je pense bien sûr au droit de visite, c'est aussi leur donner de nouveaux moyens de nouveaux outils de nouvelles capacités pour toujours mieux protéger les Français. Oui, nous devons donner à nos douaniers les moyens d'exercer leur mission. C'est la condition pour qu'il continue à obtenir des résultats et nous devons le faire en veillant à respecter scrupuleusement les droits et les libertés individuelles. Je veux saluer les travaux qui ont entouré l'examen de ce projet de loi, et notamment les deux rapporteurs Albéric de Montgolfier Alain Richard qui ont réalisé avec leurs commissions respectives. Un travail absolument remarquable avec une seule boussole encadré sans entraver. Nous devons avoir cette boussole à l'esprit le partage des 16 articles du projet de loi entre ces 2 commissions a permis qu'un travail approfondi soit engagée par chacune d'entre elles et je veux remercier l'ensemble des sénatrices et sénateurs qui ont voulu enrichir ce texte au stade de la Commission comme au stade de la séance publique nous en débattrons évidemment. Dans les heures qui viennent mais je veux d'abord souligner 2 points le 1er c'est que nous partageons l'essentiel. C'est-à-dire les objectifs finaux poursuivi par ce texte. Et je crois donc que ce texte peut rassembler très largement, par delà les clivages partisans. Le 2ème, c'est que nous devons toujours avoir à l'esprit que les spécificités du droit douanier s'explique par la réalité opérationnelle de leur travail et par le cadre juridique européen dans lequel il s'exerce et qu'elles sont sans doute l'un des agressions de l'efficacité incontesté de la douane française. Cette ligne de crête invite à la prudence. Le gouvernement comme chacun d'entre vous a à coeur de garantir les droits de la manière la plus complète possible, telle est l'objectif du dispositif du droit de visite douanières proposées par ce texte. Mais pour ma part, je veux que notre première priorité soit d'éviter que des bouleversements introduits dans le code des douanes complique la tâche de nos douaniers et de fait, facilite la vie des trafics. Je l'ai dit le premier enjeu de ce texte pour ainsi dire son fait générateur, c'est d'offrir à nos douaniers la sécurité juridique indispensable à l'exercice du droit de visite. Dont je rappelle qu'il a été dans sa rédaction actuelle déclaré non conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel. Il faut mesurer le choc qui a été la décision du Conseil constitutionnel pour l'ensemble des douaniers. L'insécurité qui a pu régner aussi depuis cette décision avec parfois certaines annulations de procédure qui n'était pas motivée par l'annulation par la décision du Conseil constitutionnel. Mais avec une forme de flou qui s'est installé un flou qu'il nous faut écarter aussi rapidement. Que possible. C'est l'objet de ce texte pour répondre aux critiques formulées par le Conseil constitutionnel ce texte réécrit intégralement l'article 60 du code des douanes pour sécuriser le droit de visite. Droit de visite qui vous le savez constituent une prérogative essentielle pour les douaniers puisqu'il s'agit tout simplement de pouvoir contrôler les marchandises, les moyens de transport et les personnes afin de rechercher les fraudes. Les articles 1 à 5 du projet de loi assure la mise en conformité du droit de visite par 3 grands moyens. D'abord le texte que vous nous nous vous proposons inscrit dans la loi, les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation au fil des années, sont ainsi codifié. Le prix un caractère contradictoire des contrôles. L'interdiction de la fouille à corps et le maintien à disposition des personnes sur le temps strictement nécessaire aux opérations de visite. Ensuite. Ce texte maintient dans la zone frontière une prérogative de contrôle étendus justifiées par la nature même des infractions douanières dans le rayon des douanes fixée à 40 kilomètres de nos frontières, ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires et routières international le droit de visite pourra continuer à s'exercer sans modification par rapport à l'état actuel du droit. Enfin le texte encadre l'exercice du droit de visite à l'intérieur du territoire. L'exercice de cette prérogative devra désormais s'inscrire dans deux cas bien précis. Soit sur le fondement de raisons plausibles de soupçonner que la personne contrôlée a commis une infraction douanière. Soit après information préalable du procureur de la République pour la recherche d'infractions douanières. Il s'agit, j'insiste sur ce point d'une information et non d'une autorisation du procureur, afin de ne pas entraver ou ralentir l'action de nos services. Cette distinction entre le rayon des douanes et l'intérieur du territoire. C'est le coeur de la mise en conformité et du point et c'est le point essentiel à la mise en oeuvre de la décision du Conseil constitutionnel. Nous avons beaucoup travaillé pour cette rédaction. Nous avons évidemment. Des juristes. Nous avons associé les organisations syndicales de douaniers, nous avons testé chacune des rédactions et une des des des évolutions auprès de douaniers du terrain pour bien vérifié que c'était compatible avec l'Europe. Activités du quotidien et ce texte a pu être validé par le Conseil d'État dans sa rédaction. Nous sommes profondément convaincus que l'équilibre retrouvé et le meilleur pour la douane comme pour la protection des libertés, comme vous, je veux que le droit protège donc le droit entravent de manière excessive et je pense que nous pouvons nous retrouver sur ce point mais vous l'avez compris, ce projet de loi ne consiste pas seulement à assurer la mise en conformité d'une prérogative essentielle. Il s'agit aussi d'adapter nos moyens d'action de mettre nos douaniers en situation de lutter le plus efficacement possible contre les grandes menaces d'aujourd'hui et de demain. D'abord, nous voulons donner à nos douaniers les moyens de lutter contre la cyberdélinquance et la cyber criminalité. L'article 9, leur permet de prendre connaissance et de saisir au cours d'une recrue d'une retenue douanière des objets, des documents qui se rapportent à un flagrant délit douanier, y compris lorsque ce support et numérique. De quoi parle-t-on concrètement de données contenues dans un ordinateur un disque dur un smartphone que nos agents pourront saisir et dont ils pourront faire une copie sur autorisation du procureur de la République ce dispositif accélérera considérablement les enquêtes douanières et leur efficacité. Ensuite, nous proposons de permettre à nos agents de procéder au gel des données stockées sur des serveurs informatiques lorsque ceux-ci se trouvent à l'extérieur du lieu perquisitionnés concrètement l'objectif c'est que les données qui sont conservés dans des Claude comme on dit aujourd'hui, comme c'est souvent le cas ne soit pas effacé par les suspects et qu'elle puisse être effectivement saisi. Vous le savez, un nombre croissant d'infractions douanières sont commises à partir de contenus en ligne. De quoi parle-t-on par exemple de vente en ligne de produits de contrefaçon ou de tabac de contrebande. C'est la raison pour laquelle l'article 12 de ce texte donne la possibilité à nos agents d'exiger des plateformes qu'elle procède au retrait de ces contenus et si ces plateformes venait à ne pas répondre dans les temps nos agents pourront demander au moteur de recherche de procéder au déréférencement du contenu ou à la suspension du nom de domaine. Là aussi je voudrais m'arrêter quelques instants la conception de ce dispositif a été rendue complexe par l'impossibilité au regard du droit européen de présumer une responsabilité générale des plateformes au titre des marchandises dont elle facilite la vente. Pour autant, nous avons trouvé une voie de passage qui permettra à la douane d'établir un dialogue permanent avec les grandes plateformes allant jusqu'à la sanction pour les plateformes qui entretiennent l'opacité du E-commerce. du E-commerce. Ensuite ce texte propose de mieux utiliser les nouvelles technologies en matière d'enquête et de renseignement douanier. À ce titre, l'article 11 prévoit l'expérimentation d'une durée de conservation étendu à 4 mois des données issues des Lecteurs automatique de plaques d'immatriculation et la Ce que nous voulons pour lutter efficacement contre les trafics de stupéfiants, c'est être en mesure de détecter les convois routiers organisés par les trafiquants. Pour cela, nous proposons d'expérimenter l'utilisation des données des Lapid profondément différentes du dispositif actuellement en vigueur. Je prends un court instant pour expliquer aujourd'hui le fonctionnement actuel des Lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation sert essentiellement rapprocher les plaques d'immatriculation détecté des fichiers déjà constitué pour détecter par exemple des mouvements de personnes déjà connus ou de véhicules. Volés le dispositif que nous proposerons permettra de procéder à des recherches pour identifier des véhicules circulant ensemble en convoi. Et détecter ainsi les mouvements de trafic on on le sait quand il y a du trafic par voie terrestre. Il y a bien souvent une voiture ouvreuse et ensuite une voiture qui la suit. Grâce à l'expérimentation de ce dispositif, nous serons en mesure d'identifier automatiquement des véhicules qui circulent très régulièrement ensemble parfois à des dates régulières, ce qui peut laisser penser qu'il s'agit de convois qui procède à du trafic. De stupéfiants ou de tabac. Je veux insister sur la nécessité dans le cadre protecteur qui est celui de l'expérimentation et du contrôle du Parlement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de disposer de cet outil pour arrêter le trafic à nos frontières. En son article 6, le projet de loi propose de sécuriser le recours par la douane aux techniques de sonorisation et de captation d'images en reproduisant le dispositif prévu par le code de procédure pénale pour les enquêtes douanières cet d'ici une une disposition essentielle et protectrice, qui permettra de mieux séparer les utilisation préventive et les utilisations répressive de ces techniques spéciales d'enquête. Je veux également souligner que le gouvernement a déposé un amendement qui vous sera soumis pour actualiser le régime d'utilisation des drone par la douane. Ce régime est aujourd'hui un complet il ne comprend pas la lutte contre les trafics de tabac manufacturé et il ne couvre pas la surveillance des frontières, alors même que cela est possible pour les services de police et de gendarmerie. Je le dis très clairement les réseaux criminels n'hésite pas à utiliser des technologies dernier cri pour commettre leurs méfaits. Si nous ne combattons pas à armes égales. Je ne vois pas comment nous pourrions remporter la bataille. Agir dans l'espace numérique faire coopérer des plateformes et les moteurs de recherche. Voilà ce que nous voulons exploiter pleinement les nouvelles technologies pour être aussi efficace que ce que nous affrontons. Voilà ce que nous devons faire. Oui les organisations que nous affrontons ne manque pas de moyens. C'est la raison pour laquelle nous devons les frapper au portefeuille. C'est sans doute un des moyens efficaces pour agir et les affaiblir. L'article 6 crée un dispositif de retenue temporaire d'argent liquide circulant à l'intérieur du territoire lorsqu'il lorsqu'il existe des indices que cet argent est lié aux activités criminelles les plus graves. Ce délit, je le rappelle existait uniquement pour les flux d'argent liquide en provenance ou à destination de l'étranger et il fallait impérativement corriger cela. C'est d'ailleurs une évolution qui va dans le sens des préconisations du rapporteur Albéric de Montgolfier dans un rapport d'information réalisée avec le sénateur Claude nous Jean elle permettra notamment à la douane de mieux lutter contre le phénomène des mules entre le territoire métropolitain et la Guyane. Nous voulons aussi réformer le délit de blanchiment douaniers. Il s'agit notamment d'inclure les cryptoactifs dans les types de fonds pouvant relever du délit de blanchiment, douaniers, enfin vous le savez, je le disais il y a un instant je veux mener un combat sans merci contre le trafic de tabac. J'avais à la fin de l'année dernière, fait un certain nombre d'annonces en ce sens dans le cadre du plan tabac que j'ai présenté à cet égard, le texte prévoit un renforcement des sanctions applicables au trafic de tabac. Nous voulons par exemple créer une peine complémentaire d'interdiction du territoire pour les étrangers qui ont fait l'objet d'une condamnation pour contrebande de tabac, comme c'est le cas lorsqu'il y a du trafic de stupéfiants. Par ailleurs nous durcissant les sanctions pénales applicables à la fabrication et à la détention de tabac de contrebande. Celles-ci sont portées de un à 3 ans d'emprisonnement si ces délits sont commis et lorsqu'ils sont en bande organisée. La peine d'emprisonnement pas souvent Je le dis, nous voyons très concrètement que des réseaux mafieux des réseaux criminels jusqu'alors dédiée au trafic de stupéfiants se sont reportés massivement sur le trafic de tabac. Estimant probablement que les sanctions sont moins importantes. Nous devons donc sanctionné le trafic de tabac de la même manière que nous le sanctionnons le trafic de stupéfiants. C'est l'objet de cet alourdissement des sanctions, la menace a changé d'échelle. Nous ne sommes plus dans le transport de quelques cartouches de cigarettes caché dans son sac en traversant la frontière nous avons démantelé sur le sol national l'an dernier 5 usines de fabrication clandestine de tabac. On parle de hangars sur le sol national. Au sein desquels étaient produits entre un et 2 millions de cigarettes de contrefaçon par jour pour alimenter le circuit parallèle sur le territoire national. Le trafic a changé d'échelle. Notre réponse doit elle aussi changer d'échelle. C'est l'un des objets de ce texte. Vous le voyez, mesdames et messieurs les sénateurs. Ce texte est bien plus qu'un projet de mise en conformité. C'est un texte de mobilisation générale contre tous les trafics et un texte de soutien total à nos douaniers qui agissent chaque jour pour nous protéger, pour protéger nos frontières, protéger les Français et vous me permettrez. De saluer les douaniers qui sont dans les tribunes de cet hémicycle qui viennent de la direction interrégionale des douanes d'Île-de-France de la direction générale des douanes ou de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et à travers eux remercier et saluer l'ensemble des agents douaniers. Sur le territoire national. Je sais que nous aurons d'ici quelques minutes des débats importants sur les garanties apportées en matière de droits fondamentaux. J'espère que nous serons ensemble, trouver les bons points d'équilibre sur les différents dispositifs afin de permettre à nos douaniers d'agir efficacement sans renoncer aux exigences qui doivent être les nôtres les douanières et les douaniers comptent sur nous. Ils attendent de la clarté de la précision et des moyens d'action. Je sais qu'ensemble nous serons capables de leur apporter leur permettant ainsi d'assurer la protection de nos frontières et surtout de nos compatriotes. Nous le leur devons je vous remercie. Merci monsieur le ministre. La parole est à monsieur Albéric de Montgolfier, rapporteur de la commission des finances. Dans la présidente. Monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur de la commission des lois, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez employé des mots à l'instant encadré sans entraver. C'est la volonté qui est affichée par le gouvernement, c'est également celle qui a guidé la commission des finances de l'eau. Nos travaux puisque le texte que nous examinons cet après-midi sur les douanes et il faut le dire, le fruit d'un travail de compromis. le travail sans doute nécessaire pour mieux encadrer certaines pratiques des agents des douanes qui apparaissent, vous l'avez dit, je le partage un peu datées, mais également. Tâté au regard de la jurisprudence mais également agir pour la protection des libertés individuelles. Et il comprend également des dispositions qui vise à étendre les prérogatives de la douane et notamment à les étendre à de nouvelles formes de criminalité de fraude. Je peux penser notamment à tout ce qui concerne la fraude sur Internet qui sur un code des douanes un peu anciens n'était pas forcément envisagé alors je vais peut-être parce contre Monsieur le Ministre corriger tout de suite ah de vos propos. Vous avez dit ce que des douanes. N'a jamais ou quasiment jamais été. Peut être sur le tabac. Ce n'est pas tout à fait le cas puisque chaque année, on peut les faire. Les douanes ont introduit à Saint-nombre de réformes. Visant à mieux sans doute lutter contre le trafic de tabac. Mais c'est vrai que sur les autres dispositions le code des douanes est un petit peu daté et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous nous proposerez une habilitation législative pour. Réformer et codifié que des douanes. Donc c'est un travail de compromis. Certains parleront de travail d'équilibre. Pour moi, il ne s'agit pas d'une contrainte je ne partage pas ce point de vue cet équilibre en effet n'est pas une contrainte, c'est la condition même du bon fonctionnement et de la portée opérationnelle des pouvoirs des agents des douanes. Faut-il le rappeler. Cela a été dit, ce projet de loi répond en effet à la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre dernier qui a déclaré non conforme à la Constitution, le droit de visite des agents des douanes et faute d'équilibre cette sans doute l'une des principales prérogatives des douanes qui a menacé, celle qui est sans doute la plus utilisée, la possibilité de fouiller les marchandises de fouiller les moyens de transport de fouiller les personnes cette décisions vous nous l'avez dit lors des 2 éditions, Monsieur le Ministre, la Direction des douanes nous l'a dit et l'a fait sans doute l'effet d'un électrochoc auprès des agents des douanes, mais elle a aussi démontré qu'il était nécessaire à la modernisation du code des douanes. Et donc c'est la raison pour laquelle nous examinons en effet depuis sans doute de nombreuses années. Un projet de loi qui est dédié aux douanes. Certaines dispositions n'ont en effet pas été modifiés depuis des décennies et il apparaît donc nécessaire d'adapter ce code, je le disais à l'instant, y compris aux nouvelles menaces et aux nouvelles technologies. Je vous rappellerai que la commission des finances a donc été saisie au fond de ce texte mais et qu'elle a délégué à la commission des lois et Jean cellule rapporteur l'examen des articles 1 à 5, 8 et 11 je laisserai sur ces articles leur présentation à d'autres collègues, Alain Richard, que je remercie pour notre travail en commun et pour la qualité de nos échanges. Pour ma part je me contenterai de vous présenter la position et les apports de la commission des finances sur les autres articles non délégué tout d'abord l'article 6, l'article 6 crée un dispositif de retenue temporaire d'argent liquide circulant à l'intérieur du territoire lorsqu'il existe des indices que cet argent que cette est lié à une activité criminelle. Je suis très favorable à ces dispositions. Vous l'avez rappelé à l'instant monsieur le Ministre Claude Mougin et moi avions porter cette recommandation, dans le cadre du rapport. Sur la douane face au très trafic des stupéfiants, rapport. Qui faisait suite à des travaux et des déplacements sur le terrain et nous avons constaté évidemment que l'activité et notamment de stupéfiants s'accompagnait du du de la circulation d'argent liquide qu'il était difficile d'appréhender, c'est l'objet de l'article 6. On ne peut pas, en effet, lutter contre les flux illicite si on élit pas en parallèle contre les flux financiers, avec un effet dissuasif plus fort et il existe bien aujourd'hui des procédures de retenue d'argent liquide aux frontières mais il en existe pas pour l'argent qui circule à l'intérieur du territoire national évidemment les organisations criminelles l'ont bien compris et le recouvre de plus en plus à des collecteurs de fonds pour. Sur les territoires qui permettent ainsi la circulation de l'argent, il faut évidemment que cette retenue temporaire soit encadré sur cet aspect. La Commission a précisé que le propriétaire de l'argent liquide. Si il est différent de la personne à laquelle était nidifier l'addition de retenue peut quand même exercer un recours contre cette décision. L'article 13 autres articles sur laquelle la commission des finances est saisie au fond a pour objectif de moderniser le délit de blanchiment douaniers en proposant une triple extension du Champ d'application de cette infraction, il prévoit, premièrement une extension de Chevron d'application territoriale permettant note seulement de sanctionner. Les opérations sur le seul territoire français mais également les activités par transport de mule entre la France et le territoire métropolitain mais sur la Guyane où il existe un fort. Trafic de cocaïne et évidemment du blanchiment douaniers il permettra également de cibler des activités qui portent sur des indications d'origine commises les sur ce point notre dispositif permettra de sécuriser l'article 13. Deuxièmement, l'article 13 étant le périmètre des fonds couverts par le blanchiment doit inclure les cryptoactifs les cryptomonnaies qui sont évidemment utiliser là aussi il s'agit d'adapter notre droit aux nouvelles réalités notamment réalité numérique et troisièmement avec l'adoption d'un amendement la commission toutes les personnes. Intéressées à la fraude pourront être sanctionnés non seulement au titre du délit de blanchiment. Douanier mais également par l'ensemble des délits d'importation et d'exportation. Sur un sujet connexe de lutte contre la fraude, j'insiste, Monsieur le Ministre, sur la nécessité d'améliorer la lutte contre la fraude à la détaxe de la TVA. C'est un point de fuite majeure, la TVA vous allez d'approuver mais il semble que sur la TVA, le gouvernement agit très peu. La preuve, c'est que dans votre plan. Avec développée à grand renfort de publicité sur la fraude le plan fraude. La commission des finances et le rapporteur général ne me contredira pas, nous avons été très d'étonné de voir qu'il n'y avait pas le moteur Donc c'était un peu étonnant, c'est le principal impôt d'après la Commission européenne, c'est l'impôt le plus frauder et le mot TVA ne finit Grey pas dans votre conférence de presse. Il y a d'autres sur d'autres sujets sur lesquels la commission des finances, vous rejoins et c'est le parti de ses préoccupations. Mais la la y compris pour les douanes, la fraude à la détaxe de la TVA fait partie de nos préoccupations. Je poursuis la que l'article 14 qui renforce les sanctions applicables aux trafic de tabac. La commission a considéré que ce renforcement et tout tout à fait opportun tout en veillant à la proportionnalité des peines. Je vous l'avez redit à l'instant 650 tonnes, je crois, vous avez dit de te tonnes saisies en 2002 22, c'est 2 fois plus que que la quantité saisie il y a 5 ans-ce que ça veut dire que les doigts ne sont plus efficaces ou est-ce que c'est une augmentation qui est parallèle à l'augmentation des prix du tabac en tous les cas, il est certain que que de plus en plus d'organisations criminelles. Ce report dans ce trafic est sans doute à leurs yeux, moins risqué, mais tout aussi lucratifs que les stupéfiants et nous soyons pas naïfs, renforcer les sanctions. C'est ce qui ce ne ne permettra sans doute pas d'assécher ce trafic qui augmentera au fur et au fur et à mesure que les prix augmentent en tous les cas, Monsieur le Ministre, vous nous avez présenté un plan du tabac, vous l'avez dit, espérons qu'il porte ses fruits. J'en viens à l'article 7 qui. Porte lui sur le renforcement des moyens des douanes en créant une réserve opérationnelle douanières. faut il y a eu des amendements ce matin. Je crois je vois Éric Bocquet qui va s'exprimer dans un instant. Il y a des amendements de suppression notamment sur le, l'article 7 je ne sais pas si je crois qu'il émane de ce groupe. Bon on va pas se méprendre sur son empereur la réserve opérationnelle c'est 300 douaniers douaniers 300 douaniers d'ici 2025 sur un effectif d'à peu près 16.500 agents donc c'est pas ce qui va révolutionner la douane en revanche. Je pense qu'il faut être favorable à ces dispositions qui permet dans des situations de forte activité dans des situations d'urgence dans des pics d'activité je je pense aux Jeux olympiques par exemple ou à d'autres événements ça permettra sont détourner les douaniers, les agents permanents. Leur mission, d'apporter un renfort qui serait bienvenu. J'aborde maintenant le sujet du numérique. L'article 9 qui permet aux agents des douanes de prendre connaissance et de saisir au cours d'une retenue douanière des objets, des documents qui se rapportent un flagrant délit douanier, y compris lorsque ce document et numérique. Ces informations sont nécessaires aux enquêtes douanières elles peuvent être contenus par exemple des ordinateurs Dell peuvent être contenue dans un téléphone portable et les travaux en commission en lien, je le dis étroit avec la commission des lois permettent de sécuriser le dispositif en particulier pour ce qui concerne la copie des données et la restitution des objets je suis saisie et nous nous sommes rapprochés des garanties qui sont prévues dans le code de procédure pénale, tout en préservant les spécificités douanières. Monsieur le Ministre, j'espère que le gouvernement saura en temps de les deux commissions nous entende sur notamment. Sur ce point, puisqu'il il fait évidemment protecteur des libertés publiques tout en notre pas l'activité des douanes. L'article 10 permet également de procéder au gel des données. Stockées sur les serveurs informatiques et notre mission se satisfait de l'équilibre a été trouvé en commission sur ces dispositions. Les agents disposeront d'un délai de 30 jours

qu'elles occupent en bas donc il se que poseront au téléchargement soit effectivement sanctionner enfin l'article 12, vise à donner une nouvelle prérogative au 12 agents des douanes, mais cette fois-ci pour prévenir la commission d'infractions par l'intermédiaire d'Internet. Donc voilà je pense que pour conclure ses travaux nous ont permis à notre commission de clarifier le dispositif de l'encadrer. Nous avons toujours été. Soucieux de la liberté d'expression et de communication de la jurisprudence et j'espère que les ajustements. La commission des finances seront vous convainc. Monsieur le Ministre. Pour enfin pour terminer et je crois qu'il s'agit de nécessité de moderniser. Je l'ai dit le code des douanes qui est un peu ancien et sur ce point qui est très technique. Nous sommes favorables à cette habilitation législative. On n'est pas favorable par nature mais là c'est c'est un texte très très technique, c'est l'article 15 qui vous permettra sans doute de requalifier la partie législative du code des douanes qui est devenue, nous l'avons dit vous l'avez dit très largement illisible et obsolète. Je vous remercie beaucoup Monsieur le rapport. La parole est à monsieur Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Monsieur le rapporteur. le point que je veux souligner en particulier simplement en ajoutant à cette description très juste du ministre, c'est la très forte évolutivité des techniques et des formes d'intervention de la douane au cours des 20 ou 30 dernières années et ça se poursuit notamment. À cause du développement du du Champ numérique et puis aussi juste un événement politique qui n'est quand même pas dénué d'importance aujourd'hui les douanes exerce beaucoup plus d'intervention au nom du code des douanes de l'Union européenne. Qu'au nom du code des douanes. De de. De la France. Donc ça fait un cadre d'intervention qui a quand même beaucoup changé. Et qui c'est vrai du coup pose le problème de l'actualisation du code. Lequel a. Sérieusement ai. Donc le texte. Le projet de loi qui nous est proposé, poursuit un double objectif, d'une part, mettre à jour. Trouver une conformité les interventions contraignante de la douane avec les droits individuels tels qu'ils sont aujourd'hui interpréter dans les 10 août avec l'évolution récente de la jurisprudence et il faut souligner que la déclaration d'inconstitutionnalité. Que nous avons subi en septembre dernier n'est pas la première. Mais qu'il y a eu d'autres reconnaissance d'inconstitutionnalité de dispositions importantes du code des douanes. Ce qui nous incite évidemment à la à la vigilance. Mais autre composante de ce texte et le ministre a été tout à fait explicite sur la nouvelle dynamique instaurer des mécanismes complémentaires de contrôle pour mieux appréhender des trafics devenu de plus en plus préoccupant.

mais évidemment nous avons développé les propositions consistant pour ce qui concerne la commission des lois consistant à préciser les limites de lieux et de durée des contrôles sur les voix et sur les lieux de transit de la douane et à prévoir l'information et le contrôle de l'autorité judiciaire. Chaque fois que le contrôle appartient le contrôle douanier a atteint une contraint une contrainte importante sur la liberté de mouvement des personnes. Les modalités d'encadrement de ce, de ces interventions contraignante. Nous les avons calquer le rapporteur de Montgolfier l'très bien dit tout de suite, nous l'avons calquer la plupart du temps sur le code de procédure pénale. Pourquoi, c'est le code qui fait l'objet de l'encadrement et de la vigilance juridique la plus importante qui lui-même aussi lieu à des déclarations d'inconstitutionnalité de temps en temps. Donc nous avons vraiment à partager cette vigilance, d'où quelques sujets de d'appréciation légèrement différent avec le gouvernement sur les modalités. Mais il nous semble que nous sommes très près en réalité d'avoir la même la même approche et la même problématique. Les de nouvelles modalités de contrôle sur lesquelles je veux appeler l'attention. C'est en effet le développement de l'accès de l'accès à des données numériques, dans des conditions beaucoup plus intrusif que qu'auparavant mais c'est absolument nécessaire dans une autre fonction essentielle de la douane qui est la lutte contre les mouvements de fonds illicites. Tout ce qui est le le blanchiment. Et puis l'exploitation des vérifications de plaque d'immatriculation qui est en effet un outil de renseignement de de sérieuses qualité. Qui permettrait de repérer les mouvements de transport de stupéfiants de grande de mais qui évidemment du fait que c'est une opération de de surveillance assez généralisé suppose également un cadre d'encadrement et, et comme nous avons choisi une semaine vont parfaitement l'approche de la problématique du gouvernement d'en faire une expérimentation sur une durée de 3 ans qui nous paraît suffisante et représentative. Il y a évidemment ah affiner les conditions d'encadrement et de d'évaluation surtout final de cette expérimentation et puis je j'insiste un instant en terminant. Sur une autre composante. De ce projet de loi qui est l'habilitation qui est demandé au Parlement et que je soutiens. Très fortement pour recodification code. Le code des douanes qui. A une structure qui n'est pas du tout celle qu'on a adopté pour les côtes de la dernière génération et qui est beaucoup plus accessible, je dois dire que par rapport aux principes qu'elle constitue à développer le Conseil constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité du droit. Le code des douanes ne passe pas la barre dans un certain nombre de domaines. Le gouvernement nous a proposé de refaire de A à Z le gros article 60 qui était celui sur le sur les fouilles sur les les visites douanières et. Nous serons amenés sans doute dans la recodification à revoir complètement la structure du code ce sera un gros travail, mais il est indispensable pour que le droit soit effectivement accessible à tous. Je crois que ce le texte tel que nous là. Nous allons proposer en la tient compte pleinement des charges opérationnelles de la douane et nous voulons partager les l'hommage qui a été rendu par le ministre assez personnels qui sont. Reconnues pour leur engagement, leur fiabilité et leur volonté de lutter efficacement contre les délits merci. Merci, merci beaucoup monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à monsieur Dominique Théophile pour le groupe RDPI. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Au nom du groupe RDPI je tiens à saluer le travail minutieux de nos 2 rapporteur en commission qui a conduit à un texte consensuel et équilibré. Ce travail répondait à la nécessité d'encadrer les nouvelles prérogatives des agents de la douane sans entraver leur mission. Le Conseil d'État a rappelé à l'occasion de la présentation de ce projet de loi qu'il était de notre devoir d'assurer. Une conciliation équilibrée la recherche des auteurs d'infractions et la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Et c'est la recherche de cet équilibre qui a guidé nos rapporteur en commission des lois comme en commission des finances un équilibre ou d'autant plus subtil que le code des douanes n'avait pour ainsi dire jamais été réformés depuis 1948. Et la montée de nouvelles formes de fraude et de nouveaux outils au service des délinquants et des contrebandiers impose de recourir à des outils. Plus efficaces et plus puissants. C'est en ce sens. Monsieur le Ministre, que le projet de loi que vous portez est une réforme d'une ampleur inédite depuis 1948. C'est le 1er projet de loi qui propose de revoir en profondeur le code des douanes et de moderniser les outils à la disposition de cette administration et ce n'est pas surprenant que le texte que nous nous apprêtons à examiner soit très technique mais il n'en revêt pas moins une très grande importance dans la mesure où il permet de répondre à l'impérieuse nécessité d'entourer le droit de visite douanières de nouvelles garanties légales pour les personnes contrôlées tout en maintenant le niveau. Même niveau d'efficacité et d'agilité pour les douaniers. Il est urgent d'agir car comme vous le savez, vous l'avez déclaré Monsieur le Ministre, la décision du Conseil constitutionnel est devenu le prétexte fallacieux de certains mal pour contester les procédures douanières. Et cette décision ne nous impose d'agir vite pour rénover le cadre juridique de l'action de la douane avant la date fatidique du 1er septembre 2023 qui a beau Jura l'article 60 du code des douanes dans sa rédaction actuelle. Le texte dont nous débattons permet également d'accompagner la modernisation de la douane qui pourrait ainsi mettre pleinement en oeuvre sa stratégie 2022 2025. À cet égard je rappelle que le gouvernement a doté la DG DDI d'un budget supplémentaire de 148 millions d'euros pour la période 2022 2025. Je souhaite profiter de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer pour saluer l'efficacité Léa le professionnalisme et le dévouement des 17.000 agents des douanes, le travail et leur engagement sont d'autant plus remarquable qu'ils sont mobilisés sur tous les fronts et sont en première ligne face au trafic des stupéfiants. Grâce à ce texte. Les douaniers seront en mesure de lutter plus efficacement contre les trafics de la et la criminalité organisée. Ils pourront notamment renforcer leur présence à la frontière numérique. Dans le contexte de des de développement exponentiel du commerce électronique et de l'utilisation des actifs numériques à des fins de blanchiment d'argent. Le défi à relever est d'autant plus grand que les trafiquants souvent un train d'avance sur les services répressifs. Au fond, je crois, mes chers collègues, que ce texte est un texte consensuel. Tant pour les nouveaux outils qu'qui propose que pour les garanties qu'il offre aux citoyens dans le respect de leur liberté et de leur vie privée. Bien entendu nous avons vu les amendements apportés par quelques-uns de nos collègues aux articles 7 et 11. Certains estiment en effet que la création d'une réserve opérationnelle douanières empêche le gouvernement de tenir la trajectoire de renforcement des effectifs de la douane. C'est oublier que la douane était le seul corps de fonctionnaires en tenue à ne pas disposer d'une réserve opérationnelle et que, par définition ce corps de réserve n'aura vocation qu'à agir comme une force d'appui pour des missions ponctuelles. Ce sera cher collègue. Un outil précieux pour la douane. Quant à l'article 11, il s'agit de des piliers majeurs de la nouvelle stratégie de lutte contre la contrebande aux frontières. Il illustre parfaitement la nécessité de réarmer la douane face à des organisations criminelles de mieux en mieux organisé. Il est bien entendu essentiel de limiter la conservation des données ainsi prélevées et d'encadrer leurs usages mais les garanties apportées par le ministre et de caractère expérimental de la mesure nous permettront de la voter sans arrière-pensée et d'ajuster, au besoin le dispositif Le groupe RDPI votera pour ce projet de loi avec un grand élan. Merci Monsieur Théophile. La parole est à monsieur Thierry Cozic pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui visait initialement à tirer les conséquences de la décision de censure du Conseil constitutionnel, relatives au droit de visite douaniers ce même droit de visite impose l'élaboration d'un nouveau cadre législatif avant le 1er septembre 2023. Vous avez souhaité, Monsieur le Ministre, profiter de ce texte pour moderniser plusieurs points législatifs relatifs notamment aux enjeux de modernisation et numérisation de notre société. Comme les cryptoactifs ou la numérisation des données. Pour ce faire, vous nous présentez donc un texte d'aspect assez technique et opérationnel avec un périmètre relativement limité. Je tiens d'ores et déjà à dire que ce texte va globalement dans le bon sens et qu'il ne suscite pas pour le groupe sert. D'opposition majeure. Souligne néanmoins qu'à l'occasion des des auditions que j'ai été amené. À mener sur le projet de loi avec les organisations syndicales, celles-ci m'ont fait part de leurs inquiétudes quant aux changements structurels. Que ce projet de loi induire. Je tiens néanmoins à porter à votre connaissance les doutes qui émane de l'article 7. Cet article me laisse perplexe. En ce qui instaure une réserve opérationnelle composée de retraités, l'administration des douanes et de volontaires dans des conditions similaires à celles existant pour les autres réserves. Il s'agirait de recruter 300 douaniers réservistes. Et ceci pour un temps de mobilisation de 45 jours la DG délit insiste sur le fait que cette réserve doit répondre à des besoins ponctuels. Cependant, monsieur le rapporteur. Lors de l'examen du texte par la commission des finances, vous avez estimé que cette réserve à permettent de se doter de compétences rares. Ce qui atteste. Vous en conviendrez du flou des perspectives générés par une telle création. Cet article a certes été adopté conforme par la commission. Néanmoins, bien que la douane soit le seul corps de fonctionnaires en tenue à ne pas en disposer à ce jour les interrogations subsistent quant aux réelles motivations président à la création d'un tel dispositif. En effet les activités des douanes sont spécifiques et ne font pas l'objet de fluctuations comparable à celle connue par exemple pour les forces de l'ordre. De plus si l'on peut comprendre la logique de besoins ponctuels lors de pics d'activité récurrent. Je pense notamment aux contrôle aux frontières en période saisonnière. Dans plusieurs parties du territoire ou exceptionnels comme les Jeux olympiques. L'article ne précise pas assez l'émission de ces réservistes. De fait, je m'interroge grandement sur la pertinence de l'instauration d'un tel dispositif qui ne visera probablement à terme qui a justifié une diminution des effectifs ou à tout le moins un gel effectif. Un gel des c'est pour cette raison que je proposerai à cette assemblée, un amendement de suppression de cet article 7. Chat échaudé craint l'eau froide et pour les douanes. Il y a de quoi être échaudé. Je rappelle que le projet de loi de finances pour 2023 à supprimer 680 postes. Après une réduction de près de 1402 1022. Et c'est plus généralement près de 10.000 postes depuis 2017 qui ont été supprimés dans la mission Gestion des finances publiques. Je crains les vases communicants. D'un côté entre la suppression des ETP et de l'autre, la création de cette réserve opérationnelle. Enfin, Monsieur le Ministre, nous avons découvert par voie de presse vos annonces en matière de lutte contre la fraude fiscale que vous souhaitiez intégrée par voie d'amendement. Dans le texte. Je note qu'après des années à nous avoir expliqué que la fraude fiscale était marginal et qu'il fallait se concentrer sur la fraude sociale. Vous prenez enfin la mesure de la problématique. Mais une fois de plus passer des effets d'annonce je doute. Des capacités à vous donner concrètement les moyens de vos ambitions. Alors vous allez me répondre que vous avez créé 1500 postes dédiés à ces missions. Ce chiffre est pourtant peu et cohérent avec la politique générale de cette administration qui vise à supprimer 3000 postes d'ici 2027. À la DGFIP. De fait, on devrait plutôt assister à un redéploiement de postes plutôt qu'à des créations d'être cela paraît peu ambitieux pour atteindre les objectifs qui sont pourtant grandement et notamment pour réponde favorablement à votre annonce visant à contrôler les 100 plus grandes capitalisations boursières. Tous les 2 ans. En conclusion, Monsieur le Ministre. Le et nous appréhendons. Manière plutôt positive. L'arrivée de ce texte. En séance. Mais néanmoins, à la fin de l'examen de celui-ci que nous confirmeront ou non cette position. Merci cher collègue. La parole est à monsieur Éric Bocquet pour le groupe CRCE. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il faut sauver l'article 60. C'est le cri d'alerte envoyée par toutes les organisations syndicales rencontrés depuis la censure du Conseil constitutionnel émanant de la QPC en date du 22 septembre 2022. Sans ce projet de loi le couperet interviendrait le 1er septembre de cette année, plus de droit de visite l'outil des douaniers par excellence, le coeur de leurs moyens d'action. Ce parti Claude, nous y reviendrons dans le débat permet un équilibre plutôt enfin tout en restreignant le rayon des douanes de façon trop important, tout comme l'oubli volontaire des axes routiers et de certains aéroports. Nous aurons des amendements en ce sens pour redonner toute sa vigueur au rayons des douanes et consacrer un droit de visite étendue mais proportionnées au service des agents et donc au service de l'intérêt général. Nous avons bien compris la double volonté du gouvernement qui à ce titre s'inscrit dans la continuité des précédents, à savoir recentrer les activités des douanes aux frontières singulièrement sur l'émission migratoire et aussi gérer la pénurie. Car quand certains s'inquiètent à outrance de l'immigration des personnes. La France est ouverte aux 4 vents aux contrefaçons et autres marchandises nos d'imposer ou non conformes. Drogue, armes bien culturel entre autres, moins de 1% des marchandises acheminées au port du Havre font l'objet d'un contrôle physique. Un entrepôt FedEx par exemple ce sont 100 visite des douanes pour 100.000 colis déposé. Il faut vraiment en France être particulièrement malchanceux pour se faire contrôler par les douanes malgré le dévouement des brigades de surveillance. La tragédie débute avec l'union douanière, instaurée en 1968, puis un marché intérieur absorbé, on a marché unique je cite un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes des services et des capitaux est assuré. Fin de citation. Assurer la libre-circulation c'est faire des douaniers et facilitateurs des échanges. Quid de la douane et des agents dépossédés du contrôle aux frontières. nous étions opposés à cette disposition. Déjà en 1987, et suit le 4 juin 1991 quand notre seul groupe à l'Assemblée avait tenu face aux injonctions de voter favorablement à la création de l'espace Schengen, la France devient le au bout d'une mondialisation incontrôlée et incontrôlable. Les douaniers, comme les usines seraient devenus inutiles comme par magie effacer d'un trait de plume de la carte administrative française. Ce sont ainsi 48,7% près d'un arrondissement sur deux qui ne compte plus un seul agent des douanes. Huit départements ne dispose d'aucun douanier l'implantation territoriale a disparu depuis 1997 alors qu'à l'époque seules 10,69% des arrondissements n'étaient pas couverts. Parmi les nouvelles menaces qu'affrontent les douanes. Monsieur le Ministre, vous en avez oublié au moins une, la disparition progressive de la douane elles-mêmes. Les conséquences sont graves et s'articule autour de la concentration des structures la désertification du territoire et aussi la détérioration des conditions de travail et et du service rendu à la population et à la société. On se résout pas, loin s'en faut, ce problème avec une réserve opérationnelle pour avoir une réserve, il faut que les effectifs soient au complet dans une équipe de football on n'a pas de remplaçant. Si l'on n'a pas assez de titulaire. Notre territoire est exposé à une pluralité de menaces qui ne se limite pas au trafic de cigarettes seules infractions directement traité par l'autre par ce texte à l'article 14, par un alourdissement des peines de prison les 250 milliards d'euros de trafic de drogue international, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le Crime ou les 4,2 milliards d'euros partis en fumette et autres consommations les trafics d'armes pullulent ou encore les trafics de médicaments de contrefaçon. Un fléau déjà mis en avant en 2009 par un chargé de mission de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, je vais le citer les produits proposés ne sont pas toujours des contrefaçons. Il y a aussi d'autres formes de délinquance. Il peut s'agir de médicaments volés ou détournés de charlatanisme ou encore des médicaments qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. La démarche de protection de la santé publique et par conséquent du consommateur est une valeur ajoutée à la protection des marques et des brevets.

nous portons une ambition forte pour les douanes qui doivent recouvrer une place centrale en métropole et réinvestir sérieusement les territoires ultramarins, la France doit prendre toute sa place en Europe dans le contrôle des marchandises et des capitaux prendre sa charge dans la lutte lutte contre tous les trafics, la France ne peut plus être. De biens issus du commerce mondial sans moyen de s'assurer de leur acheminement dans les règles, sans cela et nous n'y voyons aucun signe encourageant dans le texte qui privilégient le numérique au physique le contrôle en ligne au contrôle des marchandises une douane 2.0 a eu le droit ne présente dans tous les territoires. Pour l'heure, nous voterons contre ce projet de loi sourire de l'adoption de nos amendements et de l'évolution positive de ce texte. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Michel à neuf pour le groupe Union centriste. madame la présidente. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues. C'est un texte important que nous examinons maintenant tout simplement parce que le groupe de l'Union centriste, notamment par la voix de Nathalie Goulet, par des amendements nombreux que nous avons pu déposer. Au fil notamment TPLF est particulièrement attaché. Monsieur le Ministre, comme vous, on le sait, à la lutte contre l'ensemble des fraudes et pour cela, bien entendu, il faut qu'il y ait des moyens adaptés. La lutte contre la fraude et quelque chose d'extrêmement important dans notre société société La fraude. Graines complètement la société dans laquelle nous vivons. D'une part. Elle empêche l'État et donc les pouvoirs publics et donc l'action publique de pouvoir disposer d'un certain nombre de moyens et ceci est particulièrement préjudiciable pour tout le monde mais aussi. La fraude, hé bien c'est l'ouverture à toutes les pratiques. Toutes les dérives et on s'aperçoit que finalement. Des dérives il y en a dans, dans le monde entier, dans tous les pays, notamment parce que il y a des trafics de tout genre, que ce soit autour de la drogue bien entendu qui est particulièrement dramatique dans de nombreux pays et cela peut le devenir également en France, mais aussi sur le tabac sur la contrefaçon, Tout ce qui a pour but d'empêcher qu'il y a des relations tout à fait normal entre les uns et les autres et donc il faut que l'on s'attache à ce que. Les choses soient faites dans le bon ordre et on voit bien que depuis de nombreuses décennies, il n'y a pas eu effectivement de refonte de notre code des douanes et il était important de le faire. Ne fut-ce comme vient de l'évoquer. D'autres collègues Bocquet à l'instant par l'obligation de la décision du Conseil constitutionnel mais cela amené aussi à devoir s'adapter aux aux moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui et dont il est indispensable de doter les services des douanes. Alors Monsieur le Ministre, je dois vous remercier de l'initiative que vous aviez proposé que nous puissions aller voir sur le terrain les parlementaires volontaire. La manière dont les douanes travailler je suis pour ma part direction, l'équipe de la direction régionale de la Picardie pour regarder sur l'axe Paris-Lille comment opérer ces agents je dois saluer monsieur le Ministre, le travail qu'il mène. un, dans des conditions qui ne sont pas facile il faut le dire très clairement, parce que le flux de véhicules, le flux d'activité est particulièrement important les moyens dont ils disposent sont parfois assez réduit pour bien appréhender la réalité de ce qu'ils veulent détourner la législation de notre pays mais j'ai trouvé qu'il y avait des agents particulièrement volontaires mobilisés en tout cas très attaché à une bonne réalisation de leur travail et puis c'est vrai que cela s'est concrétisé l'année dernière, cela a été dit par notamment 650 tonnes de trafic de cigarettes. Identifié plus de 100 tonnes de trafic de stupéfiants aussi tout ça c'est à mettre à l'actif de, de nombreux agents qui. Effectuent ce travail sur le territoire national. Alors pour cela. Monsieur le ministre, il faut le dire très clairement, il faut que l'on fasse attention à ce que le périmètre spatiale sur lequel il puisse évoluer. Soit celui sur lequel les trafiquants opèrent on s'aperçoit pour ce qui concerne par exemple l'expérience que j'ai eu l'occasion de vivre. Que la plupart des marchandises arrivent des ports. Je dirais, de Rotterdam et et d'Anvers-notamment. Peut être parce que les services des douanes dans ces. Ports sont peut-être moins regardants sur. Ce qu'il y arrive peut-être aussi que l'importance. Des flux de trafic qui. Y passe explique cette position. Ceci nous amène aussi à nous interroger sur. La capacité de nos installations portuaires parce que l'essentiel du commerce maritime et des du transport de marchandises, effectué par voir maritime. Et bien sûr la capacité de nos ports à pouvoir. Réaliser plus d'opérations de transport, ce qui nous permettrait de mieux maîtriser pour. Nos services. La réalité de ce qui se passe parce que appréhender les choses, de trafic entre différents pays comme. Entre le les pays du sud de la de l'Europe et les pays où sont débarqués l'essentiel des marchandises en Europe, rend la tâche de nos agents particulièrement compliquée.

La fraude à la TVA, il faudra effectivement qu'. Il y ait d'autres volets dans le dispositif qui sera complété à l'avenir pour que nous puissions lutter efficacement contre les les fraudes mais déjà des avancées qui peuvent être obtenus dans ce texte devrait permettre. D'être plus efficient.

par les chefs que j'ai annoncé tout à l'heure. Ceci est tout à fait significatif. Les services de douane m'ont dit que récemment, ils ont pu démanteler 5 ateliers de fabrication de de tabac installés illégalement sur notre territoire. face aux enjeux financiers. Qui en découlent. Eh bien, les opérateurs n'hésite pas à installer des ateliers. A quasiment le faire sur notre territoire aujourd'hui. beaucoup plus en vigilance là dessus et que l'on soit attentif à ce que les moyens qui soient donnés à nos agents pour cela puisse être plus opérant parce que sans cela. Ce type d'atelier va se développer. Fort heureusement, vous proposez que les sanctions soient nettement accentué parce que il n'a pas de raison qu'il y ait des sanctions moindres sur le trafic de tabac. Et que ce soit particulièrement lourd sur le trafic. Des stupéfiants bien sûr sur la lutte contre les stupéfiants encore accentuée. Mais la lutte contre le la fraude au tabac doit l'être aussi et donc. Il faudra sans doute que l'on puisse. Être. Dotés de meilleurs outils pour cela. J'espère que le. Référé-suspension contre le déclin et que vous avez pris le 19 avril. Dernier pour l'utilisation de moyens aériens aéroportée. Sera validé par le. Conseil. D'État parce que là aussi c'est clair que. On prend des dispositions pour permettre de doter nos services de douanes d'outils modernes et puis. Certains, au nom de je ne sais quel. Esprit de liberté attaque ses décisions. Ceci est particulièrement regrettable. Donc il faut qu'. On puisse continuer ainsi. Vous ne demandez également Monsieur le Ministre. Une habitante n'habilitation à refonder le le code des douanes. Nous y sommes au niveau du groupe de l'Union centriste. Bien entendu, tout à fait favorable. Ce que nous souhaitons simplement c'est que. Cette à cette ordonnance face ensuite l'objet d'une ratification. que le Parlement qui confie ses responsabilités à l'exécutif puisse aussi contrôler ce qui a été réalisé par l'exécutif et donc. Cette question de la ratification des ordonnances. Qui se pose de manière générale. Parce que le recours aux ordonnances, ça a été important ces dernières années, doit l'être. De façon plus spécifique là-dessus et que nous puissions effectivement la ratifier. Ceci étant, Monsieur le Ministre, le code, le groupe de l'Union centriste votera avec enthousiasme ce projet de de loi que vous nous proposez. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Stéphane Ravier. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la criminalité en bande organisée dans les méthodes assassinat barbare font grand bruit depuis le début de l'année à Marseille prend racine dans les trafics transfrontaliers de contrefaçon d'armes de tabac et bien sûr de stupéfiants. 21 morts depuis le début de l'année dans la cité phocéenne, des quartiers entiers passés sous un autre droit vivent dans la peur des balles perdues et d'éventuelles représailles de la part des narco-terroristes qui font la loi. Ce texte visant à sécuriser les capacités de fouille des douaniers à alourdir les peines réprimant le trafic de tabac et importante des dispositions pour lutter contres les Go Fast va dans le bon sens. Cependant, il ne change pas la philosophie du problème. d'un rapport de la Cour des comptes de de 2015 pointe très précisément les enjeux, je le cite, il existe une contradiction latente entre la volonté d'assurer la plus grande fluidité du marché intérieur de l'Union européenne et la nécessité de garantir le respect des normes et règles dans les douanes veillent à l'application. La tendance de la commission a jusqu'à présent était de favoriser la libre-circulation plutôt que le contrôle la Commission européenne, encore et toujours ce boulet idéologique qui refuse de prendre en compte la réalité car l'absence de frontières nationales, a engendré de laxisme désordre et ensauvagement les différents élargissement de l'Union ont d'ailleurs pas du tout été pris en compte dans l'évolution des moyens attribués aux douanes, bien au contraire. Le flux de marchandises et de personnes intra et extra européen ayant explosé le besoin en douaniers augmentent fortement. Mais depuis 20 ans la France a perdu 3000 agents, passant de 20.000 à 17.000 douaniers à Marseille, la direction de la doit avoir fait part de ce problème, même en doublant les effectifs sur le port les douaniers seraient ne serait toujours pas assez nombreux pour répondre à l'ampleur des trafics. On entend souvent parler des effectifs de la police nationale municipale et de la gendarmerie jamais ceux des douaniers. Pourtant, si nous avions plus de douaniers, nous aurions certainement moins besoin de forces de l'ordre à l'intérieur du territoire, plus de saisie en amont, c'est moins de trafic en aval sur les 900 emplois promis au moment du Brexit en 2019, il en manque encore. Un tiers, soit 300 ce lundi 22 mai au col de Larche dans les Alpes de Haute-Provence un passeur a forcé un barrage de douane avec son véhicule 12 clandestins ont été découverts à l'intérieur, les douaniers. On le voit jouer un rôle primordial de sécurité avec la police aux frontières. Par ailleurs, le marché de la cocaïne explose dans notre pays en plus des saisies historique sur le port du Havre en 2022, avec 10 tonnes, le port de Marseille-, Fos a connu lui aussi un record avec une tonne 7 de cocaïne saisis par les douanes en France ce sont les douanes qui sont à l'origine de 70% des saisies de stupéfiants. Mais elles sont victimes de la politique du chiffre qui les oblige, faute d'effectif donc à délaisser le Stupp pour atteindre les autres objectifs imposés par les bureaucrates et les ministères. Alors Monsieur le Ministre, plutôt que de communiquer sur les centaines de postes à la DG JP il serait plus judicieux de rendre à la douane sa compétence d'enquête sur les fraudes à la TVA qui représente 25 milliards d'euros et de lui accorder des effectifs dont elle a besoin pour remplir sereinement et efficacement l'intégralité de ses missions. sur aviez. Alors la parole est à monsieur Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE. Monsieur le Président. Madame la présidente de monsieur le ministre. Monsieur le président de la commission des finances. Messieurs les rapporteurs la chers collègues en prise directe avec qui engueulent puis contemporaine, la douane a pourtant une longue histoire.

Droit de traite en. Créé à 1791. Suite au démantèlement de l'ancienne des fermiers généraux. Ce qu'on appelait alors d'abord la Régie nationale des douanes. A joué depuis plus de 2 siècles.

Aujourd'hui, la direction générale des douanes et des droits indirects. Compte un peu plus de 16.000 agents à peu près l'équivalent des effectifs du ministère des Affaires étrangères. Pour un budget d'un milliard 600 millions d'euros par an. Toutefois. chefs de la politique douanière est européenne. Dans le cas de l'union douanière qui est que constitue évidemment l'Union européenne. Ça été dit beuh froid de répandu au sein même de l'Union. Comme en matière fiscale la fraude au Carrousel sur la TVA. Qui consiste à se faire rembourser dans un pays voisin des montant de TVA qui n'ont jamais été acquitté ailleurs. La banque française intègre la lutte comme dans les fraudes et. Intra-européenne dans sa politique dite de renforcement du contrôle aux frontières intérieures de Schengen. Les techniques de froid la paraissent toujours plus sophistiqués et les droits là sont engagés dans une lutte permanente entre la guerre et le bouclier. La situation actuelle se caractérise par une recrudescence des grandes trafics illégaux. Stupéfia tabac et autres produits contrefaits, objets d'art antiquités. Animaux. Également hélas des trafics d'être s'humains ces fut illicite sont d'autant plus difficile à combattre, qui s'insère dans la masse légal dans la masse du fret illégal les rendant moins aisément détectables la numérisation de l'économie, en particulier l'usage de cryptoactifs démultiplie aussi les outils de contournement des contrôles douaniers. Face à ces défis, l'administration des douanes doit pouvoir disposer de moyens d'action efficace et correctement dimensionné.

On a mesure à nouveau la portée majeure de cette procédure, introduite par la révision de 2008 qui permet d'effectuer un contrôle de constitutionnalité à partir. Oui. de la de la rédaction de l'Arctique 60 pouvaient apparaître plus succède. Alors que les charges extérieurs se sont considérablement développées depuis la Seconde Guerre mondiale en même temps que les droits de l'individu et intégration européenne n'est pas. Du contrôle douanier elles sont restées en grande partie jurisprudentielle. Le président pour de loi procèdent à une réécriture en profondeur du code des douanes. En particulier l'article 2 qui remplace à disposition déclarée-ce constitutionnel. Par l'UCI d'. Nettement plus détaillée dont on irait peut-être de. D'aucuns diront peut-être un peu bavard. Cette réécriture. Sera. Complété par une ordonnance qui sera prise par le. Le fondement de l'habilitation d'un article quel dont je propose par ailleurs de réduire le D à deux ans, conformément à l'avis exprimé par le Conseil d'État, quoi qu'il soit, ce projet de loi constitue une base indispensable à la pérennité du 15. L'intervention des agents des douanes le cadre actuel de bananes caduc à compter, on l'a dit, du 1er septembre prochain. Plusieurs modifications adoptées en commission de rapprocher le droit à des visites douanières dans la procédure pénale. Ah oui des conditions comme l'information du procureur de la République, ma collègue Nathalie Delattre propose une série d'amendements visant à préserver les moyens légaux suffisant pour la paix, la réalisation des missions des agents des douanes. Il s'agit toujours d'assurer un équilibre subtil entre les libertés individuelles et les moyens de la puissance publique. La création d'une réserve opérationnelle sur le modèle de l'armée ou de la police. C'est une proposition intéressante pour l'administration dans plus de la moitié des agents sont sous uniforme ne voit, ne faudrait-il pas, ne faudrait-il pas également un renforcement pérenne des moyens matériels et humains de la douane. À l'instar de ce qui est dit dans nos chez certaines lois. En conclusion, les membres du groupe RDSE reconnaissent. Nécessité de légiférer rapidement cette question des douanes et se montreront attentifs au sort des différents amendements proposés avec néanmoins à la vie. Alors a priori favorable pour ce texte. Merci, cher collègue, la parole est à madame Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre. Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. À l'heure où la mondialisation entrent dans de nouvelles phases la frontière représente une limite utile qui permet de filtrer les allées et venues des personnes et des marchandises. La frontière est également un signe d'humilité et de modestie. Comme le souligne Régis Debray. Non je ne suis pas partout chez moi depuis les années 1990, 27.000 kilomètres de frontières ont été tracées et un monde virtuel en est apparu ce qui nous oblige à imaginer des répliques adaptées. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui vise à donner à la douane, les moyens de faire face aux nouvelles menaces il tire également les conséquences de la décision du 22 septembre 2022. Du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la Constitution les dispositions de l'article 60 du code des douanes. C'est la lutte contre la fraude revient à une course historique entre le chat et la souris. Cela ne signifie ni pas qu'il faille renoncer mais au contraire qu'il faut innover pour ne pas se laisser distancer. Grâce à la mise en commun du travail de 3 ministères et par l'efficacité de l'OFAS, l'État enregistré des saisies records de stupéfiants en 2022, au total ce sont 104 tonnes de drogue dont 17 tonnes de cocaïne qui ont été saisies sur le territoire national au Havre sans doute plus qu'ailleurs la douane signifie quelque chose. Véritable porte d'entrée et de sortie pour la France. Le port du Havre est aussi une place convoitée malheureusement par les trafiquants. Ainsi, plus de 7 tonnes de cocaïne ont été saisis. L'année dernière, dont une saisie record de près de 1900 kilos en une seule fois, soit la plus grosse saisie de l'histoire des douanes, selon Monsieur le Ministre Attal. De même, les saisies de tabac comme celle des déchets illégaux de cesse d'augmenter, comme l'illustrent bien la dernière saisie d'avril là encore sur le port du Havre. En 2022, les douaniers ont également intercepté retiré près de 11 millions d'articles de contrefaçon, c'est une gangrène pour notre économie. Pourtant, et malgré leur dévouement nos douaniers sont à la peine. Leur combat quotidien reçu parfois celui de David contre Goliath. Ils vivent mieux que quiconque l'effet ciseaux. Hausse du trafic. D'une part et baisse des effectifs, d'autre part ces derniers. Ayant fondu d'un quart depuis des années 90, ils n'ont pas été compensée par des gains de productivité liés notamment à l'informatique ou à la mise en oeuvre de l'espace Schengen. Les moyens restent insuffisants et les méthodes d'action demeurent limitées par une législation aujourd'hui dépassée tandis que les trafiquants, eux, ne manque ni d'idées ni de ressources tant l'économie souterraine, rapporte dès lors, il est plus que nécessaire de fournir des armes légales correspondant à la réalité rencontrer au Havre comme partout en France. Ainsi la mise en conformité du droit de visite douanière a été l'occasion pour la commission des lois de clarifier les dispositifs comme la précision apportée aux abords des lieux où les opérations des agents des douanes peuvent être conduites à toute heure. Ainsi une définition de la raison de 10 kilomètres autour des ports, aéroports et gares ferroviaires et routières apporte une limite spatiale clair le renforcement des garanties accordées aux personnes a également été un cheval de bataille de la commission en veillant au respect des fondamentaux comme la dignité humaine lors des fouilles individuelle dans le cadre d'exercice des pouvoirs douaniers est également moderniser qu'il s'agisse aussi bien des capacités d'enquête au service de la porte romance dans la lutte contre les réseaux de criminalité organisée ou bien dans la clarification du régime de transfert à l'état de la propriété des objets saisis et non restitués. L'intégration du numérique est au coeur aussi de cette nouvelle approche aussi la copie des données stockées dans un système informatique non implantées sur les 2 visité par les agents habilités illustres de la prise en compte de ces aspects innovants. L'essentiel, le numérique doit être traité avec la même rigueur que les autres aspects physiques et soumis au même examen de nos principes et liberté, un renforcement de l'échange d'informations entre les autorités judiciaires et l'administration des douanes a également été apportées pour la commission des par pour améliorer la coordination et l'efficacité. L'expérimentation des données des Lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation devra être évaluée rigoureusement pour envisager sa pérennisation. Comme pour toute expérimentation et les données conservées conformément aux préconisations de la CNIL non systématiquement au plafond maximum de 4 mois car le juste équilibre entre l'impératif d'efficacité des enquêtes douanières et la paire la préservation des droits individuels a été trouvé dans ce projet de loi. C'est pourquoi le groupe des Républicains votera en faveur de ce texte, telle que modifiée et enrichie par les travaux des rapporteurs. Merci cher collègue. La parole est à Madame Vanina Paoli-Gagin pour le groupe les indépendants. Madame la présidente. Messieurs les rapporteurs. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le pays où le commerce et le plus libre sera toujours le plus riche et le plus florissant nous disait Voltaire par le commerce et notamment internationale la France bâtit sa prospérité. La création de l'union douanière en Europe instaurant la liberté de circulation des personnes, des biens et des capitaux au sein des pays membres constitue un atout majeur pour notre économie. En facilitant les échanges. Nous avons ainsi stimuler la création d'emplois et de richesses. Cette évolution a évidemment profondément modifié le travail de l'administration des douanes. Elle a rendue plus nécessaire encore la coopération avec les services étrangers. Une Europe plus ouverte offre davantage d'opportunités mais présente évidemment aussi davantage de menaces. Il nous faut en effet assurer le contrôle d'un nombre toujours croissant de marchandises et détecter les flux clandestins des marchandises illicites. La contrebande. Cela a été dit est une activité par nature difficile à détecter et à endiguer, a fortiori lorsque les trafiquants emploient toutes les technologies disponibles pour échapper aux contrôles. Nous devons donc veiller à moderniser les outils de l'administration des douanes pour qu'elle puisse continuer à lutter efficacement contre ce fléau. La nature par essence fugace des infractions douanières justifie que la douane soit doté de pouvoirs de contrôle étant étendu. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cela a été rappelé la loi confiées aux agents des douanes le pouvoir général de procéder à la visite. Des marchandises et des moyens de transport et à la fouille des personnes. Cette prérogative général sans limite de temps, de lieu ou de circonstances a été jugé à bon droit contraire à la Constitution. Il nous faut donc désormais bâtir un régime d'équilibre permettant aux douanes d'accomplir leur mission, tout en respectant la vie privée et la liberté d'aller et venir. C'est l'objectif du texte que nous examinons laborieusement mais avec précision il dessine les contours du nouveau régime en organisant le pouvoir de visite douanières en fonction des lieux et des circonstances. Certainement plus technique et plus complexe à mettre en oeuvre ses nouvelles règles répondent cependant aux exigences de notre État de droit. Ce projet de loi modernise en outre les outils de la douane en tenant compte des pratiques les plus récentes des trafiquants. Les paiements de contrebande sont de plus en plus effectuer en cryptoactifs il était donc grand temps de les faire entrer dans le Champ de la compétence douanières. Dans les trafics comme dans la société en général l'informatique occupe désormais une place prépondérante. Plusieurs dispositions de ce texte s'adapte à cette réalité et permettent la saisie de données non seulement contenu dans les appareils des personnes contrôlées mais aussi hébergées dans les nuages de l'Internet. Via leur 16.000 agents les douanes doivent développer des compétences très fine dans des domaines extrêmement variés. Dans ces conditions, la création d'une réserve opérationnelle, nous apparaît particulièrement utile les réservistes cela été dit seront appelés à prêter main forte aux agents lors de surcharge d'activité, il faut en effet s'attendre à ce que les grands événements, que la France va accueillir soit l'occasion d'une augmentation des fraudes. Ces réservistes pourront en outre apporter des compétences rares en tant que spécialiste en matière numérique notamment. Pour entrer pleinement dans la modernité les doivent les douanes doivent pouvoir compter sur les technologies les plus récentes. L'expérimentation envisagée par le projet de loi portant sur les fichiers de lecture de plaque d'immatriculation nous semble à cet égard particulièrement pertinente. Elle permettra d'identifier les convois et de remonter les filières. Si Le monde change vite certaines choses ne varie pas la raison d'être de tous les trafics reste le profit. Notre groupe les indépendants et donc particulièrement favorable à ce que les flux financiers provenant d'infractions soit ciblée. À cet égard, la procédure de retenue temporaire d'argent. Vient combler une importante lacune en confisquant les profits, nous pourrons espérer tarir les trafics. La mission des douanes est essentiel. Cela a été répété, notre pays doit conserver la maîtrise de ses frontières avec des prérogatives modernisés et rendus conformes aux exigences de notre droit. Ce projet de loi, ils contribuent utilement et nous le voterons.

Madame la présidente, monsieur le ministre. Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Ce projet de loi le 1er texte entièrement consacrée à la douane depuis 1965. Ça en fait déjà un texte bienvenue pour ce motif car comme vous Monsieur le Ministre, nous sommes fiers de ce service public qui doit voir ses moyens conforter. La réécriture de l'article 60 du code des douanes déclarée contraire à la Constitution en septembre dernier par le Conseil constitutionnel est indispensable. Cet article concerne le coeur de leur métier, procédé à la visite des marchandises, des moyens de transport des personnes par les agents des douanes en vue de la recherche de fraude. C'est donc un texte essentiel que nous examinons, nous pensons même d'ailleurs qu'il serait possible de créer un code de procédure douanière comme il existe un code de procédure judiciaire. Ce texte procède à des adaptations des pouvoirs douanier au numérique pour mieux appréhender la cyberdélinquance douanières. Là notamment la possibilité de jeunes de geler les données hébergées sur un serveur distant au cours de visites domiciliaires douanières et de sécuriser la saisie des matériels et des notes. Il est aussi proposé de créer un pouvoir d'incitation à la vigilance des opérateurs de plateformes de vente en ligne. Quant aux marchandises disponible sur le site. Autant de défis qu'il faut relever les agents des douanes joue un rôle important dans notre société. Ils sont au centre de la lutte contre les trafics de toute nature protège l'état des acteurs économiques, les citoyens et l'environnement. Toutefois, s'agissant de cette réforme de la procédure et des actes d'enquête réalisée par les agents des douanes habilités notre groupe veillera bien sûr comme chacun à l'articulation. Équilibrée entre des objectifs de lutte contre la fraude douanière et les nécessaires garanties des droits et libertés individuelles et de la vie privée, vous procédez aussi monsieur le ministre à la création d'une réserve des services des douanes sur laquelle notre groupe exprimera justement ces réserves par un amendement de suppression de l'Arctique comme les autres groupes de gauche de cet hémicycle si le recrutement d'une réserve peut apporter un renforcement de forces disponible utile en période estivale ou de surcharge de travail, même si au fond ces périodes de surcharge sont permanentes au vu des échanges commerciaux aujourd'hui les services douaniers sont surtout en sous-effectif aggravées par la suppression de 680 postes aux derniers PLF c'est à cela, Monsieur le Ministre, qu'il faut apporter une réponse et en réformant et en recrutant de nouveaux agents titulaires. Si la France emploie près de 18.000 douaniers l'Allemagne en compte 48.000 à due proportion de la population. La France devrait disposer de 39.000 douaniers par une petite règle de 3 bien évidemment le territoire réguler et bien plus vaste et d'autres critères peuvent entrer en compte. Il n'empêche que nous considérons que la création d'une réserve opérationnelle des services de douanes n'est pas une réponse à la hauteur des défis que vous-même souligné d'ailleurs le recrutement de 300 nouveaux douaniers contre le trafic de cigarettes que vous avez annoncé n'est à l'évidence pas suffisant et sans faire l'oiseau de mauvaise augure. Je ne voudrais pas Monsieur le Ministre, que cette proposition soit en fait un cheval de Troie financier ou budgétaire qui face au cadrage budgétaire sévère que vous souhaitez imposer, créer des réserves dans tous les services publics, professeurs, infirmiers, médecins, en face des baisses de poste titulaire. Il est enfin important de donner des moyens à la hauteur de l'hommage que vous leur rendez. Monsieur le ministre à l'administration douanière. Le manque de moyens de fortes répercussions sur la répression des fraudes mais également des répercussions environnementales que je voudrais évoquer, je pense notamment au contrôle des importations au commerce d'espèces de faune ou de flore sauvages protégées aux conséquences désastreuses et dont pâtissent les écosystèmes mondiaux. D'après des études de l'environnement douaniers de l'OMD, le volume des déchets ont fait l'objet d'un commerce est passée de 45, 6 millions de tonnes à plus de 220 millions de tonnes entre 92 et 2012. Cette augmentation de 500, 102 décennies seulement à des conséquences redoutables pour l'environnement et pour les personnes notamment en Afrique et en Asie Pacifique. En 2019, ma collègue Laurence Cohen avait interpellé le gouvernement sur le risque de contamination aux pesticides des produits importés depuis le Brésil orange café soja massivement importées pour l'élevage industriel, les normes brésilienne autorise 200 fois plus de résidus de glyphosate que les normes européennes. Or, les douaniers ne peuvent rien faire quand la loi est ainsi faite qu'elle permet d'importer en toutes les qualités des substances interdites. La loi Egalim prévoit l'interdiction d'exporter des produits phytosanitaires contenant des substances bannies de l'Union européenne, mais elle ne proscrit pas l'exportation des substances actives même entre janvier et septembre, les autorités françaises ont approuvé 150 demandes d'exportation pour des pesticides interdits sur notre territoire, soit 7475 tonnes de produits fongicides, herbicides ou insecticides. Il faut protéger les consommateurs, nos agriculteurs comme nos industriels contre les importations de produits aux normes environnementales, sanitaires ou sociales incompatible avec les exigences d'un pays comme le nôtre ou d'un ou d'un continent européen qui choisi d'affronter les crises climatiques et sociales, il n'est pas tant de faire une pause sur les normes, les douaniers doivent nous aider à ne pas faire cette pause. Merci monsieur. La parole est à monsieur Jean Yves Le compte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je. Voudrais commencer cette intervention en rappelant que même si l'Allemagne a principalement des frontières internes à l'Union européenne. L à 6000 kilomètres environ 2 pourtour de frontières terrestres et maritimes. Elle a plus de 47.000 douaniers. La France, 23.000 kilomètres de pourtour de frontières terrestres et maritimes principalement hors frontières. Intérieures de l'Union et pourtant. Pas plus de 17.000 douaniers. alors que dans l'Union européenne. C'est surtout les frontières extérieures qui mérite d'être contrôlé pour assurer finalement ensuite la liberté de circulation des biens et des personnes. en commencement de cette intervention que nous devons constater que la croissance d'un certain nombre de trafics et ça a été en particulier évoqué sur le cadet des stupéfiants gangrène à la fois les États et la cohésion sociale. Nous le voyons dans plusieurs pays d'Amérique latine mais nous percevons aussi l'effet de ces trafics aujourd'hui sur. Territoire européen. Ceci doit nous mobiliser. Alors, aujourd'hui, de quoi parlons-nous nous parle finalement d'abord pourquoi ce projet de loi, d'abord parce que l'article 60 du code des douanes. De 1948 n'a pas été revu depuis et a été censurée par le Conseil constitutionnel en septembre 2022 avec compte tenu du coup de tonnerre, que cela représentait pour le fonctionnement des douanes, un report de la censure au 1er septembre 2023. Donc il était absolument indispensable de trouver l'encadrement qui permettait aux prérogatives central des douanes, c'est-à-dire la capacité de fouilles et et de visites. De pouvoir continuer à s'exercer avec un encadrement conforme à la fois à l'état de droit et aux exigences du droit européen. Alors ce texte répond à ses objectifs il adapte aussi un certain nombre d'outils au cybercrime. Et. À l'évolution du numérique et et et répond aussi aux besoins de modernisation des méthodes d'enquête. J'ajouterai parce que bien entendu beaucoup. De douaniers se sont inquiétés de cette censure de l'article 60 du code des douanes et de leur capacité de continuer à exercer leur mission que les infractions douanières par essence internationales doivent pouvoir se faire dans le cadre du droit, du droit européen du droit international et en respectant les engagements de la France, c'est ainsi. C'est ainsi que nous pouvons compter sur des échanges d'informations entre les pays et bien entendu nous ne pouvons pas nous extraire de ce droit européen et notre rapporteur nous là. Alain Richard, nous l'a rappelé tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle construire la confiance entre les partenaires européens et les partenaires mondiaux. Il est indispensable de respecter nos engagements en particulier les engagements européens et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas crier au loup, parce que cet. Article a été censuré. Il convient aujourd'hui de l'encadrer correctement, pour qu'il soit efficace et qui donne toute satisfaction à la fois pour nous-mêmes pour les libertés individuelles et pour nos partenaires et c'est aussi l'occasion, Monsieur le Ministre de rappeler combien cette administration est indispensable et doit être correctement doté, je le rappelais tout à l'heure, l'évolution des douanes allemandes et françaises mais en une année, les effectifs des douanes allemandes ont pris 4000 agents complémentaire en 2022 ce qui est loin d'être le cas de notre administration en France alors que fait ce texte d'abord Il grade les pouvoirs en fonction des lieux et des motifs et les opérations de visite ne pourront plus se pourront ne pourront se faire, pas plus que sur 12h consécutives sur une même zone et le contrôle ne pourra pas porter sur. L'ensemble du public concerné. Deuxièmement, il établit un rayon de douane conforme au code Schengen et enfin troisièmement en cas de d'infractions de droit commun constatée en flagrance, par des agents des douanes. La personne concernée sera remise aux forces de forces de l'ordre sous contrôle du procureur. Ce qui nous sommes des dispositions intéressantes et qui encadre correctement travail donc je voudrais saluer à la fois l'action des rapporteurs et du gouvernement et sous réserve de la question de la réserve opérationnelle, nous soutiendrons c'est c'est. Merci, Monsieur le comte. La parole est à Madame, Catherine Berluti pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission. Messieurs les rapporteurs chers collègues administration de la frontière et de la marchandise, la douane rempli de missions simultanées elle soutient l'attractivité économique du territoire tout en permettant la sécurité de celui-ci et de sa population. Les chiffres de l'année 2022, atteste de l'importance de ces deux missions 104 tonnes, vous le disiez tout à l'heure Monsieur le Ministre de drogue ont été saisies par nos services douaniers pour une valeur de revente estimée à plus d'un milliard d'euros. Et cela sans compter le tabac et les articles de contrefaçon. À l'ère du numérique, l'administration des douanes j'efface un double défi. L'adaptation de ses méthodes d'action a une frontière désormais également numériques. L'intensification des flux illégaux la complexification des pratiques délinquantes et l'. Stabilité de plus en plus forte des réseaux criminels, notamment grâce à l'appui des nouvelles technologies. 2022 a également marqué un tournant dans les prérogatives des douanes françaises. En effet, le 22 septembre dernier, le Conseil constitutionnel a censuré le droit de visite douanières droit qui était autant nécessaire à l'action douanières répressive que potentiellement porteurs d'atteinte aux droits individuels. Le projet de loi répond de mon point de vue à 2 enjeux majeurs dans un 1er temps, il me semble primordial d'éviter le vide juridique que pourrait créer la décision du Conseil constitutionnel en effet le droit de visite dont disposaient les agents douaniers leur permettait auparavant de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, et cela sans limitation ni de lieu ni d'horaires ni de circonstance. La censure de ce droit affaibli l'action douanières et empêche tout simplement l'exercice des prérogatives des agents lors d'un contrôle qui doit rester nécessairement inopiné pour rétablir l'équilibre. Le texte formulées par la commission des Lois du Sénat redéfini 2 caractéristiques essentielles du droit de visite, il restera d'abord, le rayon des douanes périmètre établi à partir des frontières terrestres et du littoral au sein duquel les agents des douanes dispose de prérogatives étendues de contrôle il fait ensuite une gradation en matière des visites en fonction des lieux et des motifs adaptant en conséquence le contrôle exercé par les juges et les garanties offertes aux personnes contrôlées. La visite douanières répond désormais aux exigences de proportionnalité. De l'atteinte au droit d'aller et venir et au respect de la vie privée des personnes tout en associant l'autorité judiciaire dans la recherche des infractions douanières les plus gras. Dans un second temps. Ce texte vise à adapter un code douanier datant de 1948 aux nouveaux enjeux de lutte contre les trafics à nos frontières. L'administration douanière ne dispose pas en effet des leviers juridiques nécessaires pour faire face aux nouveaux usages et des trafiquants et notamment pour appréhender le volet numérique des infractions dans la commission en ligne. De certains délits douaniers ou par le recueil de preuves informatiques par exemple les agents des douanes, non pas à ce jour la possibilité ni de prendre connaissance. Ni de saisir les pièces et documents se trouvant sur un support informatique, ce qui est totalement en décalage avec les enjeux économiques de notre époque. De même, bien que la vente en ligne de marchandises prohibées à l'importance l'importation pardon soit courante aucun dispositif de lutte contre les contenus illicites en ligne n'est prévu à ce jour par le code des douanes. Ce projet de loi vise à renforcer la lutte contre la criminalité en ligne et à moderniser les procédures d'enquête pour mieux prendre en compte la cyberdélinquance qui doit être une priorité de l'action douanières ce texte cherche à y parvenir efficacement pour conclure cette réforme constitue donc certes l'opportunité de doter les douanes de l'arsenal juridique approprié mais aussi de cadrer dès maintenant son utilisation pour prévenir toute restriction disproportionnée de des droits individuels. C'est dans cet objectif que la commission des lois a cherché à clarifier le régime des nouveaux outils dont le gouvernement entend doter l'administration elle précise que les opérations de visite ne peuvent durer plus de 12h consécutives sur un même lieu et que le contrôle ne peut porter que sur une fraction limitée. Du public présent dans cette même optique, la définition d'un rayon de 10 kilomètres autour des ports, aéroports et gares vient se substituer à la référence aux abords de ces lieux notion bien trop équivoque pour être juridiquement acceptable ces ajouts ont un objectif précis, éviter les écueils que provoquerait une autre décision d'inconstitutionnalité du texte des douanes le rôle même des douanes et par nature dérogatoire au droit commun tant il peut conduire à restreindre la liberté des individus néanmoins les enjeux frontaliers de demain sont déjà là. C'est pourquoi ce texte ne visent ainsi pas seulement à corriger nos lacunes passées ou à se conformer à nos enjeux actuels, il cherche à anticiper nos difficultés futures et à donner à notre administration les moyens d'y faire face. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est enfin un Monsieur Cédric Perrin pour le groupe Les Républicains. Monsieur Monsieur le président, Monsieur le Ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Les déclarations d'inconstitutionnalité qui ont affecté le code des douanes ont provoqué une onde de choc au sein de l'administration des douanes. Et pas que. Au coeur des préoccupations de ses agents, comme cela a été souligné à de nombreuses reprises se trouve évidemment la non-conformité de leur droit de visite à la constitution. Cette décision a eu un effet retentissant car elle porte sur une prérogative majeure des douaniers acteur central de la lutte contre les trafics et forces menant tout dans la protection de la sécurité de notre territoire et des populations. La rédaction la réaction pardon de l'exécutif n'a heureusement pas tarder, en dépit d'un certain cafouillage à l'Automne dernier qui avait d'ailleurs été anticipée ici par le Sénat. Nous pouvons a priori espérer qu'un nouveau cadre légal sera bien entrée en vigueur d'ici le 1er septembre prochain. Délai de grâce octroyée par les juges pourtant parmi les douaniers l'inquiétude ne faiblit pas. Je l'ai d'ailleurs mesuré en participant lundi dernier à une opération de contrôle routier à la barrière de péage de de Fontaine dans le Territoire de Belfort nos douaniers mènent des opérations difficiles où les techniques de dissimulation évolue sans cesse et sont de plus en plus sophistiqués. Comme un chef de division divisionnaire des douanes me l'a expliqué les trafiquants ont recours à des caches aménagées parfois élaborés, y compris lorsque les quantités dissimulé ne semblent pas pourtant le justifier. Très récemment, la brigade de Dell, à la frontière suisse a saisi 11 kilos d'herbe de cannabis dans le réservoir d'essence d'un véhicule léger ou encore des centaines de grammes de cocaïne dissimulés derrière le tableau de bord d'une Citroën C3, les moyens de dissimulation se multiplient et concerne tous les types de véhicules, y compris les poids lourds plancher réservoir marchandises caché au milieu du fret légal. De même, les moyens déployés sont de plus en plus important, comme l'illustre la mise en place de convois avec véhicule éclaireur et suiveurs, y compris pour des quantités parfois très limité. Cette manière de procéder. Est également utilisé pour le trafic de tabac. Les agents des douanes sont au coeur des activités régaliennes de l'État. Comment dès lors. Imaginer les douaniers sans prérogative spécifique ça nous rendrait un peu quand même schizophrène. C'est pourquoi nous ne pouvons pas entraver leur action et nous avons le devoir d'aller vite. Ce projet de loi parvient-il à préserver l'efficacité et la simplicité nécessaires, tout en répondant aux interrogations et aux exigences du Conseil constitutionnel c'est le délicat équilibre recherché et trouvé par nos rapporteurs dont les travaux ont été guidée par une volonté très claire, rappeler d'ailleurs à plusieurs reprises dans cette discussion encadré sans entraver. Je me félicite de leur opiniâtreté pour avoir introduit des dispositions déjà promue par le Sénat, à savoir le dispositif de retenue temporaire d'argent liquide circulant à l'intérieur du territoire lorsqu'il existe des indices que cet argent est lié à une activité criminelle tels que le terrorisme, le trafic de stupéfiants ou la fraude fiscale grave. Je salue aussi la modernisation du délit de blanchiment douaniers et en particulier la disposition qui inclut explicitement les cryptoactifs parmi les fonds couverts par ce délit à ce sujet les rapporteurs rappellent le constat du directeur de Tracfin. Les trafiquants ont vite compris qu'il était plus facile de payer en cryptomonnaies qu'en argent liquide. La modernisation et l'adaptation des moyens des douanes aux nouvelles réalités numériques suit cette même logique. Alors que de plus en plus de données sont conservées sur des systèmes de Claude, il est indispensable de rendre possible l'enregistrement des données afin d'éviter leur effacement et ainsi permettre leur exploitation ultérieure par les agents. Là encore nous pouvons saluer l'exigence de nos rapporteurs pour parvenir à assurer la sécurité juridique de ces dispositifs afin de prévenir tout risque d'inconstitutionnalité. Pour conclure, j'encourage moi aussi la création de la réserve opérationnelle douanières qui même modeste, doit permettre de faire face à des situations d'urgence et dernier corps en uniforme de l'État à ne pas avoir de réservistes. Il est très pertinent de pallier à cette lacune qui permettra notamment de conserver des profils précieux car très spécialisés. Je vous remercie. Merci madame la présidente, et merci à à l'ensemble des sénatrices et des sénateurs qui se sont. Exprimés. Je ne veux pas être très long puisque beaucoup des sujets qui ont été abordés. Je les avais abordé dans la déclaration dans la discussion générale et puis on aura l'occasion d'en échanger dans les amendements mais je voulais revenir sur une question importante qui a été. Abordé par plusieurs d'entre vous qui est celle des effectifs. Moi je veux insister sur le fait que des comparaisons faites avec des d'autres pays européens et des pays voisins doivent être faites avec des pincettes, notamment parce que les douanes en tout cas l'équivalent des douanes des homologues de nos douaniers dans ces pays n'ont parfois pas du tout les mêmes missions que nos douaniers. Donc, comparer un nombre d'effectifs dans un pays où l'émission ne sont pas les mêmes qu'en France il y a une certaine limite notamment par exemple pour ce qui est de l'Allemagne. Vous avez comparé les effectifs des douaniers allemands avec les effectifs des douaniers français. J'insiste sur le fait que parmi les douaniers allemands il y en a 8 à 10.000 qui sont engagés sur la lutte contre le travail illégal, ce qui n'est pas une compétence des douanes en France sur le fait que les douaniers allemands ont le statut d'officier de police judiciaire et donc réalise un certains nombres d'émissions qui sont qui sont réalisés par la police nationale en France. Donc il faut vraiment faire attention. De la même manière que pour l'Italie qui était aussi un exemple cité là c'est encore. Autre chose, il y a des missions de police fiscale qui sont réalisés par ailleurs des actions de renseignement fiscal, ce qui n'est pas le cas pour la douane qui a un service de renseignements mais pas celui pas dans les mêmes missions que ce con que ce qu'on constate en Italie, ça c'est sur le 1er point le 2ème point sur les effectifs notamment. Réponse à Monsieur Cozic vous avez insisté sur une réduction du schéma d'emplois dans un récent projet de loi de finances. C'est une réduction du schéma d'emplois qui étaient immédiatement liée au transfert de la gestion et de recouvrement de certaines taxes des douanes à la DGFIP. Donc quand vous transférer le transfert et le recouvrement d'une taxe des douanes à la DGFIP nécessairement les agents qui sont dédiés au recouvrement et à la gestion de cette taxe aux douanes vous transférer les emplois à la DGFIP. il y a un gain de productivité qui a été permis puisque la DGFIP gère beaucoup de taxes et recouvre beaucoup de de taxe et ce gain de productivité, c'est-à-dire la différence entre le nombre d'agents qui étaient nécessaires pour gérer ces taxes à la douane et ceux qui sont nécessaires à la DGFIP est partagé à parts égales avec la douane et donc on a plutôt un renforcement au contraire des agents dédiés à la lutte contre contre les fraudes et enfin le 3ème point. Toujours sur ce sujet-là. Les questions qui ont été évoqués sur la proposition, c'est l'article 7 de ce projet de loi sur la création d'une réserve opérationnelle des douanes. C'est une disposition à laquelle on tient beaucoup et je veux vraiment dire que les autres corps en uniforme qui ont vu une création d'une réserve opérationnelle il s'agisse des policiers, des gendarmes. N'ont pas vu en face. De réduction de leurs effectifs où ça n'a pas empêché qu'on augmente sensiblement leurs effectifs comme on l'a fait ces dernières années sur la police par exemple ou sur les armées comme on va continuer à le faire puisque dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur un renforcement très important des effectifs a été annoncée donc pour être très concret sur ce sujet là. Cette réserve opérationnelle des douanes, elle servira à 2 principaux répondra 2 principaux enjeux d'abord des pics d'activité, ça peut arriver. Soit pour ce qui est un événement très important est organisée sur un temps court, je pense évidemment aux Jeux olympiques et paralympiques pour lesquels on aura un surcroît d'activité pour nos douanes comme pour beaucoup de. De fonction publique, et donc on aura besoin d'un surcroît de mobilisation. C'est par exemple le cas quand vous avez un événement imprévu exemple Océan Viking. Le navire qui accostent sur les côtes françaises. Ce sont les douaniers qui sont mobilisés pour le débarquement, on peut imaginer qu'il puisse y avoir à ce moment-là un surcroît aussi et un soutien qui viennent de la réserve opérationnelle et le 2ème sujet c'est effectivement faire bénéficier à la douane de compétences de pointe sur certains sujets par des personnes qui potentiellement ne souhaite pas changer de métier et travailler auprès des douanes, mais qui veulent pouvoir apporter leurs compétences sur certains sujets. La réserve opérationnelle peut aussi servir à ça, mais évidemment on a beaucoup de compétences et on va continuer à développer beaucoup de compétences de pointe au sein des douanes. Voilà pour les points que je voulais. Clarifier après la discussion générale mais on va avoir l'occasion dans les prochaines heures de débattre de tous les sujets à travers les amendements. Merci, monsieur le Ministre, alors la discussion générale étant Close. Nous passons à la discussion du texte de la commission avec. Un vent l'article. 1er un additionnel qui est l'amendement 17 rectifier bis. Il est présenté par Monsieur Bocquet. merci madame la présidente, monsieur le ministre, dans la lignée de ce que vous venez dire. Vous évoquez la la question des effectifs qui est quand même importante que qu'on le veuille ou non. Vous créez une cellule de renseignement fiscal au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. L'autre annonce que vous confirmez que, conformément au contrat d'objectifs et de moyens de la douane sans équivalent temps plein seront redéployés redéployer, ça veut dire qu'on ajoute pas d'effectif donc on estime, vous estimez que les effectifs actuels sont sont suffisants. Alors les chiffres, il faut quand même en donner quelques-uns. Depuis 97, ce sont plus d'un tiers des implantations douanières qui ont disparu et 37% exactement 48% des préfectures et sous-, préfectures ne dispose plus de services douaniers et dans huit départements de métropole, la douane a purement et simplement alors j'entends bien vos bémol sur la comparaison avec l'Allemagne, mais quand même la France est quand même avant-dernière du classement européen au nombre du bureau des douanes. Au regard de ses frontières, à les 24ème de l'Union Européenne sur 27 quand l'Allemagne est 3ème avec 6 fois et demie plus de bureau de douane par km de frontière au plan démographique, la 2 est le 2ème. Pays d'Europe, il y a quand même un sujet il y a quand même un déséquilibre assez notable. Merci monsieur Bocquet, monsieur le rapporteur. Avis de la commission. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon. Vous connaissez la réponse sur les rapports là la question est pas très favorable, rapport mais au-delà de ça, je ne veux pas éluder la question. L'appréciation des effectifs qui peut se faire par rapport aux autres pays européens avec des missions qui sont différentes. Bon ça c'est le ministre qui est le plus à même de répondent sur les effectifs et il y a en effet aussi l'évolution des missions des douanes et je pense notamment au transfert à la DGFIP mais mais au-delà de ça si je veux faire part d'une conviction plus personnelle que j'ai acquise puisque ça fait des années, des années, des années que je m'intéresse qui sont des douanes, il y a plus de 10 ans. Vous avez été, je peux vous avez témoin pour les membres de la commission des finances. J'étais sans doute doit parmi les premiers à. Soulever la question de la fraude à la TVA étant allée il y a 10 ans, 12 ans à l'aéroport de Charles-de-Gaulle au fret. je m'étais aperçu de l'ampleur de la mission des la faiblesse de la modestie des effectifs au regard des volumes traités il y avait 5 douaniers 5 postiers que contrôler le fret postal. Et j'ai continué à suivre les douanes y compris dans la mission que j'accomplis Claude Mougin, sur le trafic de stupéfiants et j'en ai tiré une conclusion, c'est que les douanes n'étaient pas suffisamment armés technologiquement et que la réponse a été parfois moi dans l'augmentation des effectifs que dans les évolutions technologiques. Je prends un exemple, le frais douaniers. Moi je préfère un scanner qui contrôle 100%. Des marchandises à des augmentations d'effectifs qui ne pourront contrôler que quelques. Paquets malheureusement il en est de même pour les le le fret dans les ports, il en est de même pour le trafic de cocaïne au départ des. Ports de de avec notre collègue nous sommes allés à l'arrivée des avions à Orly. Le les Efic douaniers, permettent d'appréhender trois ou quatre mules lorsqu'on a des dizaines sur un avion. Et ben ça veut dire quoi ça veut dire que je préfère avoir des, des scanners corporels au départ un contrôle à 100% comme le font d'autres pays plutôt que d'avoir des effectifs qui ne pourront pas à cause de la lourdeur. Donc nous sommes dans être enfin ces trafics et des volumes considérables et je pense que la seule question d'effectifs ne suffit pas. Donc cet avis défavorable pour cette raison, la question relevant par ailleurs plus d'une question de d'appréciation des effectifs en PLF. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Avis du gouvernement. Oui merci maintenant le président. Je pense que c'est un amendement qui visait à remettre le sujet que vous avez abordé dans la discussion générale sur les effectifs. Je sais que les sénateurs n'apprécie pas beaucoup les rapports encore une fois j'ai eu l'occasion de m'exprimer à l'instant, ce que je veux ajouter c'est qu'à chaque projet de loi de finances, on a l'occasion d'échanger sur la question des effectifs des douanes et que par ailleurs, un rapport a été remis par la Cour des comptes en 2020 et qui fait le point sur ce que vous évoquez, c'est-à-dire la question des effectifs des douanes et de leurs missions, donc ça me semble satisfait. Merci donc. Je il y a pas de demande d'explications de vote, je mets donc aux voix l'amendement 17 rectifier bis qui a reçu de demande de retrait ou défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Amendement 55 rectifié c'est Monsieur Ruquier qui le dit. L'article 1er du projet de loi redéfinir un Champ d'action de terrestre des douanes. Figurant à l'article 44 du code des douanes. Jusqu'à présent la limite stands d'arrêter de 20 kilomètres en deçà des frontières maritimes et terrestres une distance et qui pourrait être portée jusqu'à. Kilomètres par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances. La nouvelle rédaction prévoit une limite immédiat de 40 kilomètres sans extension possible. Elle n'a pas été modifié en commission toutefois la configuration du terrain aux abords de frontières enfin entraîner des distorsions dans l'application de cette limite, par exemple dans la zone de montagne car fréquents dans les régions frontalières les dénivelés peuvent entrer des distances plus importante que sur un terrain plat ce qui ira à la limite des 40 kilomètres au moins pertinente,

Madame la présidente. Il faut préciser à notre collègue et au président OK que. Nous n'avons pas une liberté complète pour la fixation de ces distances d'intervention et il faut bien préciser que la douane intervient partout. La distance qu'on appelle le rayon douaniers pour simplement sur une zone de sur de surveillance spéciale qui permet des interventions plus général plus plus immédiate de la douane mais la douane intervient partout, dès l'instant où il y a les moyens de démontrer l'existence d'une. D'un risque de fraude et en ce qui concerne donc le chiffre de 40 kilomètres qui est déjà à mon avis le le l'élastique le plus tendu par rapport aux règles européennes. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le la situation des zones de montagne, parce que c'est c'est 40 kilomètres sans compter de façon cartographique ils sont pas du tout compter le long des axes. Mais donc, lorsque vous avez. Comme dans. Une région de montagne que je connais bien, une route qui évidemment fait des kilomètres pour descendre du col. Ça ne change pas la distance d'intervention de la douane, c'est 40 kilomètres mesuré sur la carte donc à vol d'oiseau. Merci monsieur rapporteur Monsieur le Ministre. Oui même avis que le rapporteur. Avec ce projet de loi, on le voit bien, et suite à la décision du Conseil constitutionnel, on doit vraiment réussir à rester dans l'équilibre entre les pouvoirs très importants qui sont donnés à nos douaniers notamment. À la frontière. Et puis la garantie des libertés publiques qui nous a été demandé par le Conseil et de son tout à fait compatibles à condition qu'il y a un encadrement qui soit bien. Prévu comme l'a dit le rapporteur prévoir un rayon de 40 kilomètres de la frontière. C'est un rayon important y compris quand on compare avec d'autres pays. Européens ça n'empêche pas les douaniers de d'exercer leur mission au-delà du rayon de 40 kilomètres. Simplement, c'est un autre régime qui s'applique comme je l'ai expliqué dans la discussion générale. Et je veux insister sur le fait que l'article 5 que le cinq de l'article 44 du code des douanes qu'on ne modifie pas explique que. les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes, donc les problèmes que vous évoquez sont déjà. On a déjà une réponse donc. Demande de retrait.

De la zone terrestre du rayon des douanes. C'est ça. A qui on est compris entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du Rivage de la mer et des rives des fleuves rivières et canaux. À la mer, jusqu'au dernier bureau de douane située à maman, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour du 10. Bureau

Cette loi no 1. Donc à s'assurer que le Champ d'action terrestre des douanes inclut bien les rives de l'estuaire. Vous comprenez qu'il est porté par Delattre, élus de la Gironde, mais que bien sûr, elle fait référence à 30 à l'estuaire de la Gironde. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur. Madame la présidente. Je crois que. Le président qui pourrait également retirer cet amendement Carrier pleinement satisfait. Lorsqu'il y a estuaire. Je rappelle que en droit domanial l'estuaire.

Monsieur le rapporteur. Même avis, Monsieur le Ministre, vous maintenez-vous retirer l'amendement. Merci Monsieur Ruquier le 56 et retiré le neuf. L'amendement numéro 9, il est présenté par Monsieur Savoldelli. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes, mes chers collègues. C'est dans le même esprit que des deux précédents amendements dans le dans cet amendement, nous vous demandions Monsieur le Ministre des temps le rayon des douanes à 60 kilomètres. Au moins temporairement dans une zone de territoire qui nécessiterait alors je suis le débat évidemment et les arguments qui ont été énoncés auparavant mais il faut entendre ce qu'a dit aussi mon ami et camarade Éric Bocquet. C'est que c'est pas un hasard si on est des sénateurs à poser ces questions là du périmètre. Parce qu'il y a quand même 8 départements où il y a plus de douane. Et on est pas loin des 50% de préfectures et sous-, préfectures sans douanier. Donc la question du périmètre est pas qu'une petite question. Voilà et la 2ème chose c'est que on y reviendra, vous l'avez dit tout à l'heure à l'article 7. Avec cette question de la réserve opérationnelle qui devrait faire face à un pic de charges. quand il y a un pic de charges ça suffit là. Ça, ça justifie quand même l'accroissement du nombre de contrôles avec le moins d'entraves possible pour les réaliser les démultiplier dans un rayon plus vaste. C'est pourquoi nous pensons nous qu'il faudrait avoir la faculté de porter le rayon des douanes à 60 kilomètres et c'est le sens de notre amendement. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Et madame la présidente. Je crois que le, enfin le collègue Savoldelli. Tout à fait bien résumé le débat. En réalité, le rayon des douanes est une zone d'intervention. Privilégié sans avoir à démontrer qu'il y a un risque de fraude, ou une suspicion de trafic. Donc c'est une zone d'intervention généralisée, elle doit être limitée pour des raisons de protection juridique et de conformité européenne mais il faut insister sur le fait que dès l'instant qu'ils ont la capacité de démontrer prise d'une suspicion ou lorsqu'ils ont saisi le procureur de leur intention de d'opérer un contrôle sous la forme de la visite douanières ils peuvent intervenir partout donc en réalité nous avons toujours le sujet le ministre il a bien expliqué, il y a 17.000 douaniers. Il y a des trafics multiforme. Certains un espace physique d'autres en espace numérique la bonne distribution de cette ressource humaine rare et très qualifiés ne suppose pas d'avoir trop de délimitation théorique territoriale mais en réalité une souplesse d'utilisation que prévoit l'article 60 que nous allons voir maintenant, donc avis défavorable. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Articles de j'ai une demande de parole de monsieur Oui merci madame. La présidente. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, commission des lois, commission des finances, le rapporteur général, chers collègues. Je tenais à intervenir sur cet article de. Puisque bon représentant un département les Ardennes en frontière avec. La Belgique et dans le passé, j'ai pu connaître réellement l'administration. Des douanes puisque. La maison des parents étaient contre la caserne des douanes à l'époque il y avait je dirais beaucoup de douaniers et et c'était aussi les Ardennes la ville, 7000 habitants à l'époque j'y vais avec les douanes présente ont tout lieu en toutes circonstances. Au plan routier ferroviaire et aussi fluviales avec le fleuve Meuse et c'est important et ce texte est très important parce que il y a l'histoire de la douane qui ont participé aussi largement dans le code du devoir de mémoire également et puis aussi 60 ans qu'il n'y a pas eu de texte, je crois que ça a été rappelé, vous l'avez rappelé monsieur le ministre et puis un certain nombre de collègues. Alors concernant cet article 2. Qui vise la mise en conformité du droit de visite douanières. Et ont en remplacé l'article 60 du code des douanes par 11 articles le dispositif retenu préserve les spécificités opérationnel de la douane et sa capacité de lutte contre les fraudes les trafics dont les stupéfiants. Au territoire national et hors France les tabacs de contre-contrebande la fraude financière les contrefaçons donc autant je dirais de missions qui sont très importantes, et sans oublier puisque cet article a été. examiné par la commission des lois, le lien aussi avec l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, police. Gendarmerie, services de secours, et je crois que c'est aussi un, un lien important qui est fort et je soutiendrai cet article. Merci monsieur la minime et nous passons. Maintenant à la ben la présentation par Monsieur le Ministre d'un amendement du gouvernement. Le numéro 23. Oui merci madame la présidente. C'est un amendement. Essentiellement rédactionnel mais dans la les évolutions qui ont été apportées par la discussion en. Commission. identifie la rédaction de l'article telle qu'issue de la commission identifie moins bien les les finalités du droit de visite et il nous semble important de les repréciser de les clarifier. Dès le départ et donc bien gardé les finalités du droit de visite que sont la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, ça nous semble aussi être un enjeu d'encadrement important. rédaction de de logistique qui n'a pas une énorme importance, nous pensons que les objectifs de la. De la. La visite sont précisé dans l'article 60 tirer hein et et nous reconnaissons d'ailleurs que le gouvernement a très bien fait de remplacer l'article 60 qui était confus par une série d'articles qui énumère les étapes de. De l'opération de visite et nous proposerons d'ailleurs de procéder de la même façon pour l'article 64 qui. Concerne la visite domiciliaire donc il nous semble que c'est bien dans le tirer hein que doit figurer ces objectifs et notamment l'application des différentes législations. C'est donc une différence de conception du de la de la rédaction. Mais pas une différence de fond, donc avis défavorable. Merci monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 23 qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement 24 monsieur le toujours au moment du gouvernement. Oui merci madame la présidente. C'est également. Un amendement qui propose de revenir sur une évolution intervenue en commission qui a. Transformé la notion d'abord. À D apostrophe à bord. Des ports, aéroports et gares ferroviaires par un rayon de 10 kilomètres. Ça a été évoquée, notamment par certains dans la discussion générale où certains ont dit c'est plus clair de mettre 10 kilomètres le problème. C'est que mettre 10 KM ça un sens très différents entre une zone urbaine et une zone qui l'est moins si vous mettez un rayon de 10 kilomètres sur une gare qui accueille des trains internationaux à Paris vous allez couvrir une très grande partie du territoire parisien avec le droit de visite extrêmement étendue et moins encadré entre guillemets des douanes. Par rapport à ce qui se fait habituellement, c'est la première chose, la 2ème chose c'est que la notion d'abord j'ai entendu dans la discussion générale. Une sénatrice. Interrogé le le flou de cette notion, c'est une notion qui existe dans le droit aujourd'hui puisqu'à la fois dans le code des douanes mais aussi dans le code de procédure pénale, la notion d'abord des lieux. Existe existe déjà et donc je vous proposerai de revenir à la notion d'abord plutôt qu'à celle de 10 Seul ministre avis de la commission, monsieur le rapport. Hé bien, madame la présidente de la Commission tient à sa rédaction pour une raison de clarté du droit en sachant que naturellement. Les services de la douane ne sont pas du tout tenu d'utiliser cette capacité. En surface, donc nous préférons la notion plus objective de 10 kilomètres de manière à parer aux obstacles aux risques contentieux d'une différence d'appréciation sur la notion d'abord. Parce qu'en effet il y a des notions d'abord qui existe dans d'autres textes. Mais sur ce sujet là comme nous avons un parallélisme avec la possibilité des contrôles d'identité à proximité. Des ports et aéroports qui prévoit exactement la même limite ça ça capte sa sa sa solidité. Nous préférons cette formule là et bien entendu le débat pourra se poursuivre. Si nous ne vous convainc compare. La discussion pourra se poursuivre dans la navette mais nous préférons prendre la base, la base objective d'une distance kilométrique. Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Vous souhaitiez reprendre la parole. Non, simplement j'entends ce que vous vous exprimez, je veux simplement insister sur le fait que dans l'analyse qui est faite par nos services. Cet amendement pose un vrai risque de constitutionnalité. Et que la réalité c'est que cet amendement il entraîne il entraînerait. Un droit de visite extrêmement. Élargi qui est celui de la zone frontière à 10 kilomètres des gares et des aéroports et donc dans des zones qui ne sont ne peuvent pas être considérées comme des zones de frontières arrondissement de Paris centre, on ne veut pas dire qu'on est particulièrement à la frontière de la France. Donc pour ça on a des vrais. Inquiétudes sur la manière dont le Conseil constitutionnel pourrait considérer cette ce rayon de 10 kilomètres par rapport à la notion d'abord qu'qui y a encore une fois existe dans le code de procédure pénale dans le code des douanes et qui renvoie aux rues adjacentes, des gares et des aéroports. Donc je le dis simplement, pour la clarté des débats avant votre vote. Mais voilà évidemment selon les décisions de cette assemblée on on travaillera dans la suite de la navette parlementaire pour garantir la conformité espérer de ce texte à la constitution. Merci monsieur le ministre je mets aux voix. Cet amendement 24 du gouvernement. Qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour.

Autant de points d'entrée ou de transit de de personnes de marchandises. Cela a été évoqué et non plus simplement sur arrêté du ministre des Finances. Pour information, il est aujourd'hui dans ce pays, 74 points de passage frontaliers aérien depuis la décision de 2017, signée du Ministre de l'Intérieur. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. la zone douanière est une zone d'intervention généralisée qui n'a pas besoin de d'être présente partout. Donc en ce qui concerne les ports. il y a la possibilité d'intervention ponctuelles des douanes sur décision de mener une vie douanières. Mais en revanche il est logique que pour concentrer les moyens le gouvernement choisissent les ports dans lesquels l'activité marchandises et la plus intense toujours pour cette raison de bonne utilisation des effectifs et donc, nous préférons qu'on conserve cette désignation par le ministre des Ports et soumis à la l'intégration à la, au rayon douaniers. Que le rapporteur, Monsieur le Ministre même avis. Je mets aux voix l'amendement 14 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 15. Monsieur Savoldelli. Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre groupe plaide par cet amendement. Pour une intégration des routes nationales et départementales dans le rayon des douanes de façon facultative, dont les tronçons serait déterminé par les ministres chargés des douanes et des transports. Quel constat nous faisons par la fermeture du don de brigade de surveillance intérieure et leur redéploiement aux frontières va marquer un phénomène structurel qui connaît d'après des rencontres pas d'après avec les rencontre des douanes, le tout frontières va conduire à réduire le Jean le Champ géographique d'intervention des services des douanes en restreignant le Champ du rayon des douanes. Peut être, c'est un raisonnement un peu simpliste mais vous mettez dans la peau d'un contrevenant. Dès que vous passez les 40 kilomètres du rayon des douanes vous quitter l'autoroute vous passez sur les axes secondaires ou les départementales vous êtes quasiment certain de ne pas croiser un agent des douanes. Donc, c'est un signal grave un délaissement délaissement d'une partie du du territoire. Et puis avec les procédures de dédouanement simplifiée ou à domicile en suspension de droits et taxes ça devient impossible pour les agents tout opérateur peut être autorisé à dédouaner à domicile à l'importation, il faut simplement que les douanes et agréé les locaux et là si l'opérateur recours une installation de stockage temporaire, jusqu'à 90 jours, il peut même faire l'objet de transfert de lieu de stockage vers un autre sous-autorisation des douanes. Tout ça c'est pour dire et c'est dire si les marchandises circulent avec le. De nombreuses modalités dérogatoires qui leur garantissent une liberté quasi totale. Il faut savoir qu'il existe l'autorisation d'opérateurs économiques qui permet aux opérateurs qui aurait prouvé leur fiabilité de par exemple moduler le taux de contrôle physique et qu'on et documentaire. Donc il faut comprendre moins de contrôles ou quasi plus ou alors la priorité dans les laboratoires de contrôle priorité de traitement de dédouanement réduction des données à fournir. Donc tout ça pour vous dire que nous, nous souhaitons que ne soit pas délaisser les routes nationales et départementales. Merci. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Avis de la commission. nous devons appliquer un rayon des douanes qui est sur une surface frontalière limité. Bien entendu, il reste la possibilité d'intervention sur une base spécifique justifier légalement partout ailleurs. Mais la zone des 40 kilomètres n'prolongé sur les autoroutes que simplement parce qu'on ne peut pas arrêter le trafic au milieu d'une autoroute en pleine voie et que donc l'endroit où peuvent se produire les contrôles. En débordement des 40 kilomètres, c'est le premier. La première halte de péage, vous n'avez pas du tout l'équivalent sur les autres voix et donc. Ce que vous proposez serait d'amener le rayon de 40 kilomètres au territoire entier, donc ça n'est pas le, ça n'est pas l'objectif du projet de loi et je crois que ce ne serait pas cohérent donc propose de le retrait de cet amendement. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre même avis. Et donc. Que vous maintenez l'amendement monsieur Savoldelli donc je mets aux voix l'amendement 15 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté amendement 44. Monsieur Cozic. Merci madame la présidente. Donc la fin de traduire parfaitement l'esprit et la lettre des recommandations émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 septembre 2002. Le présent amendement propose d'assortir l'application de l'article 60 tiré de d'un contrôle judiciaire prévoyant une information préalable du procureur de la République. Cet article a été inséré dans le code des douanes afin de permettre le droit de visite des agents des douanes en cas de raisons plausibles de soupçonner la commission. La commission d'une infraction douanière ou d'une infraction à certaines dispositions du code monétaire et financier. La mise en oeuvre du droit de visite et particulièrement étendu. Il est susceptible de s'appliquer à toute heure et porte sur les marchandises, les moyens de transport et les personnes se trouvant ou circulant sur la loi public ou les lieux attenant directement. Accessible au public, ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains non ouverts à l'international et qui sont situés hors du rayon des douanes. L'information du procureur de la République apporte une garantie de contrôler l'opportunité de le, de l'opération. Cet amendement s'inscrit également dans une démarche d'harmonisation procédural la procédure envisagée par cet amendement prévoit l'information préalable du procureur de la République territorialement compétent s'aligne sur celle prévue au nouvel article 60 tiré trois créé par le projet de loi afin de lutter contre la circulation irrégulière de certaines marchandises sensibles.

de l'application du droit de visite le long d'un le long d'un lieu de transit tout dans dans un lieu de transit. De manière inopinée, par les douanes. Mais à partir d'un d'une suspicion. Crédible une suspicion plausible que la douane pourra justifier en cas de litige. Dans ce cas-là, il n'est pas prévu d'intervention. De la justice parce que c'est le degré le plus limité, si vous voulez, d'intrusion et en revanche, nous le verrons dans les autres articles. S'il y a retenu ou s'il y a immobilisation au-delà d'une certaine durée. Il faudra aviser le procureur en revanche dans l'article suivant, qui le 60 tiré trois où, là, il s'agit de contrôles préventifs sans argument de suspicion plausible. Il y a une autorisation du procureur nous semble donc que votre proposition va trop loin dans la soumission des activités de la douane à la justice, sans que ce soit justifié par la gravité ni des infractions, ni de la retenue. Donc, avis défavorable. Même ma vie. Alors. Je me vois pas de d'explication de vote. Il est retiré donc la demande dans 44 est retiré. Nous passons à la présentation de l'amendement 26, Monsieur le Ministre. Oui merci c'est à nouveau une un désaccord dans la rédaction sur le nouvel article 60 que nous avons avec ce qui a été adopté en en commission des lois et notamment c'est l'objet de cet amendement, le retrait de la notion de tentative, il nous semble, je le dis ici que se retirer la la notion de. Tentative. Est un risque, il est important que le texte s'applique aussi à ces questions de tentative.

avant qu'elle ait commis son infraction sur le motif de la tentative, il nous semble important de conserver cette notion dans l'article 60. Merci. Avis de la commission. Madame la présidente. Cet amendement qui nous est proposé par le gouvernement procède. D'une lecture que nous croyons imparfaite du propre code des douanes que défend le gouvernement. L'article 409 du code des douanes dispose de façon générale pour l'ensemble du code des douanes que toute tentative de délit douanier est considéré comme le délit même. Donc vous avez déjà. Monsieur le Ministre, vous avez déjà dans le code des douanes. La disposition qui clarifie que la tentative et identifié à la commission de l'infraction de l'infraction et donc vous n'avez pas l'utilité de réinsérer des réinsérés de ré-introduire cette notion de la tentative dans les articles spécifiques du code c'est une disposition générale de 409. Explications. Monsieur le ministre. Pour aller au bout de la discussion pour des délits qui sont identifiés dans le code des ou des douanes, effectivement il y a une forme de notions ballet de tentative qui s'y rapportent, mais là on est sur les raisons plausibles de soupçonner un délit. Et donc je vous le dis, il y a l'intégralité de la. Direction générale des douanes et de son service juridique la direction des affaires juridiques du ministère, les, les juristes du Conseil d'État que nous avons sollicité et le secrétariat général du gouvernement ainsi que la chancellerie. Qui considère que il est plus sécurisant de réintroduire cette notion dans l'Arctique. Désaccord avec la commission des lois mais il me semble important de le dire. Merci. Monsieur le Ministre. parce qu'au fond. Après avoir entendu le Ministre je pense que qui peut le plus peut le moins et je ne vois pas en quoi la réintroduction du terme de tentative. Nuit à la qualité du texte que nous présentons si le ministre et des services considère que c'est un plus. Hé bien pour une fois je suivrai le ministre en ayant souligné la qualité du travail des rapporteurs. Monsieur le rapporteur. Vous avez la parole. Il me semble, madame la présidente qui. Nous devons maintenir la proposition qui a été retenu par la commission, mais que si on veut aller tout à fait dans le sens du ministre. La solution est de modifier l'article 409. Merci monsieur le rapporteur. Alors s'il n'y a plus d'explications de vote, je mets aux voix l'amendement 26 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté de façon à quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 27. Monsieur le Ministre, à un moment du gouvernement. Oui c'est un amendement qui immédiatement lié au précédent que j'ai présenté donc toujours dans la même logique. Si. Monsieur le rapporteur. Même avis. Oui ah ben oui ces discussions commune tant qu'on ne s'arrête pas là, on continue les présentations. 59 rectifié c'est Monsieur Ruquier. Merci madame la. Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est l'article 16 du présent article qui prévoit aussi que les opérations de midi douanières. Ne peut être engagée qu'après information du procureur de la République, lequel peut s'y opposer. Ça ne crée les conditions d'autorisation par le 10, procureur de la République, il s'agit d'une limite non négligeables, donner aux douaniers dans l'exercice de leur mission pour le bon nous ramène des opérations il paraît souhaitable de s'en tenir à une simple information du procureur de la République, c'est la vie à cet amendement qui vise à faciliter le travail des douaniers. Oui et quant au point pour que la République. Il va recevoir un flot d'informations ne tous les douaniers. C'est pas sûr qu'ils qu'ils lisent toutes ces informations.

mais qui jusqu'à présent le Champ d'action des douanes n'était pas des coupures dans les départements d'un nouveau cas dans égal il convient de préciser que de quelle zone 0 graphique n'était pas l'opération. C'est pourquoi cet amendement précise que la copie du PV soit transmise au procureur à huit compétents dans la zone de déroulement des opérations de contrôle. Monsieur Ruquier. Nous passons à l'avis de la commission sur ces amendements. Alors madame la présidente, sur l'amendement le premier amendement du gouvernement qui revient sur la notion de tentative qu'il souhaitent inclure dans cet article. Notre position est la même. Donc défavorable sur l'amendement de la présidente de Lattre. Sur la possibilité pour le procureur de s'opposer à la visite douanières. Il va de soi que si on considère comme une.

contraignante pour les pour les particuliers, donc il faut que le procureur et cette possibilité d'interrompre, il le fera naturellement lorsqu'ils voient un sujet de régularité ou de. De l'égalité et avec discernement mais il faut que ce pouvoir. Légal de d'opposition soit mentionnée par la loi. En ce qui concerne l'anonymisation des procès-verbaux c'est une. Réflexion juste de notre collègue Michel même mais il la satisfaction. le le droit à l'anonymisation des enquêteurs qui figurent dans le code de procédure pénale a été étendu au code des douanes et donc cette possibilité d'indemniser d'anonymisation existe déjà, elle est, elle est satisfaite donc retrait en ce qui concerne l'autre amendement de la présidente Delattre qui propose de préciser que c'est le procureur du ressort qui reçoit les informations. C'est c'est implicite. Ça n'est pas nécessaire, par définition la mention du procureur qui reçoit l'information c'est forcément le procureur du ressort du lieu. de pas nécessaire et donc retrait. Merci Monsieur le Ministre même avis alors. Je mets où. Ou hein. L'amendement 27 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement 59 rectifié de madame De Lattre c'est un avis défavorable hein. Monsieur le rapporteur, j'ai bien compris. Qui a reçu un avis défavorable. De la commission et du gouvernement qui est pour.

Donc nous allons mettre aux voix l'amendement de Madame De Lattre le 61 rectifié qui a reçu donc un avis défavorable qui est. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté à un moment 28 monsieur le ministre vous avez la parole. Oui merci madame la présidente. On est ici dans le cas où la douane fait des contrôles sur un opérateur. Agréé. Donc c'est des opérateurs économiques agréé qui dispose du fait de leur activité de facilités douanières de procédure tout à fait allégé pour leur activité. Le texte initial qui vous a été soumis prévoyait que ces contrôles. Puisse démarrer à partir de 8h du matin. La Commission a fait évoluer ses horaires et a prévu qu'il puisse démarrer à partir de 6h 30 du matin, il nous semble que c'est disproportionné on n'est pas là comme dans le cas entre guillemets. D'une perquisition et je pense, je pense que c'était. L'objet et le souhait d'aligner qui était celui de la commission mais on n'est pas dans le cas

et donc c'est peut être pas nécessaire et c'est un peu disproportionné que de prévoir que ces contrôles et lieu. Au tout petit matin et donc on propose d'en revenir à la rédaction initiale, c'est-à-dire un contrôle entre 8h et 20h. Merci monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. L'interprétation du ministre est juste nous avons perçu cet amendement comme enfin cette modification d'horaires comme s'appliquant au pouvoir depuis une visite en général alors qu'il avait un Champ d'application plus restreint et dirigée uniquement vers la la pratique professionnelle. Donc je, je ne peux pas changer la vie de la commission mais je propose de donner un avis de sagesse à cet amendement et personnellement j'entends tout à fait le l'argument du ministre on est on n'a pas cette nécessité pour le cas de la de la visite professionnelle d'aller au-delà de 8h à 20h. Merci monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Richard pour explication de vote. Oui madame la présidente. Monsieur le ministre, je prends la parole parce que je suis à l'origine. De cette. Modification de la durée du de visite décidée par la commission. J'avais effectivement. Proposé une plage horaire semblable à celle de la perquisition. On me dit que. Les agents de douane ne procède pas à des perquisitions, mais des droits de visite. J'ai bien entendu ce que dit monsieur ce le rapporteur. Je suis pas. Convaincu par la notion de. Je trouve que ça y ressemble beaucoup quand même je sais pas convaincu par la notion de surprise. Au-delà de au-delà de 6h du matin ou 8h du matin. Moi, vous l'avez compris, je voulais. Procédé par analogie avec l'article 59 du code de procédure pénale et la Commission avait donné son son accord puisque ça figure dans le texte. On on on on nous dit maintenant que L'amendement du gouvernement que cet amendement accroissant nécessité je lis les atteintes aux droits en retenant des horaires de visite excessif au regard du déroulement des activités professionnelles des opérateurs économiques concernés. Franchement je ne peux pas être d'accord avec ça parce que cet. Article. 63 terre du code des douanes prévoit que l'accès aux locaux professionnels a lieu entre 8h et 20h ou en dehors des 16h lorsque sont en cours, des activités de production de fabrication de conditionnement de transports de manutention d'entreposage ou de commercialisation donc lorsqu'on lieu des activités professionnelles. On on ne peut pas dire que en en. Les les les contrôles pouvant déjà avoir lieu en dehors des heures, on ne peut pas dire que le fait de, d'harmoniser avec. L'article du code de procédure pénale. L'article 59 dont je parlais à l'instant accroît spécialement. Sans nécessité, les atteintes aux droits ou accroît les charges des douaniers puisque ça peut déjà être le cas. Donc, moi, très franchement, je reste sur la position de la Commission et. Le Sénat appréciera. S'il faut faire droit ou non à l'amendement de Monsieur le Ministre.

Je rappelle que le Conseil constitutionnel a censuré l'article 60 du code des douanes. Que si on n'a pas un nouvel article 60 du code des douanes qui respecte les équilibres qui ont été demandés par le Conseil constitutionnel. Le risque qu'on a, c'est qu'à partir du 1er septembre prochain, puisque c'est le délai qui a été fixé fixé par le Conseil constitutionnel. Les douaniers ne plus tout simplement plus agir c'est pour ça qu'on est tous réuni et qu'on soit tous je crois l'adoption de ce texte, ensuite c'est bien légitime qu'on ait des débats sur un certain nombre de modalités qui figurent dans ce texte, on est là, on est là pour ça mais de notre point de vue c'est l'objet des nombreux mois de travail qui ont eu lieu avec le Conseil d'État, les organisations syndicales douanières. Les douaniers du terrain pour trouver le bon équilibre pour garantir que ça passe. Entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets les fourches caudines du Conseil constitutionnel et qu'en même temps ça permet aux douaniers d'agir là où je voulais vous rassurer c'est que il y a évidemment la possibilité de faire ce qu'on appelle l'équivalent de perquisition pour les douaniers s'appelle les visites domiciliaires et là vous avez un régime dédié et notamment ça peut démarrer à 6h du matin parce que. Perquisition, il peut y avoir un objectif de surprendre entre guillemets les personnes chez qui où les acteurs chez qui on seront là on n'est pas du tout sur la même chose. Cette. Disposition là elle, elle porte sur des contrôles beaucoup plus classique de comptabilité par exemple sur la un contrôle de de de comptabilité considère qu'il y a moins de nécessité d'aller à 6h du matin surprendre les les là le secteur en question, c'est pour ça qu'on est toujours dans cette recherche de la plus juste proportionnalité possible pour avoir un équilibre qui garantissent que les attentes du Conseil constitutionnel soit. On a souhaité revenir à ces ces cet horaire qui était prévu initialement. Merci, monsieur le Ministre, je vais maintenant mettre aux voix l'amendement du gouvernement le l'amendement 20. Suite qui a reçu une sagesse de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté. Un amendement et un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur le Ministre. 54.

qui précise les conditions. Nécessaires à la à la mise en Oeuvres du nouveau droit de visite douanières en conformité avec les modalités d'exercice des missions confiées aux services douaniers. Très concrètement. On prévoit dans le texte, vous le savez, que la présence douanière peut s'effectuer avec des vacations de 12h, c'est-à-dire par exemple sur un contrôle sur un auto-sur. Un tronçon autoroutier, les douaniers reste pendant. 12h de cette règle des 12h maximum. Évidemment, les bureaux de douanes et les lieux. Qui sont des lieux où il y a des douaniers qui se sont réunis en permanence avec cet amendement propose d'ajouter à ces lieux où les 12h maximum ne s'appliqueront pas les ports, les gares et les aéroports qui sont des lieux évidemment on a besoin d'une présence douanière permanente. Si Monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. Vous avez la parole pour défendre le sous-amendements à l'amendement 54 du gouvernement. Oui, nous sommes favorables à l'amendement du gouvernement qui est cohérent qui concentre les possibilités de contrôle sur la zone périphérique enfin sur le bureau, lui-même et sur la zone périphérique simplement par cohérence. Nous souhaitons appliquer également la règle des 10 kilomètres, donc nous nous rediscuterons mais c'est la position qui a été adopté par la commission. Donc nous souhaitons avoir aussi autour des des installations permanentes de douane la possibilité de poursuivre les contrôles enfin d'exercer les contrôles. Dans la limite des 10 kilomètres. C'est l'objet du sous-amendement mais nous sommes favorables à l'amendement du gouvernement. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre à vie sur le sous-amendement. Oui, par cohérence avec la vie que j'ai exprimé tout à l'heure on est opposé. À passer de la notion d'abord à celle de 10 kilomètres, je ne peux qu'être opposé à cet amendement je comprendrais parfaitement que par coordination avec le vote précédent le Sénat décide de l'adopter, mais évidemment je précise quand même que c'est un sujet sur lequel on retravaillera dans la navette parlementaire. Alors je vous propose de commencer par mettre aux voix le sous-amendement présenté par monsieur le rapporteur. Le sous-, amendement 65, qui a reçu un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté. Et je mets maintenant aux voix l'amendement ainsi sous-amendé donc numéro 54. Qui a donc l'avis favorable de la commission puisque sous-amendé qui est. Pour.

par exemple le midi des navires qui peut nécessiter le démontage des superstructures m'a plongé dans la durée représentent plutôt à 2 jours. C'est pourquoi il est proposé de remplacer les durées fixé dans le volet Antarctique par la notion non pas de certaines temps comme le le fût du canon met de temps strictement nécessaire aux opérations Fiva la formulation retenue par la Cour de cassation dans sa décision de renvoi au Conseil constitutionnel. Il sera si au juge la faculté d'apprécier la durée nécessaire en fonction des situations concrètes. Si Monsieur Ruquier. Monsieur le rapporteur. Vous avez la parole. Merci à la présidente. Donc. Je crois qu'il y a une incompréhension dans la préparation de cet amendement. Monsieur le Président Ruquier car les durées auxquelles s'appliquent l'amendement de sont pas les durées des opérations individuelles, c'est la durée pendant laquelle. Une équipe de douane ce poste sur un axe sur une ou sur un point de de passage et opère une série de contrôles donc c'est ça qui est limitée à 12h comme le ministre l'a expliqué tout à l'heure et donc cette limite de 12h il faut bien la conserver et d'ailleurs il correspond au rythme de travail des des équipes de douaniers. On ne peut pas maintenir un un contrôle routier ou un contrôle sur la les abords d'un port au-delà d'une. Peine d'une certaine durée, c'est la durée de 12h qui choisit en revanche sur la durée de 4h, c'est la durée, et on y répond dans l'article 60 tiré cette qui vient un peu plus loin. Et si la durée pendant laquelle peut être retenu une personne. Mais. Ça n'est pas une durée qui s'applique à l'ensemble de l'opération de contrôle donc je présume je je préconise le retrait de l'amendement sinon défavorable. Monsieur le Ministre même avis. Vous maintenez votre amendement Monsieur Ruquier OK vous le retirer, il est retiré. Donc le 60 rectifié se retirer, amendement numéro 29. Monsieur le Ministre. Oui merci madame la présidente. Dans sa décision, le Conseil. Constitutionnel a demandé à ce qu'on encadre davantage le droit de visite, notamment pour empêcher je cite un contrôle systématique des personnes et il nous semblait important pour respecter la décision du Conseil constitutionnel d'inscrire dans ce texte de loi qui n'y aurait pas de contrôles systématiques des personnes présentes dans un endroit. La commission a souhaité remplacer cette notion d'interdiction de contrôle systématique par un critère comportemental qui nous semble extrêmement floue juridiquement, qui peut être sujets à divergences d'appréciation. Juridique, il nous semble donc important d'en revenir au terme de la décision du Conseil constitutionnel sur l'absence de contrôle systématique. Je précise qu'il a eu d'autres évolutions de rédactionnel en en commission sur le reste sur le reste de l'article que nous conservons mais sur ce point là, il nous semble important par sécurisation juridique d'en revenir au terme du Conseil constitutionnel. Madame la présidente. Cet argument du gouvernement me paraît solide en particulier parce que cette expression de d'absence de contrôle systématique figurent déjà dans une décision du Conseil constitutionnel, donc je donne un avis de sagesse. Sur ce, sur cet amendement du gouvernement parce qu'il me paraît en effet plus. Que la formule que nous avons adopté. Si monsieur le rapporteur. Je mets aux voix l'amendement 29 du gouvernement qui a reçu un avis de sagesse qui. Pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté un amendement et un sous-amendement qui font l'objet de discussion commune. Un amendement 31 présentée par Monsieur le Ministre, au nom du gouvernement. Oui c'est une précision rédactionnelle suite à une évolution de la commission que nous soutenons et pour laquelle nous voulons apporter quelques garanties. Et je précise qu'on sera favorable au sous-amendement qui est portée par le rapporteur.

Maintenus en immobilisation. Les personnes contrôlées pendant 4h. Il est clair que ceci doit comporter les opérations matérielles de visite c'est-à-dire de fouilles mais qu'en revanche on ne doit pas y inclure la durée du procès verbal parce que le procès verbal n'est pas une obligation. Il est demandé par la personne visitée. Et par conséquent il il faut que la durée pendant laquelle s'appliquent les 4h soit uniquement celle des opérations matérielles. C'est ce que veulent dire l'amendement et le sous-amendement donc je défends le sous-amendement et je propose un avis favorable au gouvernement. Merci. Si. Monsieur le rapporteur. Donc je vais mettre aux voix le sous-amendements à l'amendement 31 du gouvernement donc qui a été présenté par monsieur le rapporteur. Avec un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté et nous passons donc à l'amendement. 31 6 sous-amendé. Évidemment avec l'avis favorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. Le 2 rectifier alors qu'qui le présente. et en fait il, il tente à précisé que les contrôles des moyens de transport qui sont spécialement aménagée à usage d'habitation type les camping-cars. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 64 du code des douanes lorsqu'ils sont en circulation ou provisoirement à l'arrêt sur la voie publique, je précise que l'article 64 d'Edward. Encadre la visite de me domiciliaires douanières est strictement encadrée et ne peut intervenir. Hormis le cas de flagrance que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention. Donc je trouve qu'il est important qu'on puisse préciser. Cette. Cette disposition et comme le disait Talleyrand ça là à ce qui va sans le dire va encore mieux en le disant. Merci madame. Monsieur le rapporteur. Oui comme nous nous en sommes expliqués avec Madame Belgorod ce matin en commission cet amendement est satisfait. C'est-à-dire qu'on a bien inclus dans la rédaction nouvelle de l'article 64. Une limitation au fait que le contrôle ne peut avoir lieu. lorsque le véhicule est effectivement utilisées comme résidence au moment du contrôle, c'est-à-dire lorsqu'il était habité. En revanche, si le véhicule, c'est-à-dire soit le camping-car soit le. La caravane Intercepté en circulation. Il est un simple véhicule et donc le, l'objectif de votre amendement est exactement satisfaits par l'alinéa 29 que nous avons inscrit dans le code. Merci et donc Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, moi je veux je veux vraiment vous remercier, madame la sénatrice. Bé parce que les questions que vous posez, elles correspondent à des. Questions que se posent évidemment les douaniers dans le nouveau régime et a des exigences opérationnelles. Pour eux, et donc comment. Mais vous pourriez tout à fait être douanières rejoint rejoindre la réserve opérationnelle des douanes par exemple que nous allons créer à l'article 7 dont vous serez membre d'honneur. Si vous là si Non vraiment, je confirme ce qu'a dit le rapporteur. Votre préoccupation et est satisfaite mais votre amendement a au moins le le le mérite entre guillemets. Du, d'éclairer les via les débats parlementaires. Une petite question sur ce sujet là mais rajouter une phrase sur le sujet nous semble un peu superfétatoire d'autant qu'on veut vraiment avoir une rédaction ciblées. Bien ce n'est pas parce que vous faites. Cet hommage cet honneur que je vais retirer mon amendement mais en effet je, je souhaite que ça soit vraiment préciser parce qu'on sait combien ce ce midi et difficile et ce texte est aussi là pour les aider et non entraver leur mission.

Il est adopté. Même vote pour l'article 5, il est adopté le 6 même vote il est adopté. Article cette parole de monsieur Laménie. Oui merci. Madame la présidente. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Alors concernant cet article 7 ou qui fait, qui peut faire mais. L'ensemble de ce texte. Et cela a été rappelé, et particulièrement technique mais aussi. Indispensable alors. Cet article 7 vise la création d'une réserve opérationnelle. Douanières. Certes. L'administration des douanes et le dernier corps en uniforme de l'État à ne pas avoir de réservistes et c'est vrai que les réservistes, on les trouve. Historiquement, je dirais au niveau militaire réserve. Opérationnelle au niveau aussi de la gendarmerie nationale. Plus récemment, de la police. Nationale réserve citoyenne également qui existe au sein de la gendarmerie. Mais c'est vrai que après on un certain nombre d'amendements qui visent. À supprimer cet article 7 bon je resterai peut-être plus. Modéré puisque l'objectif est de constituer une réserve de lors de 300 douaniers. Réservistes. En 2025. 2025. Certes. Et. Éric Bocquet. On a parlé et les collègues en ont parlé, c'est vrai que je dirais un certain nombre de départements. Non plus. D'administration des douanes et je crois que c'est la présence reste indispensable. Les effectifs ont malheureusement été réduit au fil des années ce qu'on peut aussi. Regretter alors que sur le budget de l'État on dit faut retrouver des recettes et la lutte contre la fraude entre. L'administration des douanes peut aussi jouer un rôle important et c'est vrai que l'effectif n'est plus que de moins de 17.000. Emplois. Pour l'administration des douanes et ça aussi on, on peut aussi le regretter. Alors que leur mission sur indispensable. Néanmoins je soutiendrai cet article 7 concernant cette réserve opérationnelle douanière. Je vous remercie. Si monsieur Laménie nous passons à l'examen de trois amendements identiques de suppression qui font l'objet d'une discussion commune amendement numéro 1 Monsieur Bruillet. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, on a déjà évoqué cette question au moment du du débat général et je crains que vous ne proposiez ni à moi collègue Bocquet Kosica moi-même d'être membre d'honneur de la réserve puisqu'effectivement nous demandons la suppression de cette réserve. J'ai bien écouté vos réponses. par ailleurs je vous en remercie d'avoir eu la la tension de répondre aux remarques que nous avons formulées. Il n'empêche que je ne comprends toujours pas la justification si ce n'est une justification d'ordre budgétaire pour ce renfort temporaire lorsqu'il y a une surcharge temporaire on peut décider d'augmenter effectivement les moyens mais je considère que les missions de la douane et la difficulté qui est celle des douaniers à remplir. Totalement les missions telles qu'il souhaiterait le faire justifie plutôt le renfort d'effectifs permanents qui permettra d'absorber les les efforts temporaire que vous avez souligné et qui permettra également de donner un peu d'air dans les périodes où ces renforts n'apparaissent. Vous Vous apparaissent moins nécessaire quant à la question des compétences spécifiques. Je dois dire que j'ai été étonné de cette mention parce que si nous avons besoin de compétences spécifiques. Je ne comprends pas ce qui empêche la douane de les recruter, à moins qu'il s'agisse de profil tellement pointue qu'on ait besoin qu'on ait la capacité et d'utilité que sur des opérations extrêmement temporaire. Pour notre part, nous considérons qu'au fond tous les services publics mérite d'avoir les moyens à la hauteur des ambitions qu'on leur donne, je termine juste sur un sujet à propos des réserves près qui existent déjà et du fait que la, la douane est un corps en uniforme, chers collègues. C'est aussi une administration civile et donc la création d'une réserve pour une administration civile

En sachant quand même que le le groupe socialiste par principe n'est pas opposé à cette démarche. Je voudrais quand même rappeler. Plusieurs éléments qui militent pour la notamment pour la suppression de cet, de cet Quitte, Monsieur le Ministre, à ce qu'ils soient réintégrés dans un texte ultérieur et je pense notamment au projet de loi de finances. En 1er lieu, je l'ai dit. Dans la discussion générale. Cette annonce n'est pas articulé avec une démarche pluriannuelle de fixation des effectifs de la DG DDI. années, des années de stagnation des effectifs si l'on raisonne à périmètre constant voire de. De réduction dans l'absolu. La création d'une réserve pourrait se traduire par une par une baisse des effectifs permanente de la direction générale. Cela est d'autant plus préoccupant que le gouvernement est à nouveau engagée dans une démarche de contraction des dépenses de fonctionnement des ministères. Que le groupe sert dénonce par ailleurs. Au surplus. Si l'on peut comprendre la logique de besoins ponctuels lors des pics d'activité récurrents. L'article ne précise pas assez l'émission de ces réservistes enfin monsieur le ministre. Je me permets de vous rappeler qu'il existe au sein de l'administration des douanes. Un service. Qui s'appelle Paris spécial. Qui, aux yeux des syndicats des organisations syndicales en particulier assume efficacement les missions de renfort. Qui aujourd'hui justifie à vos yeux. la création de cette réserve citoyenne. Je crois que pour l'ensemble de ces raisons. Aujourd'hui les réflexions ne sont pas assez abouti et donc je vous propose. La suppression et de leur envoyer dans un texte ultérieur, qui sera présenté au Parlement. monsieur Cosic et nous terminons avec l'amendement 10 présentée par Monsieur Bocquet. Oui merci. Le président aurait également pour le groupe communiste. Un amendement de suppression de cet article 7. Nous considérons que c'est quand même un signal extrêmement négatif envoyé aux agents des douanes. C'est une c'était une singularité qui était réservé aux aux chants militaires ou à la police à la seule exception de la réserve civile pénitentiaire qui n'était composée que de retraités de l'administration pénitentiaire des volontaires les retraités des douanes seraient engagées au même grade que pendant leur carrière alors qu'ils ne connaissent pas les services les volontaires pourrait briguer dégradent extrêmement élevé dans la hiérarchie et notamment celui de directeur des services douaniers par exemple. Comment ne pas y voir ici une inégalité flagrante. Après une vie d'engagements au sein des des des services douanes pour les anciens agents et plus encore, reconnaissez quand même qu'après avoir décidé de reporter l'âge de la retraite à 64 ans. Cette disposition est un peu particulière. Vous aviez déjà créé une réserve opérationnelle en catimini par amendement lors du projet de loi de finances pour 2022 et voilà que vous réitérer que le service public en tension. C'est l'expression à la mode nous entend leur tour viendra et vous leur proposerait de créer une réserve opérationnelle qui s'apparente à une espèce de d'armée de réserve d'autres observateurs estiment que cette proposition de création d'armée de réserve opérationnelle c'est aussi une façon de contourner les règles budgétaires de la LOLF. C'est 300 apprentis douaniers volontaire ou retraités mobilisés à raison de 30 journées permettent de respecter le schéma d'emplois en tenant compte du plafond d'emplois soumis lui au vote du Parlement. Or non seulement un réserviste et moins coûteux. Je mets ce terme entre guillemets, parce que c'est le jargon siens pour parler comme vous qu'un agent des douanes mais surtout sa rémunération mais son équipement n'auront pas d'impact sur les plafonds d'emplois vous pourrez donner l'impression de faire mieux avec moins. Mais vous ferez moins bien avec plus c'est ainsi perdre comme cette volonté de contourner les dépenses nécessaires au bon fonctionnement des missions régaliennes assuré par les douanes. Merci. Merci cher collègue. Nous passons à l'avis de la commission sur ces trois amendements identiques. Monsieur le rapporteur. À cet examen en séance. J'ai évidemment interrogé aussi bien le gouvernement, le ministre, la Direction des douanes. Et les arguments. Bon, pour le coup convaincu. Alors il y a les compétences techniques. C'est vrai, là je pense que c'est le ministre, il est le plus à même de répondre sur ce qui a été évoqué je j'entends, c'est quel type de compétences pourraient être. Nécessité d'avoir recours à la réserve. Je suis assez sensible à cet argument, mais j'étais surtout sensible à l'inciter des renfort ponctuel leur notamment de grands événements. Alors vous avez évoqué. Dire, vous avez dit certains. Peut être est-ce prématuré. C'était un sujet de PLF. Et je pense que dans les fonctions que j'ai occupé, en moto, membre de la commission des finances, je préfère en effet que les. Problèmes d'effectifs se voit en PLF bon néanmoins il y a un événement par an pour l'année prochaine

exerce. 62 cas ça ne poste. Frontière d'aéroport des missions de police de l'air et des frontières, ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie qui dans certains aéroport assure ses missions dites de la PAF de la police policière aux frontières,

et c'est la seule force en uniforme qui par rapport à la police, gendarmerie, n'est pas aujourd'hui l'armée n'a pas aujourd'hui de réserve, donc c'est la raison pour laquelle c'est une demande de retrait défavorable sur ces trois amendements qui tendent à la suppression de la réserve. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente. Oui, je m'inscris Direct vraiment dans ce qu'a dit le le rapporteur. Il s'agit absolument pas d'imaginer que la réserve. Opérationnelle. Et vocation à substituer des réservistes à des agents titulaires S'ils interviennent les réservistes. Ils sont sous l'autorité des agents titulaires. C'est c'est c'est ça n'est pas à la place de l'autre. 2ème chose. On a vu se développer des réserves dans tous les autres corps en uniforme. Si le fait de créer une réserve dans un corps en uniforme entraîner une absence. De d'accroissement d'effectifs, ça se serait vu c'est plutôt l'inverse qu'on a vu. Effectifs de la police de la gendarmerie ont été très fortement renforcé ces dernières années, alors même qu'une réserve a été créé créé 3ème chose vous avez abordé monsieur monsieur Cozic le dispositif Paris spécial les spé, comme on dit, pour le coup, ça n'a rien à voir parce que là ce sont des agents douaniers titulaires qui simplement accepte, il y a des. Compensations du coup indemnitaire notamment de pouvoir être mobilisés entre guillemets au dernier moment, parfois sur des missions ou de manière plus temporaire sur des missions ailleurs, là on est sur une réserve, c'est-à-dire des gens qui ont un autre métier mais qui, s'ils en ont la possibilité et le temps et qui a un besoin exprimé par les douanes parce qu'il a un surcroît d'activité parce qu'il y a un événement imprévu ou parce qu'il y a un événement qui justifie davantage de moyens qui peuvent venir apporter un soutien et sur les compétences qui peuvent venir aussi renforcer les douanes. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs sujets qu'on a identifié. Par exemple, on a beaucoup parlé ici de de la nécessaire modernisation sur les sujets Intelligence artificielle ou crypto-. Si il y a des personnes qui travaillent dans le privé, qui sont des spécialistes des cryptomonnaies mais qui ont envie, sur leur temps disponible de pouvoir aller aider le le service public et l'État en apportant leurs compétences aux douanes pour développer des. Attends c'est les accompagner sur ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'on les en empêcherait. On peut plutôt les accueillir, il faut qu'il puisse le faire. Sur un certain nombre de situations aussi. Au niveau Naval. On a les garde-côtes des douanes qui sont des marins, mais il peut arriver que sur certains sujets à certains points très spécifique. On a besoin là aussi d'un coup de main d'un renfort qui peut venir de l'extérieur et donc moi je je je ne comprends pas pourquoi on empêcherait à des Français qui ont un travail, qui ont envie de servir leur pays et l'état quand ils en ont la possibilité d'apporter leurs compétences, de le faire, c'est vraiment l'objet de cette réserve opérationnelle. Merci, monsieur le Ministre. S'il n'y a pas d'explication de vote je mets aux voix ces trois amendements identiques hein c'était disque reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés. Nous passons à la présentation de l'amendement 70 monsieur le rapporteur. Au nom de la commission des finances. Si la commission et est favorable à la création de la réserve opérationnelle, encore faut-il que cela soit encadré en permettant notamment administration des douanes de procéder à des enquêtes pour cession avec le comportement incompatible avec les missions et donc c'est l'objet de cet amendement et je précise que si disposition qui est similaire à celle qui était en vigueur pour les réserves de la police nationale. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. Favorable je mets aux voix l'amendement 70 de la commission qui a reçu un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est compte qui s'abstient il est adopté le 71 monsieur le rapporteur, toujours au nom de la commission hoc. Rédactionnelle. Favorable et donc je mets aux voix le 71 qui a reçu un avis favorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient est adopté. Je me vois l'article 7 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient-il être. Adopté je mets aux voix l'article 8. Même vote il est adopté. Article 8 bis même vote adopté article 9 E 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 48, monsieur Richard, monsieur le rapporteur. Oh non, commission des lois. le projet de loi propose d'insertion dans le code des douanes d'un nouvel article 323 11. Dont le paragraphe 3, vise à permettre aux agents des douanes lorsqu'une personne et demie remise en liberté à l'issue de la retenue douanière de procéder à la copie des données informatiques détenu par la personne concernée. Donc il s'agit pour le gouvernement. Et on le suit de permettre la continuation de l'enquête douanière même lorsque la personne contrôlée n'est pas poursuivi. Ce procédé qui est tout de même extensif comme droit de contrôle par rapport au droit commun puisqu'il s'agit de prendre les données de quelqu'un qui n'est pas poursuivi pénalement. Il nous semble que ça doit être l'objet d'une autorisation du procureur de la République et donc nous rédigeons cet amendement, précisant le le droit d'aller chercher les données particulières privée d'une personne qui a été contrôlé par la douane mais non poursuivi doit faire l'objet d'une autorisation écrite et motivée du procureur. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. Non pardon, pardon monsieur, mais je fais une bêtise. Nous sommes en discussion commune. Excusez-moi. Et donc c'est le 58 rectifié de Monsieur Ruquier.

au. Romain mais sur autorisation du procureur de la République afin de donner aux douanes et moyennes exercer pleinement leur mission de recherche des auteurs d'infractions en, il va falloir constitutionnelle cet amendement. Donc c'est un peu l'inverse la commission. Remplace l'autorisation du que la République par une simple information de ce dernier.

le 48 c'est un avis favorable en revanche c'est un avis défavorable pour le 58 qui propose cet amendement de substituer non pas une autorisation à une simple. Une simple information pardon à une autorisation. Ça ne paraît moins pour protecteur en terme de libertés publiques et soit les personnes et je vous rappelle que c'était à l'issue. De la retenue, soit la personne est remise en liberté dans ce cas-là, il faut évidemment avoir l'autorisation du procureur et si après les gardés à vue pour le coup, il faut l'autorisation. Ça pose d'elle-même, donc avis défavorable. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. Oui, avis défavorable sur les deux amendements. Y compris sur celui du rapporteur. On est ici sur les cas où il y a saisi exploitation des données du téléphone pendant une retenue douanière. je fais un cas très concret. Vous avez une personne qui est d'interpeller qui est mise en retenue. Douanière parce qu'on a constaté qu'elle. Était responsable d'une infraction douanière. Ce texte donne la possibilité aux douaniers dans le cas de cette retenue douanière d'exploiter les données sur son téléphone, ce qui peut être très utile parce que potentiellement on peut vouloir regarder très vite si la personne a un complice qui potentiellement voyager avec était pas très loin et si on peut éventuellement savoir assez vite qui est ce complice, je donne un exemple. Comme garantie d'encadrement dans le texte on prévoit que les douaniers pourront exploiter les données de son téléphone après autorisation du procureur, ce qui déjà mais quand même un encadrement et une étape pour. Les douaniers. La nouvelle rédaction qui est proposé par le rapporteur prévoit que cette autorisation du procureur devra être écrite et motivée. Et moi j'alerte vraiment sur les la conséquence opérationnelle pour nos douaniers. Y compris la chancellerie avec laquelle on a échangé nous a dit qu'il s'inquiétait que les parquets se retrouvent noyées entre guillemets sous des procédures où ils devront à chaque fois faire une autorisation écrite et motivée à chaque fois pour que les douaniers dans le cas d'une retenue douanière puisse exploiter les données d'un téléphone. Donc on a tous envie que les douaniers puissent. Faire leur travail de manière la plus efficace possible. Il y a déjà un encadrement, puisqu'il faut déjà une autorisation du procureur, et donc il me semble important qu'on s'en tienne à ça et qu'on ne rajoute pas que cette autorisation doit être écrite et motivée. Merci, monsieur le Ministre, je vais mettre aux voix l'amendement 48 qui a reçu un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement. Qui est pour.

Les opérations de saisies feront déjà l'objet d'un procès-. Verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisés et d'une copie de ce procès verbal à la personne placé en retenue douanière. Je le dis parce que. Cet amendement a pour objet d'ajouter le propriétaire des supports saisissent il est différent de la personne retenue ou des représentants comme destinataire du procès-verbal retranscrivant les opérations saisit Elles feront déjà l'objet du procès verbal transmis au procureur de la République et donc l'ajout sera une contrainte supplémentaire pour les agents des douanes dans le temps limité d'une retenue douanière c'est un temps qui est. Qui est qui est qui est limitée, donc il nous semble. Pas opérationnel de rajouter cette précision donc avis défavorable. des applications retirer au vu des explications du gouvernement. Si monsieur le rapporteur. L'amendement 72 et retirer 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 33. Monsieur le Ministre, au nom du gouvernement. Rédactionnelle. Rédactionnelle et le 73 monsieur. De mongol. Moi je le gouvernement de le retirer au profit de l'amendement de la commission le 73 qui est défendu. D'accord. Alors.

avons. Il nous reste donc après l'amendement 33 du gouvernement qui vient d'être retiré. Le 73 à mettre aux voix avec hein donc. L'amendement de la commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il était adopté. Je me vois l'article 9 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté après l'article 9. Nous avons 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 3 rectifier bis.

Même en cas de flagrant délit, les douaniers doivent donner au juge les motifs précis pour justifier de leur arrestation. Or. Bien souvent l'arrestation ne repose pas sur des éléments manifeste est évident mais sur des suppositions. De plus, les motifs précis justifie à l'arrestation. Ou le placement en retenue douanière doivent être transmis à la personne concernée. Or, cela a un effet contre-productif pour l'action de la douane française puisque les prévenus peuvent transmettre les motifs de leur arrestation à d'autres malfaiteurs. Il semble donc suffisant d'informer la personne de la qualification de la date et du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commises. Merci cher collègue. Nous avons un 2ème amendement discussion commune le 4 rectifié bis monsieur Moga. Merci. Donc c'est un amendement. Qu'on peut considérer de repli cet amendement vise à ne pas transmettre les motifs de l'arrestation et du placement en retenue douanière à la personne concernée. Si cher collègue avis de la commission sur ces deux amendements.

donc les amendements qui visent soit à assouplir les conditions de placement sous en retenue douanière soit à supprimer l'obligation d'information, c'est le cas du deuxième au moment du cannabis. pris émission de l'obligation d'informer la personne des des motifs. De la retenue. Ça ne paraît pour le coup être dangereux et ça pourrait sans doute présenter un risque constitutionnel donc ça doit être à mon sens encadré et c'est la raison pour laquelle.

Je les retire madame président. Merci monsieur Moga ces deux amendements trois et quatre rectifier sont retirés. Nous passons à l'article 10. À sept. Cet amendement en discussion commune. Nous commençons par le 49. Monsieur Richard au nom de la commission des lois. Alors a mais la présidente, il y a 2 aspects dans cet amendement, le 1er putain simplement une remise en forme. Car je souhaite signaler au gouvernement et à l'Assemblée que le dit amendement le dit article 64, sur lequel nous travaillons comporte simplement 49 alinéa. Donc il est extrêmement difficile de maniement et mon amendement consiste à simplement comme ça a été fait justement pour l'article 60. À propos de, du droit de visite là c'est sur le droit de visite domiciliaire que le process et les conditions légales de déroulement de cette procédure soit organisé en plusieurs articles mais nous avons par ailleurs un sujet important qui est que dans le cas de décision de Perquis de ce n'est pas une perquisition. C'est une visite domiciliaire, or la la grosse. Cette décision est prise par le juge des libertés. Et de la détention n'est pas une décision policière ou douanière. Dans le cas de la flagrance. La proposition de la Commission et que, il lui est information du procureur et que par conséquent il puisse s'y opposer. Ça nous paraît être le minimum qu'on peut mettre pour une mesure aussi contraignante qui est la visites domiciliaires inopinées. Avec donc un droit de fouille intégrale et une retenue des personnes concernées par là au domicile. Il nous semble que ceci doit faire l'objet d'un encadrement judiciaire minimal qui est l'information du

Une annulation constitutionnelle alors qu'il y en a eu d'autres sur le code des douanes. Il faut prendre cette précaution et donc. Il est l'information du procureur. Donc c'est l'objet de cet amendement. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre, pour la présentation de l'amendement 64. Oui je l'ai je le retire au profit des amendements, 74 et 75 du rapporteur Gaultier. Merci Monsieur le Ministre, l'amendement 64 et retiré long patient la présentation du 74 par monsieur de Montgolfier au nom de la commission des finances. La maintenant c'est un amendement de précision et le 75 de coordination. Merci. Si. Le 50 rectifier bis de monsieur Richard au nom de la commission des lois.

Il s'agit de transposer aux visites domiciliaires fiscale les dispositions on vient d'adopter pour les visites domiciliaires douanières Il s'agit toujours de, d'assurer l'équilibre entre le droit d'intervention de la douane, le droit de, de, d'entrée de façon très intrusive dans les documents et dans le, dans les lieux privés. Avec un encadrement judiciaire minimale.

Et nous passons donc maintenant à l'avis de la commission. Peut être des finances pour commencer. Merci à vous en.

et de ce point de vue je partage. Nous avons échangé avec Alain Richard le le fait que ça aurait mérité d'être un peu un peu mieux ordonné donc ce jeu. En revanche l'amendement 49 à un petit peu au-delà parce que. Ça a été dit à l'instant, est-il notamment il modifie le cas de la visite domiciliaire en flagrant délit.

plus d'expérience pratique sur la manière de se déroule. Des opérations douanières notamment la visite domiciliaire sur le. Cinq puisque les reste ce sont des amendements. donc sur le 50 rectifié bis donc. Cet amendement qui réécrit l'article L 38 du lit des plusieurs fiscal que relative aux deux visites domiciliaires des douaniers en matière fiscale et là c'est une demande de retrait. Parce que l'adoption de cet amendement me semble, il me semble qu'il remettrait en cause vite significativement pardon les prérogatives des douanes dans le travail de recherche d'infractions de nature fiscale. Alors ah mais, mais c'est vrai que les douanes interviennent en matière fiscale notamment pour les contributions indirectes et donc des réserves. Notamment. En particulier sur la question des systèmes de données à distance les serveurs, les Claude en anglais et donc pour cette raison. C'est une demande de retrait sinon un avis défavorable, ça doit être que le gouvernement saura nous apporter plus de précisions sur la manière de se déroule très près de manière pratique, ces visites domiciliaires. Merci beaucoup. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. je crois qu'on est tous guidés par le même objectif c'est à la fois de tenir compte des exigences du Conseil constitutionnel pour avoir un texte qui est conforme à notre Constitution et en même temps garantir l'efficacité opérationnelle pour nos douaniers qui souvent doivent agir dans l'urgence et avec la plus grande efficacité. Possible à partir de là on peut avoir des débats qui sont bien légitime. Et et c'est pour ça qu'on en débat ce soir donc je vais tout de suite donné les avis et je ne veux surtout pas que ça soit perçue comme. Une évolution politique de ma part. Évidemment, on est vraiment sur le sujet du fond des amendements mais je serais favorable aux amendements de Montgolfier est défavorable demande Alain Richard. Je vais m'en expliquer dans un instant tout de suite. L'amendement qui est proposé par le rapporteur. Richard. D'abord, il vise il réécrit entièrement le dispositif et je je le dis par ailleurs. Indépendamment du sujet sur lequel je veux dire je vais venir, qui est celui. De. De l'information du procureur de la République. Je pense qu'il y a des choses utiles dans la réécriture que vous proposez notamment une plus grande clarification. La création de subdivision etc et je pense que ce sera utile qu'on reprenne aussi cela dans le cadre de la recodification qu'on souhaite faire. Du texte pour autant. Ce, cet amendement prévoit. Que. Les visites domiciliaires suite à flagrant délit. Ne puisse être conduite qu'après information du procureur de la République qui peut s'y opposer. Je crois que c'est une évolution qui serait très lourdes et source d'un risque opérationnel pour les opérations douanières. D'autant que la réécriture complète du texte. Généra une forme d'insécurité si on si on ne si on ne vérifie pas immédiatement ce que ça implique. Je veux préciser que le flagrant délit qui soit douanier ou non requiert une action en urgence et que l'amendement risquerait de fragiliser l'information du procureur nécessite de ménager un délai permettant à ce dernier de s'y opposer. Et donc cette procédure me semble. Incompatible avec les situations visées dans lesquels la rapidité d'action pour collecter les informations nécessaires à la caractérisation des faits et tout à fait décisive du point de vue des parquets cette information en flagrance sera une source. Que nous jugeons d'encombrements inutiles pour les services de traitement en temps réel du parquet qui recevront des appels ou des mails pour les prévenir de cette visite domiciliaire alors même qu'une mesure est très actif de liberté n'est pas en cours et que la procédure douanière n'est pas suffisamment avancé dans bien des cas pour caractériser une infraction pénale justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. Cette évolution je rajoute n'est pas juridiquement nécessaire parce que la proportionnalité de la procédure n'est pas en risque dès lors que l'article 64 du code des douanes prévoit déjà La présence d'un officier de police judiciaire de que la procédure n'est applicable qu'à des délits douaniers passible d'au moins 3 ans d'emprisonnement. Trois qu'elle ne peut être réalisé que le jour même où si le flagrant délit est commis après 21h le lendemain. Et IV le contradictoire, c'est-à-dire la présence de la personne ou de de. Témoins, donc ce serait un frein opérationnel et c'est d'ailleurs déjà largement satisfait en en pratique le souci encore une fois de d'encadrement parce que compte tenu des investigations à conduire après la constatation du flagrant délit, les agents des douanes le plus régulièrement place en retenue douanière les uns fracture. Or le régime de la retenue douanière suppose nécessairement l'information du procureur de la République dès le début de la mesure par tout moyen. Donc c'est. À la fois un risque opérationnel et les les les préoccupations qui sont les vôtres me semble déjà satisfaite par tout ce qu'il y a en en amont, ça aboutirait à avoir un régime plus contraignant que celui de la procédure pénale parce que l'introduction d'une information préalable du procureur de la République, avant le déclenchement de la visite revient à introduire des garanties qui irait au-delà de celle qui existe dans le code de procédure pénale, même si on a eu pas mal de débats sur ce sujet là, je sais que vous en êtes en désaccord. Pour les perquisitions effectuées pendant l'enquête de flagrance pour lesquels aucune information du procureur n'est prévue. Très complexe pour les agents des douanes la visite domiciliaire en flagrance fait partie des prérogatives de contrôle auquel les agents des douanes sont très attachés au regard de son efficacité opérationnelle. Une évolution restrictive ne serait donc pas comprise par les agents alors qu'il s'inquiète. De la rédaction du droit de visite au terme de l'examen parlementaire. Il me semblait important. Pour les débats que nous avons de préciser tous ces points là. Merci monsieur le ministre je monsieur le rapporteur. Je crois qu'il est utile de poursuivre un peu le dialogue puisque précisément nous légiférons. À la suite d'une déclaration d'inconstitutionnalité du fait que les. Capacités d'enquêtes et de mesures coercitives de la douane n'étaient pas suffisamment encadré. Il me semble. Discutable. Monsieur le Ministre. De dire que la proposition que je fais dans cette afin que la commission des lois fait dans cet amendement. C'est-à-dire que le procureur souhaite visée et qu'ils puissent mais pas nécessairement préalablement qu'il puisse à tout moment. S'opposer à la procédure serait excessif par rapport à ce qui se passe en matière pénale, en matière pénale, le code de procédure pénale prévoit que le procureur contrôle tous les actes de. d'enquête et d'instruction qui sont faits par le. Les officiers de police judiciaire et naturellement, c'est le cas de la près de la perquisition. Donc dans le cas de la perquisition en droit général il y a bien. Autorisation et contrôle du procureur. Il me semble que de laisser passer ce texte sans corriger ce risque constitutionnel qui figure sur le le droit de perquisition douaniers en réalité c'est bien de ça qu'on parle est une imprudence et je crois préférable de maintenir cette disposition qui permet au procureur simplement d'être informés de s'informer pour savoir quelles sont les infractions qui sont poursuivis et Monsieur le Ministre, vous avez dit vous-même que ça ne peut s'appliquer que lorsque sont poursuivis des infractions d'une gravité supérieure à trois au moins égale à 3 ans de prison. Donc ce ne sont pas des dispositions banal. Il me semble donc logique que le procureur exerce un contrôle minimal d'opportunités sur ces perquisitions qui sont quand même des mesures très très intrusif dans la vie privée et je crois donc. Il vaut mieux retenir ces dispositions. Merci monsieur. Sur le rapporteur je vais mettre aux voix l'amendement 49 rectifié qui a reçu, c'était un avis du gouvernement, donc le gouvernement est défavorable. Même avis. Non non je j'ai dit on est on est partagé. Parce que. Les salles, j'entends bien ce que dit à Alain Richard. Mais l'aspect opérationnel il y a des aspects personnels qui sont. qui me voilà le le qui me gêne, je prends l'exemple de la saisie de marchandises. Ça veut dire que toute saisie de marchandises qui est quand même une opération assez courante. Des sinistrés. J'ai bien compris aussi.

le PJ me paraît déjà une première garantie et dès lors qu'on est sur d'autres procédures à l'à ce moment-là en effet, le procureur a été visé par tout moyen donc je vois là j'étais. Je je. Je, je ne voudrais pas qu'on n'ait un changement révolutionnaire, bon je, j'entends bien, je ne mesure pas à ce stade moi je serais plutôt pour suivre l'avis du gouvernement, ce serait plutôt un avis défavorable mais je le ministre-ce veut peut-être nous apporter des précisions. Monsieur le Ministre, si vous pouviez nous préciser votre avis. Pour répondre au rapporteur Richard mais on est sur des sujets très importants donc je pense que ça justifie qu'on est clair. La discussion du. La décision du du Sénat dans le code de procédure pénale, on prévoit bien que ces perquisitions en flagrance se font sous le contrôle du procureur. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une information préalable du procureur. Ça veut dire qu'il y a un officier de police judiciaire qui est présent pendant l'opération, qui rend des comptes à l'issue. Ou à la justice. Bien évidemment c'est ce qui est aussi prévue par le code des douanes. S'agissant des sujets dont on parle ici il y a bien un officier. Judiciaire qui apporte les mêmes garanties et qui rend des comptes au procureur à la justice ensuite. Mais le fait qu'il disait dans le code de procédure pénale. L'expression que c'est sous le contrôle du procureur ne ne ne ne veut pas dire qu'il y a une information préalable. Ça veut dire qu'il y a un officier de police judiciaire qui est là pour, à l'issue de l'opération, rendent des comptes à la justice qui est le cas aussi de ce qui est prévu pour, pour les opérations douanières. Merci Monsieur le Ministre. Donc je vais mettre aux voix l'amendement 49 rectifié qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas Z opté amendement 74 de monsieur le rapporteur de la commission des finances, qui a reçu un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il. Adopté. L'amendement 75. De monsieur de Montgolfier toujours qui a reçu un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. L'amendement 50 rectifié bis. Qui a reçu un avis. Amendement 76. De monsieur de Montgolfier au nom de la commission des finances favorable du gouvernement qui est pour. Olivier. Contre, abstention il est adopté de 69 de la commission des finances avec le même avis favorable pied pour contre, abstention, adopté. Article 10 je le mets aux voix qui est pour. Contre. Abstention, adopté article additionnel après l'article. Ah oui j'alors il est Il est 8h, je vais donc suspendre l'ASEAN celle sera reprise à 21h 30 pour la suite de l'examen de ce texte. La séance est suspendue.